La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Nous n'avons pas reçu d'observation. Il y en a-t-il en séance. Je n'en vois pas un procès-verbal et adoptée sous les réserves d'usage, monsieur le 1er ministre. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement notre séance est retransmise en Direct sur publie. C'est là et notre site internet, chacun sera attentif au respect des uns et des. Autres et au respect du temps de parole. Je vais donner la parole à notre collègue Jean-Louis Lagourgue pour le groupe, les indépendants, république et Thierry. Vous avez la parole. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, en l'espace d'un mois la réunion aura connu 2 épisodes cycloniques particulièrement intense, avec pour conséquence principale de sérieux dommages pour les infrastructures agricoles du territoire alors que Lille se trouve dans un contexte économique très contre, en raison notamment de la persistance de la crise sanitaire, le passage du cyclone Batsirai il y a quelques semaines, puis M. ce week-end, a plongé le monde agricole de la Réunion, dans une nouvelle situation inquiétante. Les pertes se chiffrent au jour tué à plus de 47 millions d'euros à l'échelle de l'île, ce sont près de 1000 hectares qui ont été ravagés par la violence de ces cycles. Derrière ce chiffre se cache évidemment des pertes de revenus et de trésorerie des exploitants des exploitants dont les finances sont déjà très tendu. Face à la situation, l'État a répondu présent, ceci et mérite d'être soulignée par l'intermédiaire du ministre des Outre-mer qui a déclenché rapidement la procédure de reconnaissance de catastrophe naturelle, je salue cette réactivité du gouvernement, en espérant que l'ensemble du territoire, soit les 24 communes bénéficient de cette reconnaissance de calamité agricole, cependant, il est à mon sens indispensable que l'État aille plus loin dans la démarche en mettant en place des mesures d'aide complémentaire qui permet au monde agricole de panser ses plaies et de le relever rapidement à la tête de souhaiter donc savoir, Monsieur le Ministre, si une suite favorable sera accordée à la demande des agriculteurs réunionnais de pouvoir bénéficier par exemple d'une prolongation des mesures liées à la COVID, comme le péage ou de la mise en place d'un fonds d'aide exceptionnelle d'urgence, je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Outre-mer monsieur Sébastien Lecornu vous avez la parole monsieur le Ministre. Merci monsieur le président du Sénat, mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, la gorge était effectivement il y a quelques jours à la Réunion, faisant suite au cyclone Batsirai et malheureusement un 2ème cyclone a frappé l'île de la Réunion et cette partie de l'océan Indien et fort heureusement, il faut démarrer par là. Il n'y a pas eu de victimes parmi nos concitoyens, il n'y a pas eu de victime mais les dégâts matériels sont importants et vous l'avez souligné ce sont les agriculteurs qui payent le tribut le plus important à ces catastrophes climatiques votre question était donc Direct je répondrais de manière très directe sur les agriculteurs, nous allons faire 4 choses la première des choses, Monsieur le Sénateur, c'est de réduire tous les délais d'instruction, on le sait, classiquement, il faut un an nous allons ramener ce délai à 5 mois ce qui sera le maximum de ce que les services de l'État s'affairent en lien avec la Chambre d'agriculture de votre territoire pour instruire les différents dossiers, la 2ème des choses, c'est que je viens de valider le déclenchement du fantôme, le Fonds de secours outre-mer pour 20 communes à la Réunion, les autres communes vont être étudiés prochainement, ce qui va nous permettent de déclencher, c'est la 3ème chose le l'ensemble des procédures de calamité agricole dès le mois de mars, dans un délai donc particulièrement réduit et, enfin, par rapport à votre question sur les problèmes de trésorerie avec Julien Denormandie, Olivier Dussopt, nous allons passer des instructions aux différents organismes collecteurs de faire preuve de bienveillance sur les différentes échéances pour les cotisations sociales ou un certain nombre de rendez-vous fiscaux pour permettre à ces exploitations de passer ce cap et enfin oui nous allons maintenir les prêts garantis par l'État pour les agriculteurs de la Réunion pour leur permettre de passer ce cap de trésorerie qui va être difficile, la solidarité nationale et là, nous le devons à l'ensemble des lyonnaises et des Réunionnais et à leurs agriculteurs, en particulier. gauche. Donner la parole au président Roger Karoutchi. Pour le groupe Les Républicains.

il y a quelques mois, le président de la République, lance un ultimatum au Liban. Le Hezbollah, tenu par l'Iran, répond non, il ne se passe rien. Il y a peu de temps, l'Arménie. Nous demandons, nous exigeons le retrait des forces des milices turc Erdogan dit non, il ne se passe rien. En cours. En Afrique, nos troupes courageusement ont lutté contre les jihadistes aujourd'hui les milices russe. De Wagner sont là. Le Mali, Tchad, Centrafrique et les gouvernements africains nous demandent de quitter les pays en question. Il y a quelques jours, le président de la République négocie avec Vladimir Poutine pense obtenir une désescalade. Les troupes russes envahissent immédiatement le Donbass et menace le reste de l'Ukraine. Alors Monsieur le ministre, est ce que vous n'avez pas le sentiment que, face à des gens qui eux ne respectent pas le droit international, le simple respect de ce droit ne nous affaiblit pas. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge des affaires européennes Monsieur bonne. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, Karoutchi. Peut-être pourrions-nous avoir sur ce sujet dans la gravité du moment qui nous réunit un peu de responsabilité et un peu de hauteur que le monde qui nous entoure soit dangereux et difficile, c'est un fait que la France ne puisse en décider autrement, c'est une réalité, je crois que le bilan que vous avez tracées de manière partiale et partielle ne reflète pas tout à fait la réalité des choses d'abord nous avons à chaque fois pris les responsabilités qui étaient celles de la France, le président de la République, en tête depuis 5 ans, quand le président Trump est sorti de l'accord de Paris, c'est la France, avec ses partenaires européens qui a sauvé cet accord qui a permis qu'ils survivent jusqu'à la réintégration des États-Unis, quand la crise sanitaire nous a frappé dans tous les pays du monde, c'est nous qui avons pris l'initiative de faire du vaccin bien public mondial de nous protéger par l'initiative européenne quand il y a eu des crises internationales, le président ne s'est jamais dérobé, quel que soit le moment, quel que soit le contexte et les campagnes de certains à ses responsabilités, il y a pris des risques, c'est ainsi que se fait la la politique internationale, si on vous avez écouté, je pense notamment à votre collègue, Monsieur Jacob, l'Assemblée nationale, qui disait qu'il fallait dialoguer plus avec Monsieur Poutine, il y a 15 jours, nous n'aurions rien fait, nous avons le plan de la République l'a fait, il a tenté cette chance : fallait-il en faire autrement, je ne crois pas que les choses soient compliquée, nous n'avions aucune naïveté à cet égard, mais regardez ce qui s'est passé de manière plus profonde, vous me permettrez de prendre l'exemple européen, la France était de retour, la France a été efficace, nous avons permis d'avoir un plan de relance européen qui a sauvé notre économie, nous avons permis d'avoir un plan de relance européen qui a préservé l'Europe nous avons agi toujours nous occupe aujourd'hui dans la crise qui nous occupe aujourd'hui, ne vous en déplaise, l'unité et la fermeté internationale, nous l'avons construite, c'est la France, vous nous l'avez réclamé qui a pris les initiatives ces derniers temps, c'est la France qui a pris en effet ses responsabilités pour essayer de construire cette réponse, alors on peut dire que le monde n'est pas dans une situation facile, je crois qu'il serait difficile de l'imputer la responsabilité auprès de la République, nous avons toujours pris nos responsabilités et un exemple qui me tient à coeur et qui vous tient à coeur aussi, Monsieur le Président, Karoutchi, celui de l'Arménie, en particulier, vous pourriez saluer les résultats qui ont été obtenus ces dernières semaines par l'engagement du prendre la République notamment au sommet du Partenariat oriental en décembre avec enfin la libération d'un certain nombre de prisonniers reconnaissez au moins avec honnêteté les avancées quand elles sont là. Monsieur le Président, Karoutchi. Vous voyez, Monsieur le Ministre, je vous parle de problèmes de fond vous remettez ça sur le président de la République, moi je ne suis pas en campagne, elle. Je vous dis, je vous dis, je vous dis simplement face à face, non, mais les milices. Ils ne sont pas sincères réagir dans cet hémicycle, non, mais peut-être que vous êtes au Parlement, vous n'êtes pas dans votre bureau. Mais je je vous dire, je vous dis simplement. Je vous dis simplement que face à des pays comme l'Iran, comme la Chine, comme la Russie, comme la Turquie qui ne respectent pas le droit international qui ne respectent pas les règles du multilatéralisme de l'après-guerre, hé bien nous sommes faibles pas. Nous vous nous. Tous les Européens, certains pays, les Kurdes, les Arméniens, les le, le Liban, les pays africains comptent sur une Europe forte, sur un pays fort, hé bien changeons de politique en France et en Europe pour être fort. Merci, la parole. C'est à notre collègue François Bonneau pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors que l'Est de l'Europe semble sur le point de s'embraser. Je voudrais d'abord avoir une pensée comme nous tous, pour les Ukrainiens, pris depuis 8 ans dans cette spirale de violence au mépris du droit international. La France, quant à elle, ne peut penser que ce conflit n'aura aucun impact sur elle. Le risque est particulièrement grand en matière énergétique. Notre pays comme les autres pays européens et dépendante durablement du gaz russe. Il faut donc se préparer à une rupture d'approvisionnement que cette rupture soit voulue ou subie. Avec 2 conséquences potentielles. Premièrement, en cas de rupture totale un épuisement nos stocks de gaz. Deuxièmement, encadre rupture partielle une répercussion rapide sur le prix de l'électricité en Europe. En effet, vous le savez, Monsieur le Ministre, le prix le électricité sur le marché européen se base principalement sur le prix du gaz. Si les relations venait à se distendre encore. Alors ce conflit armé, pourrait avoir un effet majeur sur l'économie française sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens, déjà très entamée par l'inflation récente. Monsieur le ministre, le gouvernement a-t-il envisagé l'impact de telles sanctions vis-à-vis de la Russie. à-t-on une stratégie dans l'hypothèse où ce risque se réaliserait. Sur le plan européen, peut-on découpler une bonne fois pour toutes, le prix du gaz, du prix de l'électricité, enfin, comment comptez-vous gérer les possibles pénuries de gaz et d'électricité à venir. On vous répondre, la parole est à madame la ministre de la transition écologique Madame Barbara Pompili. Merci monsieur le président, Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Bono, vous l'avez dit le président Poutine a pris une décision grave pour l'Ukraine pour la sécurité du continent européen et la situation à la frontière est très préoccupante, le président de la République mène une action résolue pour faire face à ce danger d'escalade, mais sur la question que vous soulignez, en réponse à vos interrogations, je veux tout d'abord vous dire que même si la Russie devait cesser ses exportations, ce qui n'est pas à l'ordre du jour actuellement nous ne courons pas de risque d'approvisionnement en matière énergétique, qu'il s'agisse des carburants ou du gaz en particulier, nous avons des stocks stratégiques de pétrole important qui couvre près de 90 jours dans près de 3 mois de notre consommation et qui nous permettent de faire face à des perturbations d'approvisionnement et je vais donc être très clair à ce sujet, les Français ne risque pas de manquer de carburant ou de gaz pour se chauffer dans les prochains mois, s'agissant des prix de l'énergie, le gouvernement s'surveille évidemment la situation de très près, nous avons démontré au cours des derniers mois, notre capacité à agir chaque fois qu'il s'est avéré nécessaire pour protéger le pouvoir d'achat des Français, je citerai évidemment l'indemnité inflation exceptionnelle de 100 euros ou encore les bouclier tarifaire en matière de gaz et d'électricité, je me suis entretenu hier soir avec la commissaire européenne à l'Énergie Kadri Simpson et nous avons discuté de tous ces points et de la de la bonne coordination au sein de l'Union européenne sur ces questions, nous avons également des contacts réguliers avec le gouvernement des États-Unis pour envisager des actions coordonnées si la situation le justifiait donc le gouvernement est évidemment pleinement mobilisés protégera comme il a su le faire, ces derniers mois, non seulement notre approvisionnement en énergie, mais aussi le pouvoir d'achat des Français et je rajoute que sur cette question de la fixation des prix, nous avons déjà depuis un certain temps eu des discussions avec la Commission européenne pour revoir le ce qu'on appelle le Market designs et je crois que c'est le bon moment pour avoir ces discussions avec la Commission. Monsieur Oui, madame la ministre, la dépendance de l'Europe au gaz russe a augmenté en 10 ans de 24 à 40 %. Pour passer au gaz naturel liquéfié qui pourrait être une une solution ce sera coûteux et ce sera long. Donc il est urgent. D'avoir une politique énergétique qui diminue notre dépendance au gaz russe. La parole est à notre collègue Fabien Gay pour le groupe communiste, républicain, citoyen. Le juge devait la parole. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Vladimir Poutine a décidé unilatéralement, lundi soir, de reconnaître les républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk cette décision inacceptable et dangereuse intervient après la non application des accords de Minsk l'atteinte portée à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et l'imminence d'un conflit armé constitue un échec collectif qui est celui de toutes les parties en présence, pourtant l'escalade continue, l'Allemagne a annoncé hier après-midi, la suspension de l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2, les États-Unis et l'Union européenne, annonce de nouvelles sanctions économiques alors que celles prises jusqu'ici contre le régime de Poutine ont été contre-productives, le cerveau et renforçant ses élans ultranationalistes plus inquiétant encore, l'OTAN institution bellicistes et obsolète, survivance de la guerre froide s'est réuni hier avec les autorités autorités ukrainiennes alors que plusieurs de ses membres se déclarent prêts à se déployer en Lituanie depuis 2014 les exactions nourrissent les haines et le poison nationaliste notamment Donbass pour l'apaisement dans la région, il faut en finir avec l'esprit de vengeance et de haine, notre responsabilité, celle de la France, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la responsabilité de tous les dirigeants politiques européens et du monde et de se dresser résolument contre la guerre et de n'avoir à l'esprit que les seuls intérêts des peuples ukrainiens, russes et européens ses intérêts sont mutuelle et se résume en un mot : la paix, non pas comme une étape, venant après la guerre, mais bien quand même projet politique qui implique des efforts considérables de part et d'autre pour en créer par l'action politique et diplomatique, les conditions réelles seul ministre nous vous faisons humblement une proposition : celle de l'organisation sous l'égide de l'ONU d'une conférence extraordinaire paneuropéenne de coopération et de sécurité collective incluant la Russie et l'Ukraine, c'est pour nous le moment, je vous remercie. Pour vous, la parole est au secrétaire d'État au sort des Affaires européennes, vous avez la parole monsieur le Ministre. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, nous partageons je pense surtout, c'est bon et c'est la position constante du gouvernement lui prend de la République, les efforts nécessaires doivent être déployés sans relâche encore aujourd'hui pour préserver la paix, je ne partagerai pas, en revanche, votre analyse sur le rôle, en l'occurrence de l'OTAN, organisation bellicistes et vous dit pardon dans la situation dans laquelle nous sommes, il faut être très simple et très claire nos alliances, nous savons où elles sont, c'est l'Union européenne et c'est l'OTAN, ce n'est pas nous, ce n'est pas l'OTAN, ce ne sont pas les États-Unis, Amérique, ce n'est pas l'Europe qui a voulu un conflit et qui a violé gravement le droit international, il faut quand même revenir aux faits. Nous ne pouvons pas nous avons eu ce débat tout à l'heure, reprocher à la France d'avoir ménagé ses efforts pour ouvrir la voie à la diplomatie à une solution politique et à la paix, mais il faut constater, il faut constater ensembles que c'est la Russie et le président Poutine, qui, en début de semaine, a choisi le chemin d'une violation très grave du droit international, cela aboutit à une réaction d'unité et de fermeté européenne et occidentale, nous l'assumons par l'imposition aujourd'hui même de sanctions qui sont coordonnées avec nos principaux partenaires et décidé au niveau européen la solution que vous proposez, dans lequel des Nations-Unies, nous l'avons évoqué le prendre la République l'a dit dès lundi en proposant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour commencer, c'est notre responsabilité de membre permanent, forcé de constater là aussi que la Russie n'a pas accepté de prendre un chemin diplomatique et de paix à l'occasion de cette discussion aux Nations-Unies, donc nous ne sommes pas dans la surenchère, certainement pas, nous ne sommes pas la provocation, certainement pas, nous sommes dans la réponse proportionnée, mais extrêmement ferme à des agressions et des violations territoriales qui ont été choisis à ce stade par le président Poutine et par la Russie, nous devons le constater mais nous efforts diplomatiques soi-disant sur se poursuivront et je salue le fait que vous les souteniez. La parole est au président François Patriat pour le groupe du Rassemblement des démocrates. On Aspire si l'indépendance, vous avez la parole monsieur le président, Monsieur le 1er ministre samedi prochain, le salon de l'agriculture à Paris ouvrira ses portes et vous savez, les centaines de milliers de Français qui s'y rendront le salon de l'agriculture, c'est un hymne au territoire à la ruralité à l'agriculture, c'est un moment d'excellence et du Made in France à un moment de rencontre entre les villes et les campagnes autour de découverte et d'échanges, c'est un rendez-vous d'autant plus attendu que la version 2021 avait été annulé à cause de la pandémie, c'est un lieu où la profession agricole fait découvrir ses réussites mais aussi où elle fait remonter ses inquiétudes, parfois même ses désespoir et parfois même ses colères au cours de ces dernières années, la profession agricole a dû faire face à des crises climatiques, sanitaires financières auxquelles le gouvernement et le Parlement ont apporté des réponses nous tous ensemble d'ailleurs, il est temps Monsieur le 1er ministre de faire un bilan qui réformes accomplies pour lesquels nous avons su allier à la fois une vision claire et ambitieuse, avec une méthode basée sur la concertation, je pense à France relance et au plan protéines pour notre souveraineté alimentaire, je pense aux loi Egalim pour le revenu au doublement de la surface en bio à la protection des sols au développement des circuits courts aux retraites agricoles et plus récemment à l'assurance-récolte et au plan massif lancé par les assises de l'eau, chers collègues, vous avez voté ces lois pour la plupart, nous avons su prendre des initiatives qui répondent à la fois à notre modèle social, économique et à l'urgence climatique en quoi toutes ces réformes qui ont jalonné ces 5 années pour permettre à notre agriculture d'être au rendez-vous de la 3ème révolution agricole fondée sur le numérique, la robotique et la génétique, je vous remercie.

Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le président, François Patriat, merci de me donner l'occasion. C'est parce que c'est la dernière séance, ce que vous êtes déjà dans sa logique. Je reviens à l'objet de la question, Monsieur le Président, qui me donne, disais-je l'occasion avec vous toutes et vous tous de rendre hommage à nos agriculteurs. Effectivement, à quelques jours de l'ouverture d'un moment très important pour eux et pour toute la nation Le Salon de l'agriculture nos agriculteurs, puisque vous avez évoqué, monsieur le président, Patriat. La crise sanitaire qui ont été, je le rappelle au rendez-vous, toujours là, jamais, pas un seul jour la France d'a manqué s'alimenter par cette par ces temps par ces temps difficiles au cours de cette crise nos agriculteurs qui, vous le savez, c'est un élu d'un département très rural, natif d'un département encore plus rurales qui vous parle. Qui sont évidemment absolument indispensables à notre nation qui luttent courageusement contre des transformations considérables que vous vivez, mesdames et messieurs les sénateurs dans vos territoires, vous me permettrez, puisque c'est la dernière président de rendre hommage aussi à mon ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Oui, parce que je vais vous dire là, vous ne pouvez pas je vois que certains applaudissent, mais au fond de vous-même, on Phone vous-même dans vos territoires dans vos départements, vous le voyez agir vous savez les relations et la confiance qu'il a su drainer oui oui oui, vous pouvez dire non, moi je vous dis ce que je pense, je suis là pour répondre, messieurs dames, vous êtes type de pas être d'accord, mais j'affirme qu'il a su drainer la confiance de cette profession dans les graves difficultés qu'elles traversent, oui, oui, bon, et il l'a fait, je vais vous dire pourquoi, bien sûr, parce qu'il est talentueux mais il l'a fait parce que nous déployons une politique agricole extrêmement ambitieuse, nous sommes aux côtés des agriculteurs de France, de la même façon que l'industrialisation ou la réindustrialisation de notre pays figurent parmi nos premières priorités le soutien, c'est la même chose à l'agriculture est indispensable,

qu'est ce que nous cherchons à faire ensemble, je sais que vous partagez tout ça toutes et tous, d'emblée, les faire vivre de leur travail, c'est la première priorité, les faire vivre de leur travail et de celle-ci travaille et Dieu sait s'ils travaillent de réforme, vous les avez voté alors ne criez pas, on a un, à l'initiative que vous les avez voté la loi, et ça c'est monsieur le président, un processus intéressant la loi Egalim la loi Egalim oui mais si vous voulez bien sûr la loi Egalim 1 et 2 c'est intéressant parce que la loi Egalim, hein nous avons reconnu qu'elle n'avait pas atteint son objectif, nous l'avons dit sinon on n'aurait pas proposé un 2ème texte et nous veillons comme le lait sur le feu, je le dis parce que c'est maintenant et que je me sers de votre tribune pour lancer un appel très clair à tous les professionnels, nous veillons très fermement aux négociations commerciales qui sont en cours et qui ne peuvent pas se conclure au détriment de nos agriculteurs, c'est quand même un changement de pied par rapport à certains textes qu'on a connu et dont l'objectif 1er c'était la baisse des prix par la concurrence, vous vous souvenez tous de ça dont Egalim c'est un sujet central, la revalorisation des petites retraites agricoles, là aussi, texte voté à l'unanimité d'abord pour les anciens exploitants puis pour leurs conjointes et conjoints, ça c'est une avancée majeure à mettre au crédit de ce quinquennat mesdames et messieurs les sénateurs, vous le savez, d'autant plus que vous l'avez approuvé et puis je termine là- dessus oui, ben oui, j'aimerais bien que vous êtes tellement que j'aimerais prendre le micro, tout l'après-midi. Et puis non, non, mais attendez, vous le savez bien, vous avez parlé, Monsieur le Président, Patriat qui connaissait si bien à ce sujet. Des catastrophes climatiques, j'ai été chef du gouvernement pendant la plus terrible depuis des décennies, elle a frappé beaucoup de vos départements, c'était au printemps dernier, je crois que vous avez tous reconnu que la réaction a été à la hauteur, mais surtout, au-delà de la conjoncture parce que je ne suis pas le 1er, chef du gouvernement à avoir débloqué des crédits car il y a une crise agricole, on a fait aussi, je le rappelle pour la filière porcine récemment on l'avait fait pour les éleveurs, là, c'est pour une catastrophe climatique, nous vous avons proposé ça s'est terminé par une CMP conclusive un changement complet de l'assurance-récolte ça aussi, depuis quand moi j'en entends parler, mesdames et messieurs les sénateurs, depuis des années et des années, nous l'avons fait merci beaucoup. Monsieur Patriat vous renoncez. La parole est à notre collègue Jean-Yves Leconte pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Monsieur le président, Monsieur le 1er ministre ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, la situation en Ukraine est en cet instant, au coeur de nos inquiétudes. Les récentes décisions de Vladimir Poutine, sont une menace pour l'Europe, mais aussi pour le monde un peu plus qu'il y a qui il y a 8 ans s'est levé pour arracher son droit à une perspective européenne est aujourd'hui menacée, il est menacé par ce qu'il a revendiqué cette liberté et cette indépendance qui aujourd'hui nous à lui nos destins sont aujourd'hui liés, la France a appelé ses ressortissants à quitter l'Ukraine partir pour protéger sa famille pour se protéger, rester pour accomplir sa mission marquer sa solidarité avec ses proches, c'est un choix qui appartient à chacun, en conscience, et qui peut évoluer, mais la France lance un appel pour inciter à quitter l'Ukraine, la question de monsieur le ministre est donc la suivante : comment faire si les avions se font rares et chers, comment faire si c'est si personne ne vous attend en France beaucoup disposent de solutions, mais que faire pour les autres, pour les accueillir, quelles dispositions sont prises par le Centre de crise et de soutien, l'anxiété monte en Ukraine, plus de 200000 personnes vivent sur la ligne de contact et sont directement menacés, les morts et les blessés augmente chaque jour un important exode est à craindre, nombreux sont ceux qui se mobilisent pour faire face à une telle situation, en espérant qu'elle n'arrivera pas tout à fait, les besoins sont immenses médicaments équipements en traumatologie, soutien psychologique, accueil des réfugiés, quel sera l'apport de la France, quel sera l'apport de l'Union européenne face à ses besoins et à ces menaces que prépare-nous dans ce cadre. Pour vous et pour la parole. Le secrétaire d'État en charge des affaires européennes, c'est le ministre. Merci beaucoup monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, le compte, vous avez rappelé la gravité de la situation que plusieurs sénateurs ont déjà évoqué, vous soulignez une dimension humanitaire humanitaire et humaine de cette crise, notamment la situation de nos ressortissants qui étaient évidemment notre priorité, nous avons, c'est la responsabilité du Quai d'Orsay adapter nos recommandations pour les voyageurs comme pour nos ressortissants sur place, à 3 reprises au cours du mois de janvier, et nous l'avons fait face à la dégradation de la situation sur place encore ce week-end avec un message d'évidence, nous demandons à tous les voyageurs d'éviter de se rendre en Ukraine, bien entendu, et nous avons indiqué à nos ressortissants que sauf motif impérieux, il était nécessaire et plus prudent de quitter l'Ukraine, vous ne connaissez la communauté française en Ukraine, au début de la crise étaient environ, évalué à 1000 personnes près d'un millier principalement des binationaux, c'est pour cela que bien sûr il faut évaluer la situation au cas par cas, certains pour des raisons nécessaire certains par engagement et solidarité peuvent faire le choix de rester d'accompagner ceux qui sont proches, et nous analysons les choses au cas par cas, c'est aussi la raison pour laquelle nous avons mobilisé notre ambassade qui restent ouvertes, dans un format toujours opérationnel évidemment resserré, compte tenu de la situation, vous le comprendrez mais pour accompagner nos ressortissants pour traiter chaque situation nécessaires et c'est aussi l'instruction qui a été donné par Jean-Yves Le Drian au Centre de crise qui avec notre poste consulaire analyse chacune des situations et chacun des cas particuliers, vous évoquez aussi le cas humanitaires au-delà de nos propres ressortissants et de la Communauté française ou franco-ukrainienne, la France est au rendez-vous depuis le début de la semaine, les autorités ukrainiennes ont fait appel à ce qu'on appelle le mécanisme de protection civile de l'Union européenne qui apporte de manière préventive en l'espèce un certain nombre d'équipements de santé le protection des tentes, des kits et la France a fait partie des 5 premiers pays européens dès lundi, qui a répondu présent et qui achemine qui a déjà acheminé, d'ailleurs, depuis mardi, un certain nombre de matériel au cas où et pour protéger non seulement la communauté française, mais aussi l'Ukraine avec lequel la solidarité est absolue et continuera à s'amplifier. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour ces réponses, mais n'oublions personne il y a des gens qui ont besoin effectivement d'être accueillis. De pouvoir avoir les moyens de voyager s'il décide de rentrer, cela doit être absolument dit et répété et pouvoir être fait et préparée face à l'importance de la menace des dispositifs à la hauteur des risques pour l'ensemble des Ukrainiens en matière humanitaire c'est essentiel. Si la parole est à notre collègue et rigole pour le gros du rassemblement. Démocratique et social européen de la parole. Merci monsieur le président, ma question s'adresse à Madame la Ministre de la transformation et de la fonction publique. Cela fera bientôt un an que le Sénat a adopté la proposition de loi du groupe RDSE relative à la lutte contre l'électronicien, le constat est clair et partagé par tous les bancs de cet hémicycle, dans une société de plus en plus numérique près de 14 millions de Français en sont exclus, par manque d'équipement par manque de réseau et surtout par manque de compétences. Des difficultés qui touchent d'abord les plus fragiles, les personnes en situation de précarité sociale, en situation de handicap, les personnes âgées et les étrangers, plus grave, c'est dans l'accès aux services publics que les difficultés sont les plus importantes, puisque 40 % de la population ne se sont pas à l'aise avec les démarches en ligne. Cette situation entraîne un recul de l'accès au droit, particulièrement inquiétant. Malgré les efforts déployés, je pense notamment aux Maisons France service une partie de la population demeure exclu ou en difficulté face aux démarches qui permettent d'accéder aux droits légitimes. C'est le constat fait une nouvelle fois par la défenseure des droits dans ce rapport publié la semaine dernière, plus de 80 % des réclamations qui lui sont adressées concernent les services publics, avec quasiment toujours un problème via les dématérialisation ou à l'impossibilité pour l'usager d'échanger avec l'agent s'occupant du dossier. 3 ans après son précédent rapport sur lequel je vous avez déjà interrogé la situation, a peu évolué, c'est désormais à l'usager de s'adapter aux service public souligne la défenseur des droits, et c'est heureux renversement de la responsabilité dans l'accès aux droits qui repose désormais sur l'usager plutôt que sur l'administration. Madame la ministre nous entrons aujourd'hui dans un la phase de déploiement de l'espace numérique de santé qui va entraîner une dématérialisation accélérée dans un domaine hautement sensible aussi, pouvez-vous nous préciser comment, dans ce domaine comme dans l'ensemble des services publics, l'accès au droit de nos concitoyens peut être garanti, je vous remercie. Bon vous réponde, la parole est à la ministre de la transformation de la fonction publique, madame de Montchalin, vous avez la parole. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur, d'abord vous dire que nous partageons pleinement et totalement vos alertes, la politique du gouvernement depuis 2017, elle tient en quelques mots, et elle est essentiel, c'est d'avoir un service public qui soit efficace qui soit plus proche des Français et qu'il soit humain et notre ambition très concret, je vais le détailler a été précisément que ce soit au service public de s'adapter et pas aux Français et que les Français et le choix faisait le choix d'avoir un service de proximité nouveau avec ces nouveaux guichets de proximité que sont les espaces France service 25 dans votre département qu'aient le choix d'avoir un contact téléphonique qu'ils aient le choix d'avoir également du numérique quand il souhaite faire sa démarche par le numérique, nous avons donc choisi de ne pas choisir entre des moyens différents, parce que les Français doivent avoir un service public qui leur correspondent, vous avez parlé de l'espace numérique en santé, nous avons pris l'engagement que pour toutes les démarches dématérialisées numérisé, il y a toujours désormais un accompagnement physique pour l'espace numérique de santé, ça peut être un pharmacien un professionnel de santé pour tous les aux démarches cessera dont les francs service un engagement que nous avons pris avec Jacqueline Gourault et nous prenons très au sérieux ces alertes de la défenseure des droits parce qu'elle est une vigie essentiel et nous avons ainsi résolument engagé un travail avec les associations d'aide aux plus fragiles, aux plus vulnérables, j'étais la semaine dernière en Eure et Loir dans une France, service d'abord qui est trop peu connu des Français, puis avec le préfet avec toutes ces associations qui accompagnent les plus fragiles, les familles rurales, les retraités et nous avons demandé avec Jacqueline Gourault que dans chaque département, dans le mois qui viennent, dans un espace France service ces acteurs qui suivent les Français parfois déconnectées parce qu'ils n'ont pas été formés parfois qui ne veulent pas avoir accès au numérique ou qui ne connaissent pas assez franc service qu'il puisse être accompagnés notre enjeu, ce sera jusqu'à la dernière minute et jusqu'à la dernière de ce gouvernement le considérer qu'il n'y a pas de fatalité à la fermeture, que nous devons accompagner chacun que de l'humain doit être mis sur le terrain et nous n'avons pas, contrairement au précédent quinquennat considéré qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de laisser passer un mouvement certes inexorable, mais sur lequel nous avons beaucoup à faire pour accompagner chacun dans ses services publics qui doivent rester accessible proche et humain.

Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la culture. Elle porte sur l'épisode judiciaire qui traverse une nouvelle fois le quotidien La Provence, qui au fil des années devient hélas la figure éponyme des turbulences que traverse la presse française à l'heure où une commission d'enquête mène en nos murs, un travail de fond sur la concentration dans l'immédiat les conditions qui préside la procédure de cession, visant le rachat de 89 % des parts de la Provence revêt une acuité particulière et nous interroge à plus d'un titre, elle nous interroge en 1er lieu sur les procédures de rachat d'organismes de presse verrouiller en amont par le biais d'une clause d'agrément, la procédure de cession d'actifs à dévoyer le droit applicable, censé garantir le pluralisme de la presse et cela pour flécher le rachat de la société dans les mains d'un seul homme, comment ne pas s'indigner dans le quand le 4ème pouvoir garant de la formation des citoyens et de la vitalité démocratique et menacé de prédation par l'oligarchie économique, comment ne pas réagir alors que nous connaissons, que vous connaissez l'importance de ce groupe de presse pour Marseille et la région sud et pour la Corse, garant de la diffusion de la pluralité de l'information et des opinions, comment, alors que l'État pourtant créancier principal dans cette procédure peut-il rester silencieux et accepté la cession d'un journal, responsable d'une émission citoyenne dont le prix de rachat reste le seul élément déterminant sans qu'aucun impératif sur le volet social sur l'indépendance des rédactions ne soit formulée, comment pouvez-vous sans réagir, laisser cette procédure, être le triste reflet de l'effondrement démocratique en France, comment, enfant de Madame la Ministre, laissez l'avenir de 850 emplois en Provence et en Corse, de 6 entreprises, outre celui de 2 titres de presse régionale encourir telle risque alors même que le président de la République ne cesse de communiquer sur l'importance de la réindustrialisation du pays et l'sa préservation de l'emploi dans quelles mesures comptez-vous agir pour répondre à ces enjeux politiques, économiques et sociaux. On vous réponde, la parole est à madame la ministre de la Culture Madame Roselyne Bachelot. Il avait la parole, Madame la Ministre. Monsieur le sénateur, Paris je vous appelez mon attention sur les turbulences que traverse le titre La Provence La Provence, vous l'avez rappelé c'est un quotidien régional extrêmement important, 75000 exemplaires il tient particulièrement au coeur des Marseillais, mais également puisque le groupe détient le titre Corse-Matin, le seul quotidien insulaire, il tient aussi particulièrement au coeur des Corses alors vous l'avez signalé également cette procédure de rachat, c'est la procédure de rachat de 89 % des parts qui était détenu par Monsieur Bernard Tapie il ne revient pas à l'État d'intervenir dans la procédure de rachat, c'est le tribunal de commerce qui va juger bien entendu du meilleur repreneur de ses parts à la fois sur le plan financier, sur le plan social et bien sûr sur le plan des des investissements nécessaires, car les investissements qui vont être utiles pour que ce quotidien fait quotidien marche ces investissements sont extrêmement importants, nous suivons cette procédure avec une grande attention comme nous suivons toutes ces procédures, je veux rappeler, Monsieur le Sénateur, que dans le cadre du plan de relance, nous avons soutenu à hauteur de 480 millions d'euros, la presse quotidienne pour lui permettent d'exister, de traverser ces turbulences et que bien entendu autant que nécessaire, le Fonds stratégique pour le développement de la presse pourra être convoqué devant toi le demander, demander une subvention dans ce cas, en tout cas, nous suivrons avec une particulière attention le sort de 850 salariés, c'est certes une procédure privée mais ce n'est pas pour cela que l'État est absent, je vous en donne ma garantie merci monsieur le sénateur. Merci de me donner la parole maintenant. Au président François-Noël Buffet pour le groupe Les Républicains. Merci, merci. Merci monsieur le président, ma question s'adresse à Madame la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Dans quelques minutes, cette séance sera suspendue, c'est la dernière de notre quinquennat puisque le parlement suspendra ses travaux à la fin de la semaine pour cause d'élection présidentielle, il se trouve que c'est donc un peu l'heure des bilans. Et au bilan de la sécurité, nous avons un certain nombre de questions, en tous les cas une en particulier à vous poser. Nous n'avons eu de cesse de constater ces dernières années une augmentation forte du niveau des agressions à l'égard des personnes physiques. Les chiffres que nous connaissons et qui ont été portés à notre connaissance, par vos propres services indique que depuis 2017 le nombre de coups et blessures volontaires a augmenté de 18 % que depuis 2017 les risques ont augmenté de 60 % que les agressions sexuelles de 38 % et les menaces contre les élus ont été multipliés par 3, c'est donc un point particulier qui intéresse évidemment spécifiquement les Français, qui est de constater que, malgré les efforts que vous nous avez annoncé voire même nous avons accompagné dans ses efforts, à l'occasion d'avis budgétaires ou de vote dans cet hémicycle les effets ne sont pas là et moi j'ai une question très simple : depuis 2017, cette augmentation n'aimait pas une stabilisation, c'est une véritable augmentation que s'est-il passé et quelle explication pouvez-vous nous donner. Pour vous répondent : la parole est à la ministre déléguée. Charge de la citoyenneté Madame Schiappa vous avez la parole. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le président de la commission des lois, j'avais d'abord prévu comme c'est notre dernière séance de questions au gouvernement au Sénat de saluer le travail que vous avez mené comme président de la commission des lois, ainsi que tous les membres de votre commission et votre prédécesseur, monsieur le sénateur Philippe Bas parce que nous avons eu des lois difficile à voter ensemble avec des désaccords parfois profonds, mais toujours dans le respect, je crois, dans le sens de l'intérêt général et je voudrais vous remercier pour cela pourrait vont donc maintenant à votre question, je voudrais vous dire qu'effectivement les choses que vous avez cités sont extrêmement importants et préoccupant sur la question de la violence à l'égard des élus, notamment il y a ce climat de violence qui nous préoccupe, et vous savez à quel point nous sommes mobilisés, les circulaires ont été prises par le garde des Sceaux, par le ministre de l'Intérieur, des dispositions de formation des maires également des intervention du GIGN pour mieux protéger les les élus, donc de nombreux dispositifs sont déployés et sont mises en oeuvre à cet égard, en ce qui concerne les violences faites aux personnes, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons déployé un certain nombre de dispositifs pour inciter notamment les femmes et les victimes de violences intrafamiliales a davantage porter plainte et davantage s'adresser aux forces de l'ordre, ce qui fait que nous avons, c'est vrai, une explosion des dépôts de plainte ce qu'on appelle un contentieux de masse parce que nous avons, y compris des faits antérieurs qui aujourd'hui sont dénoncés ou des faits qui auparavant étaient considérés comme des banalités des drames conjugaux, des faits divers des crimes passionnels qui sont désormais dénoncer auprès des forces de l'ordre et auxquels la police et la gendarmerie apporte ses réponses en cumulé, vous l'avez rappelé il y a plus 10 milliards d'euros d'augmentation budgétaire sur le sur le quinquennat 10000 policiers et gendarmes supplémentaires, c'était un engagement du président de la République en 2017, cet engagement est bien tenu, le ministre de l'Intérieur a donné des impulsions fortes, notamment avec le bobo de la sécurité est ce qu'il faut faire encore plus, la réponse est oui, et c'est d'ailleurs pour cela que le président de la République à Nice, invité par monsieur le maire, Christian Estrosi a souhaité présenter à la la prochaine grande loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, présenté par le ministre de l'Intérieur et qui nous permettra d'encore mieux protéger les Français dans la droite ligne de ce que nous avons fait depuis 2017, je vous remercie. Madame la ministre, d'abord je vous remercie de vos remerciements, je pourrais vous les renvoyez mais je voudrais simplement vous dire que je peux comprendre une partie de l'argumentation sur les violences faites aux femmes, effectivement, il y a un effort réel dans la capacité de libérer la parole en revanche sur les risques, c'est plus de 60 % d'augmentation, la violence sur les élus et et croissante, encore la semaine dernière un maire du Rhône, ce qui m'inquiète, c'est le rapport de la Cour des comptes, en réalité, qui dit très clairement que, malgré l'augmentation budgétaire qui vous a été accordé, malgré le fait qu'il y a eu plus de policiers recrutés, il n'y a pas eu d'effet par rapport à la lutte contre les violences et cela, je n'arrive pas à me l'expliquer, ce sera, je le crois un de vos échecs ou une de vos erreurs, en tous les cas. Merci, la parole est à notre collègue Jean-Claude Tissot pour le groupe socialiste, écologiste d'homme d'État. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre de l'Agriculture, mes chers collègues en matière agricole, le programme d'Emmanuel Macron, en 2017 mettant en avant, de grandes priorités le rééquilibrage de la valeur au sein des filières et les pesticides au début du quinquennat le discours de Rungis et les états généraux de l'alimentation, on peut faire croire à une réelle volonté de changer la donne, le président de la République, on mettait ainsi une loi, je cite : permettre aux agriculteurs de vivre du juste prix payé la loi il y anime très modestement corrigés par la loi Egalim 2, vous l'avez dit monsieur le 1er ministre a rapidement montré toutes les limites de la théorie du ruissellement appliquée à l'agroalimentaire, avec une baisse du prix d'achat aux producteurs en 2019 le bilan d'un constat d'échec unanimement partagée, sauf, bien sûr, au sein de la grande distribution, le candidat Emmanuel Macron avait également promis, je cite, un calendrier prévoyant l'élimination progressive des pesticides et le développement d'alternatives, d'alternatives, 5 ans plus tard, toujours pas de calendrier et presque toujours autant pesticides on constante en nous, on constate en outre un manque de transparence de l'ONU, puisque le nom du indicateur de référence du plan Ecophyto n'a toujours pas été publiés pour 2020 alors qu'il aurait dû l'être, en décembre 2021, pouvez-vous nous donner Monsieur le ministre, ce bilan quant aux alternatives, une première brèche a été ouverte avec la réautorisation des néonicotinoïde pour la filière betterave finalement, à quoi bon rechercher des alternatives si le gouvernement accepte de détricoter la loi à la demande, le bilan, un échec de l'aveu même du président de la République sur le glyphosate, qui devait être interdit, sous 3 ans et dont les ventes ont à peine baissé de 2 % la déclinaison que vous allez faire, ne pas qu'avec le PSN, Monsieur le Ministre, confirme encore le choix d'une orientation qui se traduit par la chute du nombre d'exploitations et d'emplois, l'insuffisance des revenus des agriculteurs et une dépendance à des substances nocives pour la santé et l'environnement ainsi l'augmentation du seuil d'accès à l'ICHN va encore entraîner la disparition de petites fermes dans mon département de la Loire, cela concerne 69 exploitations au final vous avez tourné le dos à vos objectifs initiaux pour conforter un modèle agro- industriel qui se noie dans ses propres dérives monsieur le Ministre, ne pensez-vous pas qu'il est temps de changer de direction. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de l'alimentation. Si on Monsieur Julien Denormandie. Merci beaucoup monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Tissot je crois que fondamentalement nous ne partageons pas forcément la même vision, vous me direz. C'est beau, en démocratie, que d'avoir des visions différentes, mais je voudrais vous. Vous répondre d'abord sur une vision, une méthode et les résultats, la vision, c'est la souveraineté agroalimentaires de notre pays, la vision, c'est de pouvoir avoir notre indépendance alimentaire la vision, et d'ailleurs vous ne l'avez jamais dit dans vos 2 minutes de questions, c'est d'abord la mission nourricière de notre agriculture, ne l'oublions jamais : c'est trop facile, que de l'oublier ensuite la méthode, la méthode, c'est de remettre la science et la raison, au centre de tout remettre la science et la raison, au centre de tout, c'est souvent plus courageux que d'être dans le sens du vent au gré de prises de position d'injonction et du yakafokon et je crois que remettent la science et la raison, surtout pour quelqu'un qui connaît si bien l'agriculture que vous messieurs Tissot, c'est quelque chose de fondamental et vous savez à quel point je me suis engagé dans ce combat pour plus de sciences et plus de raison dans nos politiques agricoles enfin sur les résultats, monsieur Tissot depuis 2017, vous parlez des produits phytosanitaires, depuis 2017 les substances les plus préoccupantes : moins 93 mère, de moins 40 % le bio, vous en parlez souvent, on a doublé depuis 2017 la surfaces agricoles en bio dans notre pays, nous sommes aujourd'hui le le pays d'Europe avec la plus grande surfaces en bio, quand vous prenez la question de la rémunération, la loi Egalim 2, elle vient d'être votée, vous en connaissez beaucoup de mandature qui remet l'ouvrage sur le métier, quand il considère par eux-mêmes que la loi Egalim a n'a pas été assez loin, c'est pas forcément ce que font généralement les politiques, nous l'avons fait et nous nous battons, comme l'a dit le 1er ministre et puis je voudrais simplement terminer puisque c'est ma dernière de cette session, pour remercier l'ensemble du Parlement, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous tous, on a souvent eu des désaccords, mais on a toujours trouvé en Intelligence accords je voudrais saluer la présidente Prima, le rapporteur Laurent Duplomb et vous dire et vous dire mesdames et messieurs les sénateurs, que dans le monde agricole, la politique du dépassement, ça marche et je suis sûr que ça peut marcher dans d'autres secteurs et donc fait le choix de cette politique du dépassement. La parole est à Madame Dominique Estrosi. Sonne pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président, ma question s'adresse à monsieur le 1er ministre et je vous propose d'y répondre, il y a 5 ans, le candidat Emmanuel Macron promettait un choc de l'offre afin de faire baisser les prix de l'immobilier, il promettait la construction de 60000 logements étudiants et de répondre aux besoins des ménages aux revenus les plus modestes, force est de constater, 5 ans après le nombre de permis de construire et de mises en chantier est passé sous la barre symbolique des 400000 cette crise du logement, peut-être l'une des plus graves pour notre pays depuis l'hiver 54 ans, qui a conduit à l'appel de l'abbé Pierre est le fruit de décisions qui ont pénalisé l'ensemble du secteur baisse des APL de 5 euros réduction du loyer de solidarité supporté par les bailleurs sociaux, augmentation du taux de TVA à 10 % pour le logement social, fin de l'aide aux maires bâtisseurs zigzag avec le PTZ, fin de l'APL accession attaque de la maison individuelle, la politique du logement d'Emmanuel Macron n'aura été que des coups de rabot successifs des louvoiements des dérobades faisant payer aux Français le prix fort de cet immobilisme, alors Monsieur le 1er ministre quelle était votre réponse face à ce décalage décalage si gros entre les promesses du président de la République et la réalité de son échec en matière de logement.

Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Dominique Estrosi Sassone d'abord je voudrais vous remercier pour votre engagement sur ce sujet, du logement et je voudrais associer Valérie Létard Viviane Artigalas et Marie-Noëlle Lienemann, qui travaille depuis de nombreuses années sur ce sujet et avec vous, nous avons avancé, nous avons avancé dans la loi 3DS puisque nous avons eu une CMP conclusive sur le sujet du logement social et sur la loi climat et résilience et donc je voudrais saluer le travail que nous avons fait au Sénat sur cette question du logement, les permis de construire, mais vous le savez, madame la sénatrice sont à 470000 sur les 12 derniers mois et nous avons plus de permis de construire dans ce quinquennat que dans le quinquennat précédent 2 1000000 270000 dans le quinquennat actuel 100000 de plus que dans le quinquennat précédent les mises en chantier sont également supérieurs dans ce quinquennat que dans le quinquennat précédent, donc nous avons redressé la construction en France, la construction neuve a repris et c'est important, nous avons aussi investi comme jamais dans la rénovation énergétique des logements avec une vraie révolution avec ma prime rénovent nous y mettons maintenant 2 milliards et demi plus autant de certificats d'économie d'énergie, un 1000000 de Français ont déposé un dossier dans cette période où les prix de l'énergie sont chères dans cette période où la rénovation énergétique est à la fois bonne pour le pouvoir d'achat est bonne pour la planète est bonne pour nos artisans, nous sommes au rendez-vous et nous n'avons pas laisser sur le côté, les plus fragiles : puisque nous avons ouvert 200000 places 200000 places d'hébergement d'urgence et nous avons aussi permis à 330000 personnes d'avoir accès au logement, à partir de la rue ou de l'hébergement, même sur le logement étudiant finalement 57000 logements étudiants ont été livrés et 16000 logements pour les jeunes nous avons encore des besoins, bien sûr, mais nous les soutenons, l'une des jolies réussite de ce quinquennat c'est également la multiplication par 10 de la garantie Visale 660000 contrats ont été signés pour des personnes qui n'ont pas de garant qui n'ont pas de possibilités de cautionnement dont vous voyez, nous avons été au rendez-vous pendant ce quinquennat sur le logement.

le président de la République a une nouvelle fois montré sa déconnexion avec les aspirations des Français, une autre politique du logement était possible et elle est toujours, il est urgent, demain, d'entreprendre de véritables réformes pour répondre à ce besoin essentiel : permettre à chaque Français d'offrir un toit à sa famille. La parole est à notre collègue Amalia Caire pour le groupe de l'Union centriste, ma chère collègue prenait la parole. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les Ministres, chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre chargé des comptes publics, dans son rapport public annuel, la Cour des comptes, alerte sur la situation des finances publiques, il indique que le redressement imposera de réaliser 9 milliards d'économies supplémentaires par an jusqu'en 2027, monsieur le Ministre, les élus locaux sont très inquiets de cette situation, car ils craignent ce que l'on pourrait appeler l'effet Hollande entre 2013 et 2018 la DGF est passé de 41 à 27 milliards d'euros sous le quinquennat de François Hollande et le début de celui d'Emmanuel Macron, les dotations aux collectivités ont donc servi de variable d'ajustement pour redresser les comptes publics, il serait catastrophique pour les collectivités, que cela se reproduise et ce pour 3 raisons : premièrement les finances locales ont été plombés par la crise sanitaire et les charges qui en ont découlé n'ont jamais été intégralement compensée, encore hier, ma collègue sénatrice Jocelyne Guidez évoquer la compensation financière insuffisante pour la mise en place du service minimum d'accueil pour les enfants des écoles, l'autonomie fiscale locale a été substantiellement réduite par la suppression de la taxe d'habitation et enfin les collectivités sont mises à contribution pour des chantiers colossaux qu'il s'agisse de la transition énergétique ou du logement, la préoccupation des élus locaux et d'autant plus grande qu'en 2021, les recettes fiscales locales ont été plus dynamique que prévu, ce qui pourrait être utilisée comme prétexte pour encore amputer les dotations alors Monsieur le ministre ma question est simple, est la suivante : pouvez-vous nous garantir qu'une fois de plus, la DGF ne sera pas la variable d'ajustement, la : l'instrument pardon du redressement des comptes publics, je vous remercie. On vous réponde : la parole au ministre délégué en charge des comptes publics du. Merci monsieur le président, madame la sénatrice, vous m'interrogez sur à la fois la situation des finances locales et sur les perspectives en matière de notation votre question tombe à pic, si vous me le permettez, j'ai présenté ce matin aux associations d'élus et hauts responsables des délégations aux collectivités territoriales du Parlement les l'exécutions comptables des collectivités pour l'année 2021 cette année 2021 qu'une année de reprise, c'est une bonne nouvelle, les recettes fiscales sont dynamiques, les compensations pendant la période de crise ont joué le rôle que nous attendions qu'elles jouons et nous avons à la fois une reprise très forte de l'épargne brute comme de l'épargne nette des collectivités, une capacité à faire face aux engagements et une dynamique pour 2022 qui s'annonce particulièrement bonne puisque, à titre d'exemple, les fraction de TVA affectée aux collectivités régionales, départementales ou intercommunal va augmenter de 6 % cela représente une augmentation de 2 milliards d'euros, et par ailleurs, vous le savez, la révision des valeurs locatives va permettre une augmentation de 3,4 % de celle-ci et en conséquence une augmentation des recettes de la taxe foncière de 1 milliard 600 la situation est donc bonne, et en 2021, à la fin de l'exercice, lorsqu'on le regarde, le niveau d'épargne brute, le niveau de trésorerie, la situation des collectivités, globalement, je sais qu'il y a toujours des individualités meilleur qu'au début du quinquennat pourquoi est-ce que c'est possible, c'est possible parce que nous avons maintenu la DGF à 27 milliards d'euros dans son enveloppe globale, c'est possible parce que nous avons maintenu les dotations d'investissement à leur niveau, et c'est possible parce qu'à l'occasion de la crise, nous avons mobilisé 9 milliards 300 millions d'euros pour aider les collectivités sur 2 ans 9 milliards 3 qui ont permis de compenser les pertes de recettes fiscales et domanial avec le filet de sécurité, d'accompagner les régies de mobiliser 2 milliards et demi d'aide exceptionnel à l'investissement des collectivités et d'accompagner les autorités organisatrices de mobilité ce gouvernement madame la sénatrice a tenu un engagement majeur du président, qui est la stabilité des dotations et la visibilité ainsi que la compensation intégrale des recettes fiscales que nous avons supprimé à l'occasion de telle ou telle réforme comme la taxe d'habitation, si monsieur le président me le permet à un trait de malice, vous me demandez de prendre un engagement, je vous réponds que c'est ce que nous avons fait depuis 5 ans, vous convient plus que ce qui avait été fait précédemment, et c'est ce qui vous inquiète le plus, c'est l'avenir plutôt que ce que nous faisons, gardez-nous. La parole est à Madame Christine L'avare pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président, il nous faudra aussi engager des réformes structurelles et réduire les dépenses publiques, ne laissons pas croire aux Français que l'on pourra réduire la dette uniquement par la croissance, monsieur le 1er ministre ces paroles ne sont pas celles d'un représentant d'une de vos oppositions non ce sont des propos tenus par un de vos ministres devant la commission des finances du Sénat et des mots à la réalité des faits il y a un grand pas, déjà en 2017, le candidat Macron appelé, je le cite, au sérieux et à la responsabilité en matière de finances publiques car, et cela est écrit dans son document de campagne : l'État est lourdement endetté, son premier engagement : réduire les déficits en faisant 60 milliards d'économies, 5 ans plus tard, que constatons nous le répète, le rapporteur général le dit assez souvent la dépense courante a augmenté de 60 milliards 2ème engagement, faire des choix et ciblé un nombre de dépenses prioritaires, 5 ans plus tard, après le quoi qu'il en coûte sanitaire depuis quelques mois, nous vivons le quoi qu'il en coûte électoral, pas moins de 25 milliards de dépenses supplémentaires ont été annoncées de points depuis le mois de juillet dernier, hors plan de relance, hors plan France 2030, le dernier rapport de pays du FMI publié en janvier dernier, préconise à la France de revenir à un déficit de 3 % dès 2025 et de procéder à un ajustement budgétaire important à partir de 2023, vous avez décidé de reporter après les échéances électorales, la publication du programme de stabilité et du programme national de réforme pour autant, la représentation nationale et les Français sont en droit de connaître les réformes structurelles que vous allez mettre en oeuvre, ma réponse est simple ou quelles sont-elles. On vous réponde, la parole est à monsieur le 1er ministre. Je vous l'ai dit j'ai j'ai déjà la nostalgie, monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, non mais sujet évidemment éminemment important, très grave, très structurelles auxquelles, croyez-le bien, j'attache une importance très particulière et la réponse évidemment pourrait là aussi que a longtemps mais je veux vous dire et avec vous, à travers vous à tous mes concitoyens et mes concitoyens que comme vous j'attache beaucoup de respect et d'importance à l'équilibre des finances publiques et à la restauration parce que c'est une question de souveraineté à la restauration des comptes publics Première éléments soyons très factuel, si vous le voulez bien, on peut faire tous les commentaires qu'on veut d'abord. Jusqu'à un tout petit événement qui est venu frapper le pays au début de 2020. Les finances publiques de la France était en voie de redressement.

il y a une commission européenne, dois-je rappeler qu'au début du quinquennat puisque vous y avez fait allusion, nous étions dans une procédure engagée par la Commission européenne au titre du déficit excessif, que je sache, elle avait été levé avant 2020, c'est ça c'est des faits, alors on peut dire que c'est pas assez, ça ne va pas assez vite, très bien, on pourrait aussi faire un peu d'historique sur finances publiques si vous voulez, j'y suis prêt puis est arrivée la crise considérable et brutale, profonde. Juste un mot : non, non, elle a pas bon dos, la crise alors pas bon dos monsieur a sa vérité et on devrait être fier de ce qu'on a fait, écoutez-moi la crise sanitaire, nous en avons beaucoup parlé ici a eu des conséquences économiques considérables, je vous le rappelle. En 2020, le PIB a chuté de moins 9 %. Je fais partie de ceux ici quand bien connu, la précédente grave crise que la France a traversé subprimes 2008 2009, je vous rappelle, moins 3 % 3 fois moins ce genre beaucoup perd 3 % du PIB moins 9 %. avons, nous avons décidé le président de la République a décidé un du quoi qu'il en coûte, ça, ça veut dire éviter que notre économie que les entreprises que des salariés s'effondre et immédiatement après le plan de relance 100 milliards d'euros, vous y avez fait allusion. Je vais vous dire mesdames et messieurs, c'était absolument indispensable dès lors que ces dispositions et c'est ce qui fait la différence, la France le voulait, en 2009 2010 avec la crise présente ses mesures marche et en marché était indispensable parce qu'elles ont été décidées dans un cadre européen coordonné, vous savez, toutes et tous ici que 40 % du plan de relance française sera remboursé par l'Union européenne et vous savez toutes et tous ici, que ça ne peut marcher puisque nous parlons de politique budgétaire que si il y a une politique monétaire qui l'accompagne, et c'est ce qu'a fait et que continue de faire la Banque centrale européenne, vous savez tout ça parfaitement et cet homme plein de relâche, pardonnez-moi, qui marche. Oui 7 % de croissance en 2021 nous avons puisque vous parliez du FMI, moi je lis tous les articles du FMI, le dernier rapport de la Cour des comptes, je connais bien cette noble institution, rassurez-vous, et je sais comme un travail. Bon rapport du FMI, il disait à la France retrouvera la la croissance qu'elle avait avant la crise, c'est-à-dire en 2019 début 2022, on l'a fait à l'été, or les Françaises et les Français l'ont fait à l'été 2021 à partir de là, oui, je suis tout à fait clair avec vous, bien sûr, ça a accru notre déficit budgétaire et notre dette évidemment Et nous avons une stratégie de redressement mais là aussi on a une stratégie non non mais attendez, il faut le dire aux Françaises et aux Français, s'entend bien, ça ne sera pas la purge qui a été fait et tous les experts sont unanimes là-dessus, on la paie encore entre 2011, 2000 12000 imposé pour beaucoup par l'Union européenne, ça n'a pas marché ça a relancé le chômage alors que là, vous le voyez, il est au plus bas depuis des années et des années, mais oui mais oui mais oui les tuer, madame, vous, vous vous dites ça, mais pensez aux jeunes la précédente crise, plus 31 % d'explosion du chômage des jeunes, celle-ci en étant moins 10 grâce à l'apprentissage, vous m'avez toujours dit, j'ai toujours entendu dire : on est très pour l'apprentissage, on en a fait 725000 l'année dernière, on n'avait jamais vu ça, c'est au bénéfice de nos concitoyens, donc oui madame, hein, il faut redresser la croissance pour diminuer. L'autre déficit budgétaire et puis il faut avoir une trajectoire, je l'ai dit 5 % cette année, cap sur 3 % en 2027 faits jugés raisonnables par les organismes, il faut qu'avec des réformes structurelles, en particulier celle des retraites qui doit venir au bon moment au bon moment parce que la, l'art de la réforme, c'est de choisir le bon moment. La France, par son travail remboursera ses dettes et se félicitera des choix économiques qui ont été faits pendant la gestion de cette crise. Merci monsieur le 1er ministre d'avoir pris le temps de me répondent : vous m'avez parlé d'une stratégie, je l'attends parce que je ne l'ai pas réussi à la déceler dans votre réponse, vous m'avez parlé du redressement des finances publiques entre 2017 et 2019, je voudrais juste vous dire que si on rapporte la on met en basse en 2017, la dette des pays de l'Union européenne, pendant que la dette française n'évoluaient pas la dette de l'Irlande et du Pays-Bas par exemple, diminué de 15,7 en fait donc c'est bien de se réjouir de sa stabilité, Kant, les autres ont progressé sur la même période, vous m'avez parlé de souveraineté nos dépenses publiques, c'est très vrai, tellement vrai que le ministre de l'économie à Dieu dans sa réponse à la Cour des comptes précisé que la question de la qualité de la dette française n'était pas en cause, au regard de notre situation actuelle, je voudrais juste dire que si jamais le conseiller, puis ministre de l'Économie, puis président de la République avait géré les finances de la France comment était géré les finances de l'Allemagne, nous aurions aujourd'hui 1000 milliards de dettes en moins, c'est l'équivalent de 10 plans de relance ou l'équivalent de 30 Plan France 2030. 2030. Est à d'autres collègue Thierry Cozic pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. merci, monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'économie, donc en son absence, je pense que c'est Madame Grégoire, madame la ministre. Le gouvernement a annoncé une recapitalisation du groupe UDF lapsus révélateur. De prime abord, cette décision est louable mais selon cela semblait être un peu l'arbre qui cache la forêt, de fait, l'État actionnaire est à nouveau est à nouveau tombé dans ses 2 pires travers. Les 2 1 milliards que vous allez faire payer aux contribuables vont compenser d'une main ce que votre mesure sur le plafonnement tarifaire a pris de l'autre par cette recapitalisation, le président-candidat qui se veut le président du pouvoir d'achat devient celui du pouvoir de rachat. Et ce rachat, il se fait au détriment de l'intérêt général pour restaurer la confiance des investisseurs privés. La confiance, ça n'a pas de prix et il va en falloir lorsque l'on connaît l'ampleur des chantiers qui attendent EDF dans les 50 prochaines années. Comme je le déplorer, il y a un mois, ce tour de passe-passe ne masque que trop que trop mal votre absence de vision à long terme en faveur d'une politique énergétique sérieux en France. La politique du carnet de chèques ne peut constituer l'horizon indépassable de vos investissements en matière d'énergie. Nous avons déjà perdu 5 ans, et nous ne pouvons plus attendre la crise ukrainienne nous prouve que nous devons être le moins dépendant possible d'entités extérieures au-delà de la question énergétique. C'est une question de souveraineté nationale qui s'impose à nous et ce, alors que nous évoluons dans un monde de plus en plus conflictuels. Un réel état stratège doit opérer, il en va de la protection du pouvoir d'achat de nos concitoyens vos mesurettes ne contiennent que trop peu la flambée des factures d'énergie que vit le pays. Madame la ministre, pouvez-vous dire à la représentation nationale, quelles mesures structurelles, envisagez-vous de fronde afin de garantir la pérennité et la viabilité financière du groupe EDF, condition sine qua non au maintien d'une politique énergétique économiquement soutenables pour tous nos concitoyens. Monsieur le sénateur que zic, je ne vous apprendrai rien et Bruno Lemaire, je le sais, a eu l'occasion de vous le rappeler, EDF traverse un moment un peu particulier, la production d'électricité en 2022 sera faible, elle sera même au plus bas, du fait de l'arrêt de plusieurs réacteurs, vous le savez aussi, ce qui représente une perte de pas moins de 11 milliards d'euros de revenus pour le groupe. Dans le même temps, le président de la République a annoncé depuis Belfort, il y a quelques jours, la nécessité d'investir dans la construction de six nouveaux EPR d'étudier la construction de 8 autres et de lancer 50 nouveaux champs éoliens. Vous le savez nous limitons l'augmentation de la facture d'électricité des Français à 4 % vous parlez de mesurettes, c'est quand même une grosse mesurettes puisque c'est un effort considérable d'EDF qui représente un coût estimé entre 7 7 et 8,4 milliards d'euros grosse mesurettes, dans ces conditions, nous n'aurons de cesse de le rappeler et de le redire : l'État n'abandonnera pas l'État n'abandonne pas et n'abandonnera pas EDF en qualité d'actionnaire de contrôle d'EDF, l'État soutient totalement le plan d'action de l'entreprise qui a été adopté par son conseil d'administration, il y a quelques jours, l'augmentation de capital de 510 millions d'actions va se traduire pour l'État, qui détient près de 84 % du capital par une souscription de 415 millions exactement avec maintien du droit préférentiel, ce qui représente un apport de 2,1 milliards d'euros pour EDF, en second lieu, Monsieur le Sénateur, que l'État va prolonger au moins pour les exercices 2 1000 22 et 23 son engagement actuel qui consiste à percevoir ses dividendes en titres comme le proposera l'entreprise à l'ensemble de ses actionnaires, c'est un double engagement : c'est un engagement d'aujourd'hui, mais c'est aussi un engagement pour demain et l'État réaffirme ainsi sa confiance dans la direction de l'entreprise et dans l'ensemble de ses salariés, ça permettra, monsieur le sénateur à EDF de restaurer ses comptes tout en continuant d'investir dans l'avenir, je vous remercie. la parole est à notre collègue Max Brisson pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président, ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale, monsieur le Ministre, c'est la Cour des comptes qui le dit, donc ce n'est pas la peine, comme hier, de vous mettre en colère contre moi, écoutez vos collègues et puis vous savez, on ne se met pas en colère contre la Cour des comptes que nous, dit-elle, que la performance du système éducatif français reste médiocre, malgré l'importance des moyens mobilisés que les systèmes scolaires et les plus performants sont ceux qui donne plus de place à chaque établissement ce qui fédère la communauté éducative autour d'un projet et encourage les enseignants à être novateur et que, constate la Cour chez nous une autonomie des établissements très encadré, un système éducatif très centralisée, une chaîne managériale qui contrôle fortement les marges d'action des établissements, c'est encore elle qui constate que seuls 10 % des décisions éducatives sont prises au niveau des établissements et 2 % à peine en autonomie totale, ma question est donc très simple, monsieur le Ministre, vous qui êtes depuis 5 ans aux manettes, que pensez-vous de ce constat implacable de la Cour des comptes.

comme à chaque fois que je vais devoir répond non seulement à votre question, mais aussi à ce que vous direz après parce que vous vous laissez un temps important pour après, et donc j'en profite pour faire le le bilan général et le faire à la lumière de ce qu'a dit la Cour des comptes, d'ailleurs je pourrais partager l'essentiel de ce qui vient d'être dit, je voudrais vous indiquer d'abord sur la question de l'autonomie des établissements, mais j'ai l'impression que ça vous a échappé que la réforme du lycée, conduire à une bien plus grande autonomie des lycées parce qu'il y a beaucoup plus de choix et pour l'équipe éducative et pour les lycéens. Mais puisque votre question porte plus globalement sur finalement le bilan que nous avons, je voudrais vous dire. Que de 2017 à 2000 22 et cette attestée par des chiffres que la Cour des comptes connaît aussi les élèves de France à l'école primaire ont progressé, je pourrais vous parler de beaucoup de choses, je pourrais vous parler de devoirs faits au collège, je pourrais vous parler de la réforme du lycée, je pourrais vous parler des cités éducative, je pourrais vous parler de ce que nous avons fait avec les vacances à prenante, maintenant que nous sommes un ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse et des Sports, mais puisque le temps me manque, je me concentrerai sur ce que j'ai affiché comme étant, ma première priorité, c'est-à-dire : lire, écrire, compter, respecter autrui et puisque vous aimez les chiffres, je vais vous en donner, lire à voix haute en CE1, l'écart était de 14,5 points entre les réseaux d'éducation prioritaire et le reste du pays, il est de 7 8 points à la fin de ce quinquennat pour comprendre des phrases lues les élèves qui rentrer en CE1 ont gagné 1, alors même que dans le monde entier l'UNESCO estime que, du fait de la crise sanitaire, les élèves ayant 10 ans sont 50 % de plus désormais à ne pas maîtriser les savoirs fondamentaux dans le monde entier, alors je vous le dis, oui, notre politique de l'école primaire commence à porter ses fruits, les savoirs fondamentaux se sont renforcés et nous serons très certainement un des très rares pays qui a fait cela en traversant une crise très grave non seulement une crise sanitaire mais une crise éducative à laquelle la France a grandement échapper, heureusement pour nous, et nous devons en être fiers, j'en profite pour remercier tous les professeurs de France tous les personnels de l'Éducation nationale et toutes les collectivités locales pour le rôle qu'elles ont joué en la matière, je vous remercie. ministre d'être cet après-midi, tous vos collègues ont été beau joueur, pas vous, promesse, vous avez fait beaucoup promesse : donner plus d'autonomie aux équipes éducatives, bilan : il n'y a jamais eu autant de discours prescriptives de circulaires et de vade-mecum promesse: donner la priorité à l'école primaire, bilan 28 % des élèves ont une maîtrise insuffisante en mathématiques

retisser le lien de confiance entre la société, l'école, bilan 53 % des Français estiment que l'école fonctionne mal, 65 % sont pessimistes quant à son devenir, une proportion qui atteint près de 80 % chez les enseignants, je sais que ce que vous disent les enseignants et les Français du haut, d'autres questions solitaire vous ne voulait pas la tombe et qu'est-ce qu'il vous disent non, définitivement, monsieur le ministre, l'école ne se porte pas mieux aujourd'hui qu'en 2017. Merci. La parole est à notre collègue chante. De pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président, ma question s'adresse au ministre des solidarités et de la santé, monsieur le Ministre, face à la dégradation de la situation sanitaire en Martinique et en Guadeloupe, vous avez lancé au début du mois d'août, un appel à la solidarité nationale, invitant les soignants à se porter volontaires pour partir en renfort dans les Antilles, plusieurs centaines de soignants se sont portés volontaires pour venir prêter main forte aux hôpitaux surchargés, l'arrêté du 17 août 2021 du ministère des solidarités et de la santé portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des profits Neil de santé en exercice ou retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie de Covid 19 prévoit l'indemnisation de ses soignants, or à ce jour, des centaines de soignants attendent toujours d'être rémunérés pour leur travail, il semblerait en effet que cet arrêté ministériel prévoit la rémunération des médecins et des infirmiers mais qu'il ait oublié tous les autres, c'est-à-dire les aides-soignants, les laborantins, elle est kinésithérapeute, par exemple, selon la presse, 6 mois après s'être arrêté, il y aurait ainsi plusieurs centaines de soignants à avoir travaillé gratuitement pour garantir la continuité des soins dans un contexte d'urgence sanitaire, si telle est le cas, ce n'est pas acceptable, monsieur le Ministre, comment se fait-il que des centaines de soignants qui se sont portés volontaires pour aller sur le front du Covid ne soit toujours pas rémunérée.

Merci Monsieur le le président madame la sénatrice, messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice de Seine que cette dernière question à cette dernière séance de questions au gouvernement, soit l'occasion avant toute chose, et avant de répondre à votre question de saluer, nous tous, collectivement, les milliers de personnels qui ont été mobilisés depuis 2 ans pour apporter un appui majeur, la gestion des conséquences de la crise Covid à laquelle nous avons été tous confrontés et, notamment, en particulier nos concitoyens en Outre-mer, depuis le début de la crise sanitaire, nous avons mobilisé toutes les énergies et ressources disponibles, vous l'avez évoqué grâce à des renforts mais aussi par des livraisons, je le rappelle, de matériel de dépistage de façon massive de protection de vaccination ou encore par des opérations inédite d'évacuation sanitaire solidarité nationale a joué à plein pour l'ensemble des territoires ultramarins qui ont connu des périodes difficiles, pendant ces 2 années, ce sont 9000 effectivement, professionnels de santé qui ont été envoyés en renfort dans ces territoires ultramarins pour faire face à l'urgence, la grande majorité a. Fort heureusement, c'est normal bien été rémunérés suite à cette mobilisation. Il existait toutefois un retard de la rétribution financière pour une centaine d'aide-soignants qui des vacataires sans emploi ou retraités, et qui n'étaient pas couverts, c'était un oubli par l'arrêté interministériel de réquisition signée le 17 août 2021, vous l'avez cité, contrairement aux autres aides soignants salariés but personnel mobilisé une soixantaine environ, connaissait le même sort même retard de paiement pour la même raison, et notamment les masseurs kinésithérapeutes, que vous avez évoqué dans votre question, le ministère s'est immédiatement saisi de cette question pour trouver une solution rapide afin de les indemniser de régulariser cette situation qui n'est pas acceptable, vous avez raison de le dire et je partage ce point l'arrêté du 17 août 2021 a été modifié, le 14 janvier 2022 pour permettre à la rémunération de ces aides-soignants non salariés les autres personnels que que j'évoquais les caisses primaires d'assurance maladie procède d'ores et déjà au versement la régularisation des situations a débuté dès la mise à jour de l'arrêter ces versements prendront bien évidemment en compte, comme pour les autres professions listées dans l'arrêté l'ensemble des rémunérations des primes associées les versements une fois encore, sont en cours et la situation va se régulariser dans les prochains jours. Merci monsieur le ministre pour les précisions que vous m'avez apporté dans votre réponse, donc j'ai bien compris que cet arrêté du de mi-janvier devait devrait apporter des solutions rapides aux personnels concernés mais qui, pour certains depuis 6 mois, se trouvent dans des difficultés financières, parce que c'est très bien de saluer l'engagement des soignants sur le front de la crise sanitaire, mais cette reconnaissance, elle passe aussi par une juste rémunération, je vous remercie. Merci, mes chers collègues. à l'occasion de ces dernières questions d'actualité au gouvernement inscrite à notre ordre du jour après sa suspension, je tenais à vous remercier monsieur le 1er ministre pour la constance de votre participation, et j'ai ressenti que malgré, parfois, certains irritants, vous vous sentiez bien au Sénat. Permettez-moi d'associer à ses remerciements, ceux des membres de beaucoup de votre gouvernement qui ont également contribué par leur présence, fidèle à la vitalité de nos propos. Je voudrais saluer le ministre en charge des relations avec le Parlement, tout particulièrement pour la qualité des relations. Il a pu avoir avec nous et qu'il continuera. Nos travaux parlementaires sont à compter de la fin de cette semaine, simplement, je me rappelle mes chers collègues, suspendus. Vous instances nos commissions, nos délégations nos missions d'information de commission d'enquête vont poursuivre leurs travaux de contrôle. Je vous rappelle, mes chers collègues, vous pourrez naturellement continuer à interroger le gouvernement dans les prochaines semaines à travers les questions écrites. Or, à l'approche de la fin de la législature, le ministre en charge des relations le avec le Parlement, le c'est le nombre de questions en attente ne cesse d'augmenter. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, vous m'en voudrez pas, mais vous n'avez répondu votre ministère à aucune question, depuis le 22 juillet de l'année dernière.

En tous les cas, mes chers collègues. Va assurer comme vous le savez la continuité des institutions restera disponible car nous vivons monsieur le 1er Ministre nous avons. Changer sur ce point, nous échangerons vendredi avec les présidents de groupe et le président de la commission des Affaires étrangères. Sur notamment la situation en Ukraine et restera disponible s'il apparaît. Certes, de le réunir en séance plénière, lié à la situation que connaît notre pays et notre continent européen, voilà ce que je voulais vous dire Monsieur le 1er ministre je vous donne la parole. remerciements, Monsieur le Président, Larché que je voudrais élargir, si vous me le permettez à l'ensemble du Sénat puisque, quelles que soient nos divergences, nos sensibilités, nos positions et elles sont évidemment bien légitime dans une démocratie, la première chose que je voudrais vous dire depuis que j'ai eu l'immense honneur d'occuper ses fonctions de chef du gouvernement, c'est-à-dire depuis juillet 2020, c'est que nous avons beaucoup travaillé au service de notre pays, ai-je besoin de rappeler parce que cela ne se sait forcément pas toujours, et qu'en dehors de la crise sanitaire et des textes législatifs que celle-ci à supposer le gouvernement et le Parlement ont eu une activité intense, j'ai fait un petit calcul : Monsieur le président, je ne sais pas s'il est rigoureusement exact mais pas loin, l'activité législative par exemple a été équivalente à ce qu'elle était dans une période hors Covid donc ça veut dire que nous avons finalement doublé notre travail, notre action au service de ce concitoyens et c'est une chose que je voulais souligner devant vous, parce que ça n'aurait pas pu faire évidemment dans le cadre de nos prérogatives respectives sont une collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, je voulais vous dire simplement que j'ai essayé d'exercer ma fonction dans le plus grand respect des assemblées parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, je vous ai toujours parler, vous avez parlé d'irritants monsieur le président, il y en a eu quelques fois, mais en tout cas je vous ai dit toujours ce que je pensais avec sincérité et soyez assurés dans le seul but de rechercher l'intérêt général, je pense que ce respect dû aux assemblées de parlementaires, il tient aussi au respect qui est le mien de la Constitution et des institutions de la Ve République, auquel j'ai pu, à de multiples reprises vous dire mon profond attachement. Et je pense qu'il est particulièrement nécessaire, il l'est toujours mais dans les moments de crise, de tension et de difficulté très forte que traverse depuis de très longs mois nos concitoyennes et nos concitoyens, je voudrais monsieur le président, adressé des remarques ciment particulier à vous-même, aux institutions qu'ensemble, nous avons créé, je pense à ces comités de liaison pour renforcer le lien entre l'exécutif et le législatif, je voudrais remercier chacune et chacun des présidents de groupe, toutes tendances confondues, avec lesquels je pense avoir noué des relations de respect et de confiance, voilà, je ne serai pas plus : plus long et bonne route à notre démocratie parlementaire.

L'ordre du jour appelle une déclaration du gouvernement, suivie d'un débat sur cette déclaration en application de l'article 50 Thierry 1 de la Constitution relatives à l'engagement de la France au Sahel et c'est une demande du gouvernement. Je donne la parole à Monsieur le 1er ministre Jean Castex, monsieur le 1er ministre.

Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, la semaine dernière, le président de la République, entouré des présidents du Conseil européen. De l'Union africaine et de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a annoncé, en lien avec nos partenaires européens et africains les principes d'un engagement renouvelé au Sahel, cette décision s'inscrit. En cohérence avec l'annonce de la réorganisation de notre dispositif. Qui vous vous en souvenez, avait été faite par le chef de l'État au mois de juin dernier, tout en prenant acte d'une dégradation des conditions politiques. De notre présence au Mali. Cette décision a été prise collégialement dans un cadre partenarial totalement préservée, aussi bien avec nos alliés africains qu'européens, elle traduit notre volonté. Et notre détermination à poursuivre, je le dis d'emblée notre engagement dans l'esprit de Takuba dans la lutte contre les groupes terroristes islamistes au Sahel. Cette nouvelle donne, nous conduit à renouveler et à adapter notre dispositif en accélérant, finalement, un certain nombre d'évolutions décidées ces 2 dernières années, en particulier lors des sommets de peau et de N Djamena. Ces considérations, en effet, monsieur le président du Sénat m'ont conduit à demander que soient soumis à la représentation nationale, en ma qualité de chef du gouvernement, une déclaration au titre de l'article 50 tirer 1 de la Constitution, portant sur la réarticulation de notre engagement au Sahel et cette déclaration sera suivie d'un débat. Depuis plus de 9 années maintenant l'action des gouvernements qui se sont succédés, a été marqué, je le crois, par la plus grande transparence dans l'information des assemblées parlementaires. J'en veux pour preuve la constance avec laquelle. Votre commission des affaires étrangères. De la défense. Et des forces armées, sous l'impulsion de son président, que je salue tout particulièrement à travailler sur ce sujet, auditionnant régulièrement les mini-ça les chefs militaires concernés et produisant des travaux d'une très grande qualité le débat que nous allons avoir doit nous permettre de répondre aux interrogations des Françaises et des Français. Il est également l'occasion de nous incliner à nouveau devant le sacrifice de nos 59 soldats morts au Sahel au service de notre pays depuis le mois de janvier 2013 j'ai mesdames et messieurs les sénateurs, en cet instant une pensée toute particulière pour eux, pour la famille et pour leurs camarades blessés. Je veux également dire à tous nos militaires qui mettent leur engagement et leur courage au service de la sécurité des peuples ça il Combien notre fierté et grande et notre soutien total. Plus largement, l'action de la France au Sahel est également l'oeuvre de beaucoup, diplomate, gendarmes, policiers, agents de l'État personnel du secteur privé qui incarne partout là-bas. Nous ne l'oublions pas, comme nous n'oublions pas nos journalistes enlevés et assassinés à Kidal en novembre 2013, ni nos jeunes humanitaires qui ont perdu la vie au Niger. Anne, août 2020 lâchement abattu par des terroristes fanatisés, L'une de mes premières missions comme 1er ministre que d'aller accueillir. Leur sépulture à l'aéroport d'Orly. J'ai également une pensée pour tous nos ressortissants, donc je veux dire ici que la sécurité fait l'objet de toute notre attention, enfin je veux solennellement réaffirmer notre soutien et notre amitié aux populations sahéliennes qui sont finalement en première ligne face aux groupes armés et qui subissent de plein fouet l'insécurité alors qu'elles vivent par ailleurs souvent dans une extrême pauvreté. Notre débat doit être. Dans ce contexte, empreint de dignité et de responsabilité, quand vous le savez, par ailleurs, les forces informations et les manipulations en tous genres, nourrissent des soupçons et les fantasmes. Mesdames et messieurs les sénateurs, notre présence au Sahel et fondée depuis le 1er jour sur un objectif clair : lutter à la demande des pays de la région contre les groupes terroristes et contribuer à en protéger les populations. Et nous avons de ce point de vue, obtenu des résultats incontestables en 2013, vous le savez bien, le Mali était au bord de l'effondrement et son armée n'était que l'ombre d'elle-même, le nord du pays était passé sous le contrôle de groupes armés liés à Al-Qaïda et la décision courageuse du président Hollande de répondre positivement à l'appel pressant des autorités maliennes et des autorités régionales a permis d'enrayer une offensive dit à East, qui avaient atteint le centre du pays et menaçaient Bamako en quelques semaines par une action audacieuse et déterminée de nos forces armées, la progression des groupes terroristes a été stoppée et les repaires jihadistes du nord du pays, ont été démantelés. Si nous avons empêché le Mali de s'effondrer. Nous avons également neutralisé les projets d'installation d'un proto-État inspiré par l'idéologie islamiste la plus radicale la création d'une zone sanctuaire pour les groupes terroristes qui aurait constitué un péril mortel pour la région et pour notre sécurité, a été entre. Mais je veux rappeler ici que notre présence militaire au Sahel, dans le cadre multilatéral qui a le sien. Nous a permis depuis lors et jusqu'à récemment encore des succès significatifs N'ont laissé aucun répit aux groupes terroristes, qu'ils soient affiliés à Al-Qaïda ou âge et les objectifs. Qui leur avaient été fixés ont été pour l'essentiel, atteint, je veux en particulier rappelé l'élimination de plusieurs chefs internationaux de ces mouvements. Ceux de la filiale sahélienne d'Al Qaïda que nous avons combattu dès 2013 et dont nous avons neutralisé les principaux responsables dans leur numéro 1, c'était en juin 2020, l'émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique membre du haut commandement d'Al-Qaïda. Mais aussi ceux de Daech, au sommet de Pau, début 2020 les chefs d'État se sentent accordé, je vous le rappelle, pour concentrer leurs efforts contre la filiale de Daech au sein l'État islamiste du Grand Sahara qui s'installait dans la zone dite des trois frontières aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso, ces efforts aussi ont été couronnés de succès puisque nous avons neutralisé les 4 plus hauts cadres de cette organisation entre mai et et septembre 2021, dont le fondateur, en plus d'affaiblir durablement les organisations terroristes, cela a modifié l'envergure de leurs ambitions, les amenant à renoncer à l'instauration d'un califat territoriaux. Par notre action résolue contre le terrorisme, je veux solennellement le à le rappeler devant la Haute Assemblée et surtout devant les Françaises et les Français. Qui se demandent toujours parfois pourquoi nous sommes là bas nous participons activement à la protection de nos compatriotes dans la région et nous empêchons ces groupes jihadistes de créer une base territoriale et d'acquérir une liberté d'action, leur permettant de se projeter dans des attaques qui pourrait toucher le sol national. Ces succès, nous ne les avons évidemment pas obtenu seul. Ils sont d'abord le fruit d'une volonté des États du Sahel de traiter ensemble les défis qui se posait à eux à travers le G5 Sahel que nous soutenons de manière active. Autre élément essentiel de notre action politique, elle visait à impliquer de manière croissante les États européens à notre démarche, avec une véritable prise de conscience chez nos partenaires que la sécurité pas simplement de la France de l'Europe se joue aussi dans cette région du monde aujourd'hui, grâce à l'action patiente et persévérante de la France et de l'Union européenne au travers d'EUTM Mali: l'armée malienne a été reconstituée, c'était une priorité stratégique et nous avons eu un rôle déterminant dans cette reconstruction en formant plus de 15000 cadres et soldats la force Takuba au sein de laquelle 10 pays européens se sentent engagés progressivement ensemble aux côtés de l'armée malienne incarne, me semble-t-il, également, cette évolution du rôle de l'Europe. Est ce que les Européens sont capables de réaliser dans des environnements sécuritaire complexe. Autre orientation majeures bien connu du Sénat. L'approche globale qui est la nôtre, à travers 4 piliers complémentaires de nombreux acteurs. Se sont mobilisés dans le souci de produire une réponse large et transversal aux immenses défis de cette région. Le terrorisme mais aussi plus globalement l'insécurité prospère en prenant appui sur la pauvreté mais aussi sur la faiblesse, voire parfois l'absence de l'État et de ses services aux populations, si bien que la réponse de fond au phénomène insurrectionnel et au terrorisme, ce sont des autorités démocratiquement légitime, c'est la présence de l'État de droit, c'est le développement économique et social, l'Alliance pour le Sahel n'comme vous le savez, en 2017 et consolidé au sommet de Pau en janvier 2020, qui incarne le mieux cet engagement de la communauté internationale dans toutes les directions, avec plus d'un millier de défaut de projets de développement qui ont été financés. Oui, mesdames et messieurs les sénateurs, notre action s'est fondée sur le principe, re-rappelé avec force encore récemment par le président de la République que l'intervention d'une armée étrangère ne peut se substituer à l'action d'un état souverain ni s'émanciper d'un cadre multi-latérales. En sortant du cadre de la transition, les autorités maliennes ont clairement choisi de rompre avec la communauté internationale, la France et ses partenaires africains et européens se devait de tirer toutes les conséquences de ce choix grave du pouvoir malien. La communauté internationale a aujourd'hui comme interlocuteur au Mali des autorités, de fait, issu d'un double coup d'état et qui ont renié un parrain leurs engagements dans quelques jours, vous le savez, il aurait dû y avoir. Des élections au Mali. Consacrant la fin d'une période de transition qui dure déjà depuis plus de 18 mois, il n'en sera rien car la logique qui prévaut et le maintien au pouvoir de la junte, le plus longtemps possible la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et l'union économique et monétaire ont placé le Mali sous un régime de sanctions très strict, l'Union européenne, la communauté internationale et bien sûr la France sont pleinement solidaire de cette décision, ce régime a fait par ailleurs le choix de s'appuyer sur une organisation privée bien connue de mercenaires russes Wagner dans le modèle économique repose sur la prédation des richesses des pays dans lesquels elle opère opère le constate en particulier en Centrafrique, cette milice nourrit la guerre car la guerre la nourrit ses exactions contre les populations ces entraves à la mission des Nations unies sont multiples et documenté, sacrifiant les conditions d'une paix durable l'appui européen et international dans lequel la France s'inscrivait et s'inscrit à la demande des autorités maliennes s'exerce quant à lui, sans aucune contrepartie financière, ni intérêts cachés, il n'est aujourd'hui plus possible de nous investit dans un pays dont les autorités ne souhaitent plus coopérer ni avec les Européens, ni avec leurs voisins africains et entrave leur capacité d'action à l'image du mauvais procès fait récemment à nos alliés danois qui souhaitait s'engager dans la force Takuba peut-on imaginer un seul instant poursuivre nos efforts diplomatiques financiers et notre coopération alors que nous sommes accusés de mettre à 9 un agenda caché qui irait à l'encontre des intérêts du peuple malien. La prise en compte de cette réalité impose de repenser notre dispositif en le repositionnant en dehors du territoire malien, mais toujours dans l'objectif de lutter contre les terroristes sur le plan militaire, nous serons donc amenés à fermer les bases de Gossi Ménaka et enfin Gao la manoeuvre s'effectuera en bonheur d'insécurité, comme l'a précisé le président de la République et durera entre 4 et 6 mois, nous allons d'ailleurs renforcer notre dispositif logistique à partir de la métropole, les opérations seront conduites de manière intégrée avec nos partenaires de Takuba car la France assume son rôle de Nation cadre et agit en responsabilité, elles devront aussi être exécuté en bonne Intelligence et en coordination avec les forces armées maliennes et bien sûr la Minusma et nous nous y employons, d'ores et déjà, Madame la Ministre des armées nous conduisons. Ces opérations suivant notre calendrier et notre organisation en donnant la priorité à la sécurité de nos soldats et à celle de nos ressortissants. Le Niger a fait part de sa disponibilité pour faciliter cette évolution du dispositif, nous permettant ainsi de faire transiter nos flux logistiques jusqu'au port du Golfe de Guinée, mais aussi d'envisager notre redéploiement dans d'autres pays de la région, j'y reviendrai. Notre appui au peuple malien que nous respectons profondément sera préservée au travers des programmes de l'alliance pour le Sahel sous réserve évidemment que ces programmes ne puisse faire l'objet d'aucun détournement pour faciliter des mercenaires ou le terrorisme, nous continuerons de la même manière d'oeuvrer pour que la Minusma s'puissent pleinement remplir son mandat au profit, là encore, de la protection des populations et en soutien de la mise en oeuvre de l'accord de paix d'Alger. C'est donc sur des bases renouvelées que nous allons mesdames et messieurs les sénateurs, poursuivre notre engagement contre les groupes terroristes au Sahel. Il Il n'y a pas que l'attitude de la junte au pouvoir au Mali, qui conduit la France et ses alliés à adapter leur approche et réarticuler leur dispositif. Il nous faut tout pour. Temps prendre en compte l'état de la menace, l'état de la menace terroriste qui a évolué sous l'effet de l'action conduite par la coalition ligués contre elle. Ne pouvant, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, constituer un sanctuaire, les groupes liés à Al-Qaïda ont dû se disséminer. Dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, l'attaque du 9 février dernier au Nord du Bénin, dans laquelle un de nos compatriotes, a été tué et à laquelle nous avons vigoureusement réagi en neutralisant dans le sud du Burkina Faso, où ils avaient trouvé refuge, une quarantaine de terroristes, cette attaque en témoigne avec une douloureuse actualité cette reconfiguration de la menace terroriste, au-delà des évolutions du Mali nous conduit donc aussi à adapter notre stratégie et notre organisation. La première révolution de notre engagement et précisément en lien avec la dissémination de la menace, malgré la défection de la junte malienne le G5 Sahel demeure un cadre pertinent pour coordonner les actions. Cependant, il y a aujourd'hui une nécessité d'adapter la réponse en l'élargissant aux zones périphériques du Sahel et la France continuera de jouer un rôle fédérateur, nous parlons ici de zones vulnérables situés aux frontières nord de pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire le Togo ou le Ghana. Nous nous appuierons pour cela sur le cadre multilatéral existant de l'initiative dite d'Accra évidemment toujours un lien avec la CEDEAO. Nous sommes déjà évidemment en pourparlers avec les pays de la région, mais je veux ici être clair. La lutte contre le terrorisme, finalement ne sera gagnée localement que par les Africains eux-mêmes. Dès lors, nous devons leur apporter un appui adaptée en construisant l'avenir avec eux, avec méthode et sans précipitation, nous avons donc la volonté partagée avec nos partenaires d'être encore davantage en soutien des États et de leur population, en partant de leurs besoins, pour pouvoir mieux y répondre en complément de ce qui se fait déjà en matière de coopération et d'aide au développement, nous nous appuierons sur l'Alliance pour le Sahel qui, depuis 2017. Permet de fournir ce soutien aux acteurs locaux qui déploient des politiques publiques et des programmes en matière de développement ainsi un effort doit être clairement porté sur le volet civil de prévention à travers des actions concrètes en soutien de secteurs clés, je pense notamment à l'éducation à la justice et au domaine social qui permette d'affirmer la présence de l'État et de renforcer la société civile. La 2ème évolution réaffirmée par le président de la République, jeudi dernier, à l'issue des concertations approfondies conduites avec l'ensemble de nos partenaires concerne la physionomie de notre présence militaire dans un contexte de très grande sensibilité des opinions publiques et je l'ai dit de d'évolution de la menace. Notre approche c'est clair doit être encore plus intégrés, qu'elle ne l'est déjà, il s'agit de mettre en oeuvre un dispositif plus souple, plus Agile, plus modulable reposant sur des implantations dans la taille et la localisation, doivent être revues, nous l'avons déjà évoqué avec le président Cambon. Ce redéploiement s'effectuera d'abord au Niger puis dans les pays voisins, selon des décisions prises ensemble, la France dispose dans la région, je vous le rappelle, de forces prépositionnées en république de Côte d'Ivoire et au Sénégal, qui pourront venir en appui des États et de leurs forces de défense et de sécurité lorsque cela sera nécessaire, et bien entendu, sur leur demande, elle, conduite également des actions de coopération civile et militaire au profit des États du Golfe de Guinée, lesquels pourront être développés ou réorienter à l'image de ce que nous avons construit précédemment, nous voulons poursuivre notre engagement avec nos alliés européens qui l'ont réaffirmé avec force la semaine dernière, selon le même, pardonnez-moi cette formule esprit Takuba qui a fait la réussite de ces opérations. Mesdames et messieurs les sénateurs. La présence de la France au Sahel. Doit évoluer. Pas seulement parce que l'évolution de la position du gouvernement de fête Malia a changé. Et bien sûr en partie pour cela, la France et c'est son honneur respecte profondément la souveraineté des États, c'est l'État malien qui a sollicité avec ceux de la zone, l'intervention de la France et de la communauté internationale en 2013, nous prenons acte du changement radical opéré par la junte malienne, mais nous ne renonçons en rien à ce qui est la justification majeure de notre présence au Sahel, la lutte contre le terrorisme islamiste pour protéger la zone et les populations qui vivent pour assurer aussi, comme je l'ai dit la sécurité de notre propre pays et nous avons obtenu de réels succès dans des conditions extrêmement difficiles et qui le demeure grâce à l'engagement exceptionnel de nos soldats et parfois au prix de l'avis de certains d'entre eux nous continuerons. D'appliquer les principes fondamentaux qui structurent notre intervention dont nous nous sommes attachés à renforcer l'effectivité, la concrétisation ces dernières années et qui vante encore d'la phase nouvelle qui s'ouvrent le multilatéralisme, à la fois, bien sûr, je l'ai dit, avec les États de la zone, ce qui n'est pas simple, vu la fragilité de beaucoup d'entre eux et des graves difficultés qu'ils doivent affronter, mais aussi avec l'implication politique et militaire de nos partenaires et amis européens, là encore, le Sénat connaît toutes les contingences qui peuvent freiner ce mouvement mais elle a aussi. Patiemment, nous avons agi et progresser, c'est l'intérêt de l'Afrique, c'est l'intérêt de l'Europe, c'est l'intérêt de la France, qui a joué, joue et continuera à jouer un rôle essentiel auprès de l'Union européenne en la matière. Second principe le recours à une approche de plus en plus globale et prenant davantage en compte les intérêts des populations des sociétés civiles et des opinions publiques leur acceptation être aussi une clé de la réussite de nos interventions, les questions majeures de sécurité sont imbriqués avec d'autres problématiques et ai-je besoin de rappeler ici, Monsieur le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, la vision qui est la nôtre et que nous portons en matière d'aide au développement, notamment depuis la loi novatrices et ambitieuses proposées par le gouvernement et voté à l'unanimité du parlement l'été dernier, là encore, nous avons collectivement progresser en dépit d'innombrables difficultés car ainsi va le monde, c'est bien dans ce cadre global et pour mieux un assurer l'effectivité que s'inscrit la réorganisation de notre dispositif militaire en réponse aux évolutions des réalités géopolitiques de cette zone et plus globalement de l'ensemble du monde réorganisation qui est, je le crois mesdames et messieurs les sénateurs, profondément conforme. à la fois aux intérêts de la France. De l'Afrique et de l'Europe, je vous remercie. Merci monsieur le 1er miné. Dans Dans la suite de notre débat, je vais donner la parole aux orateurs des groupes. Oui, d'abord la parole au au président, Bruno Retailleau, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, Monsieur le 1er ministre madame. Messieurs les ministres, monsieur le président de la commission chers Christian Cambon, chers collègues, ce débat est un peu particulier puisque vous venez de le rappeler, Monsieur le 1er ministre il intervient après la décision, puis l'annonce de cette décision du président de la République de retirer nos forces du Mali pour Les réarticuler ailleurs au sel. Je ne veux pas polémiquer parce que je pense que pour ce débat, nous devons avoir la bonne hauteur. La bonne hauteur d'abord vis-à-vis de nos armées vis-à-vis de nos armées, que nous avons envoyé combattre là-bas pendant près de 10 ans sur un terrain très, très difficile, et ils l'ont fait, au nom de la France, la bonne hauteur aussi parce que nous pensons tous ici, quelles que soient les bancs que nous occupons assez 59 soldats qui ont laissé leur vie. Et je voudrais dire, peut-être avec mes mots à leur famille, peut-être certaines nous écoute-t-il. Que, ils ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour la France, ils sont morts pour nos valeurs, ils sont morts pour protéger le sol français. D'attaques terroristes, peut-être, et ils sont tombés. Sur le Champ d'honneur pour que ne tombe pas le Sahel aux mains des pires ennemis de la France. Je veux dire aussi, Madame la Ministre, que nous pouvons et nous devons même. être fiers de ce qu'on fait en Afrique, nos armées, vous l'avez rappelé Jean Castex. Vous l'avez rappelé Serval a été un succès en 2 mois 400 jihadistes tués en 2 mois, les principales villes du Nord libéré. Et aussi en quelques semaines, les principales bases de ces terroristes neutralisés sans la France sans l'intervention de la France au Sahel et au Mali, nous aurions eu Raqa. Là-bas. Et il faut le redire, nous aurions eu en réalité la constitution de ce proto-État d'un État islamiste d'un califat au coeur du sel. Donc, rappelons ici solennellement avant ou au début d'engager ce débat que ce qu'ont fait nos militaires. Que ce qu'a fait l'armée française en Afrique. Très peu d'armée très peu d'armée, on doit en être conscient. Aurait pu le faire. Dans ces conditions. Sur un territoire aussi large. Avec des moyens finalement assez limité. Et je pense que leur mérite nous oblige. Il nous oblige à ce que nous-mêmes d'ailleurs sur le sol français. Nous soyons intransigeants avec les menaces islamistes. Que notre main ne tremble jamais ici en France, le front est extérieur, le front il est aussi intérieure. Mais il nous oblige aussi à ce que leur réarticulation le retrait se passe dans la dignité, madame et vous y répondrez j'espère vous donnerez les garanties pour que ce retrait ce redéploiement soit totalement sécurisé. La bonne hauteur, ça signifie pour notre débat. Un débat honnête. Parce que franchement. à quoi sert un débat si c'est un débat convenu débordant d'autosatisfaction. ça ne nous empêche pas de reconnaître, je viens de le dire. Que Serval. à a été un succès que nous avons ensuite dans l'opération Barkhane engranger des victoires, vous avez rappelé en juin 2020. Nos troupes ont tué le leader d'Aqmi. Vous avez rappelé aussi que l'État islamique au Grand ça, elle avait été pratiquement neutralisé. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Allons au-delà et plus profondément dans l'analyse. Avec, non pas l'opération Serval mais la continuation de Barkhane nous avons fait un pari, ce pari et reposait sur le fait que nous puissions réduire contenir ces groupes armés en attendant la relève la relève des forces locales. Je pense que ce pari, nous n'avons pas pu le gagner. Parce que dans cette course de vitesse. Qu'il existe entre eux une érosion naturelle des opinions publiques manipuler sa guerre informationnelle. Fait partie des armes aujourd'hui presque conventionnel. Il faut aussi la contrée et nous n'avons pas pu bien la contrée mais cette érosion finalement ce ce double mouvement l'érosion dans le temps du soutien des opinions publiques et puis la montée en régime en puissance des forces locales cette course de vitesse, nous l'avons perdu. et, aujourd'hui, en essayant d'être un peu objectif lorsqu'on regarde sur le plan politique, diplomatique. Ou même militaire que se dit-on, est ce que la présence de la France en Afrique, dans cette zone a été renforcée dans son influence, je ne le crois pas. Est ce que la menace jihadiste a été fortement réduite, je ne le crois pas non plus. Elle a plutôt augmenté, elle menace désormais des pays dans le Golfe de Guinée. Que s'est-il donc passé, je pense que il y a eu, à travers les succès des erreurs des erreurs d'ordre militaire. Des erreurs d'ordre diplomatique. Les héros militaire sans doute pour Barkhane et sa prolongation a été lorsque nous avons au début engagées Barkhane de penser que nous pouvions nous disperser à l'époque, je vous rappelle l'opération Sentinelle sans doute était telle nécessaire l'Irak sans doute était-ce une opération si nécessaire mais dans le format de nos armées se diviser, se disperser, c'était finalement s'affaiblir parce que on ne gagne ce genre de guerre quand tapant vite et très fort. 2ème élément concernant l'aspect militaire, il y a eu un certain nombre d'illusions, je pense que c'était beaucoup présumé de penser que, en très peu de temps, nous pouvions relevé une armée comme celle du Mali, qui était une des armées les plus faibles et les plus corrompus d'Afrique, c'était sans doute une illusion, même sans doute fallait-il le faire, de croire que le G5 Sahel la force pouvait exister en tant que telle, sans la perfusion française sens habitude culture de planification. D'État-Major commun. Une grammaire en réalité d'une intervention sur le terrain qui est essentielle lorsque on veut être efficace. Vous avez parlé de Tabqa comme de l'esprit. C'est cela, si je file la note fort tabou qu'a été de leur Takuba était de l'ordre de l'esprit dans une dimension. Si j'ose dire, un peu immatériel. Vous enlevez les 400 militaires français de Takuba, qu'en reste-t-il l'esprit oui l'esprit seulement l'esprit quant à la minute pas, peut-être faut-il reconnaître, chers collègues, qu'elle a toujours été incapables de faire autre chose que de se protéger elles-mêmes, et encore, avec l'appui de nos forces, voilà pour les militaires, maintenant je pense que les erreurs les plus conséquences ont été des erreurs diplomatiques, la première erreur d'analyse a été lorsque le président de la République a annoncé, je crois que c'était en juin 2021 juste après le sommet de Pau, sans grande concertation avec nos partenaires africains un retrait progressif ce retrait progressif, il a été un double signal, un signal vis-à-vis de la junte, qui l'a saisie comme un prétexte et évidemment je rejoins monsieur le 1er puisque vous avez dit sur la junte évidemment mais vous comprenez que devant ce signal, la junte la CENI la saisie comme un prétexte pour aller dans les bras, justement, de Wagner et d'une autre puissance que la puissance française et puis vis-à-vis nos propres partenaires qui étaient réticents à s'engager plus au moment même où ils ont entendu ce signal, on leur disait : On Va Se progressivement certes mais se retirer, ça n'est pas à croire que, eux, dans un mouvement inverse il allait substantiellement se réengager, c'est en ce sens que je pense que il y a une erreur diplomatique, je pense que la plus grosse erreur, c'est la politique africaine. Je pense que la plus grosse erreur a consisté, et je la date du discours de Ouagadougou du président de la République, c'était très tôt dans son quinquennat je crois que c'était en novembre 2017 lorsque, il y a une réinterprétation de la politique africaine. Cette politique africaine devant se baser notamment, c'était un pari l'encore sur la société civile africaine mais. Les représentants de cette société civile étaient en fait des représentants, comment comment dire, de la diaspora africaine. Souvent issus de la grande bourgeoisie, avec une représentation franchement il était une représentation qui peut-être contestable, mais nous nous sommes détournées des autorités, les autorités de fait ou de droit, peu importe, de ceux qui gouvernaient, un certain nombre de pays et nous avons créé, par exemple, bien sûr, le Conseil présidentiel pour l'Afrique et de proche en proche, nous avons désorienté nos partenaires, je veux rappeler que dans un certain nombre de réunions, la voix, données aux autorités publiques était une voix, données, parmi d'autres dans des ateliers, donc il y a une profonde désorientation et je pense que nous avons affaiblit notre politique africaine alors en disant cela, que faire désormais. Se retirer pour tirer un prêt surtout ce que nous avons fait, évidemment, non, je vous rejoins, il faut bien sûr rester au Sahel se redéployer dans les conditions que vous avez cité il y a quelques instants, je n'y reviens pas notamment à Niamey au Niger, mais je pense que il faudra aussi pour l'avenir, réexaminer tirer un certain nombre de leçons parce que on on peut tirer bien sûr des leçons de cette expérience et je pense que très largement ce que m'inspire pas Serval, mais surtout Barkhane et sa continuation ces 3 leçons qui sont des leçons qui tiennent à nos illusions françaises, je crois que la première illusion c'est que on ne peut pas dans un état quasi faillite finalement avec une action militaire qui ne combine pas efficacement une action civile de développement aboutir à des résultats, c'est une illusion très occidentale mais définitivement la France peut être une force d'action rapide en Afrique, c'est à dire que la France peut être un pompier mais qui est un incendie, mais la France ne peut pas être le gendarme qui restaure, ça c'est un 1er point qui est important et qui je crois est une illusion largement partagé en Occident 2ème illusion c'est l'illusion européenne peut-on se servir, entre guillemets, des Opecst comme un terrain d'entraînement pour constituer ce qui peut être un embryon d'armée européenne, je pense que on y trouve très vite des limites, je l'ai dit tout à l'heure, sans la France sans la France takuba avaient des difficultés à vivre et en réalité derrière Takuba c'était la France et la 3ème, illusion, c'est la politique africaine je pense que cette politique africaine entre l'angélisme que nous semblons avoir et la Real politique évidemment que d'autres puissants, je pense à la Russie, je pense à la Chine déploie sur le continent, il y a sans doute une marge cette marche peut-être c'est le réalisme c'est faire avec les autorités, les autorités qui sont en place, dialoguer parce que le propre de la diplomatie c'est de dialoguer, parfois avec des partenaires qui sont parfois peu recommandables, mais le réalisme, je pense être absolument nécessaire si on veut demain avoir une diplomatie un peu efficace, voilà pour terminer ce que je veux vous dire et pour l'avenir, je pense que on peut d'abord redire que parmi les 27, nous sommes le seul pays, la seule nation désormais qui dispose d'un modèle complet d'armée capable de se projeter à l'extérieur et et c'est quelque chose de fondamental qu'il faudra entretenir et nous parlementaires nous ne l'oublierons pas dans les projets de loi de finances cher Christian Cambon, le 2ème élément sur lequel je souhaite terminer mais l'Afrique est un continent en devenir démographique, elle est instable et l'avenir de l'Afrique nous concerne l'avenir de la l'Afrique engage notre destin et et je pense que nous devons à travers nos actions toutes nos actions, pas seulement militaire, diplomatique, mais aussi avec l'AFD, Dieu sait si, dans cette enceinte, nous avons parfois réclamait beaucoup, beaucoup plus de transparence, une meilleure articulation entre l'action militaire et l'action, si l'action humanitaire, la France, mais surtout l'Europe et la première puissance humanitaire si demain on veut convaincre les populations parce que, aujourd'hui, quelle est la situation, la présence de la France hier était souhaitable, désormais les redoutés et les presque même repoussé donc recombinant nos forces parce que la France doit rester en Afrique, c'est notre histoire mais c'est, je pense aussi un destin commun et notre avenir, merci. La parole est notre collègue Jean. Le peu de ce qu'il nie pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le président, Monsieur le 1er ministre Madame et messieurs les Ministres, chers collègues, il y a 3 semaines, lors d'une question d'actualité au gouvernement, le président du groupe socialiste, écologiste et républicain nous a demandé ce débat mais ce 1er ministre c'est un enjeu démocratique est une bonne manière de construire une politique internationale efficiente et durable tout au long de ce quinquennat le président Macron a préféré une approche descendante dans la relation entre le pouvoir exécutif et législatif, la preuve, ce débat arrive après la décision présidentielle, c'était donc plus véritablement un débat pourtant il serait dommageable d'en faire un moment d'opposition caricaturale ou un quitus des décisions élyséennes avant toute autre considération, nous pensons avec gravité, à celles et ceux qui ne sont plus là, ils sont morts pour la France pour ce qu'elle est et représente ici et dans le monde pour ces 3 mots qui la fondent, liberté, égalité, fraternité, je ne pensais émue pour leurs familles et leurs proches, mes fonctions passées m'amenés à les rencontrer et j'ai pu mesurer leur courage dans ces épreuves tragiques, je veux leur dire que la flamme du souvenir de de s'étendre à jamais. Elle ne compensera ni le chagrin, ni la tristesse de celles et de ceux qui restent, mais notre mémoire ne les oubliera pas permettez-moi aussi d'apporter notre soutien unanime à tous les blessés et à leurs familles, la République est et sera à leurs côtés ici je veux saluer le travail du service de santé des armées et des personnels de l'Institut National des invalides sans eux aucune projection de nos armées ne serait possible. Alors que le départ du Mali est annoncé comme vous l'avez fait aussi monsieur le 1er ministre nous pensons à toutes les ONG qui oeuvrent sur le terrain au service des populations locales à tous ces journalistes aussi qui, par leur travail, permettre de faire vivre la liberté et la démocratie, j'ai ici une pensée pour Olivier Dubois enlevés dans la région de Gao, il y a 10 mois et dont la famille sont nouvelles attend de soutien du gouvernement français Depuis 9 ans, les armées françaises, sont engagées dans un théâtre d'opérations complexes faisant preuve d'un professionnalisme sans faille. Répondant à l'appel du gouvernement malien menacé par des groupes jihadistes. Nos troupes sont intervenus en quelques heures, en 2013, sur décision du président François Hollande comme vous l'avez aussi rappelé l'opération Serval a consisté à se projeter rapidement et apporter d'initiative aux confins du Sahel pour protéger la démocratie et les populations menacées, ni plus ni moins, cette opération n'a jamais été une offensive de conquête, il faut le dire et le redire, les armées françaises, européennes, non, à aucun moment, étaient des forces d'occupation en chaque instant, elles se sont inscrites dans un cadre relationnel clair avec l'ensemble des 5 pays concernés géographiquement par l'opération Barkhane, dont en 1er lieu le Mali Barkhane a été initiée pour procéder à une autonomisation des forces armées locales singulièrement cette armée malienne fortement affaiblis et incapables de faire face à la menace qui acculer, en janvier 2013. En ce sens, l'accord signé le 16 juillet 2014 entre les ministres maliens et français de la Défense, précisé que l'opération Barkhane identifier les principaux domaines de coopération de défense, l'échange d'informations et consultations régulières sur les problèmes sécuritaires formation conseil Entraînement et équipement, bien entendu, il s'agissait de permettre au Mali de faire front face à la poussée djihadiste et de raffermir sa souveraineté, celle d'un pays démocratique, de lui donner la stabilité nécessaire pour administrer librement l'ensemble de son territoire au service des Maliennes et les Maliens. Il ne s'agissait pas de construire un autre état ou d'imposer telle ou telle partie au peuple malien, voilà ce qu'étaient les objectifs de l'opération Barkhane ni plus ni moins, dans ce contexte, les armées françaises n'ont jamais été défaite sur le terrain militaire en chaque instant ces femmes et ces hommes, tous ces personnels des armées de terre, de l'air et de et de maire, qu'ils soient en première ligne, ou en soutien, tous ont affronté le feu qu'ils oeuvrent dans l'ombre ou dans la lumière toutes et tous ont su se distinguer aujourd'hui, il nous revient à nous, parlementaires, au nom de tous les Français de les honorer, on fait l'instant nous affirmant que les annonces de ces derniers jours ne sont pas celles d'une défaite militaire mais la marque visible et durable d'un manque de clairvoyance, de la part de l'exécutif pour la stratégie quant à la stratégie de la France au Sahel, ce que ne pointant ce n'est pas tant la décision de quitter le Mali, c'est que cette décision soit prise sous la contrainte et non pour répondre à un agenda politique. La première contrainte, c'est le rejet de la présence française, notamment avec le revirement de l'opinion publique, ces mêmes citoyens qui avait applaudi l'intervention dans les rues de Bamako, Tombouctou et Daho et partout dans le pays en 2013 manifestent aujourd'hui pour le départ des Français, c'est là le fruit d'une savante stratégie d'influence diligentée par Moscou qui franchit une ligne de plus avec l'arrivée de la société Wagner. Ensuite, une contrainte diplomatique quant aux relations avec le pouvoir central de Bamako. Le dialogue ne pouvait qu'être rompue tôt ou tard avec cette junte qui privatise le pouvoir après l'expulsion de notre ambassadeur, une humiliation pour la France, la junte exige désormais le départ immédiat des troupes internationales un retrait précipitées, désordonnées représenter une faille dans laquelle son engouffreraient des terroristes, qui souhaitent porter des coups à nos forces, nous appelons à la plus grande vigilance sur la garantie totale de la sécurité de tous les personnels, je salue ce que vous avez dit hier, monsieur le 1er ministre à l'Assemblée nationale concernant ce retrait, qui serait, qui ne seraient pas imposés dans le temps et que la sécurité de nos troupes seraient bien sûr préservé et puis enfin une triple contrainte tactique politique et sécuritaire avec l'arrivée de la milice Wagner après s'être déployée partout en Afrique, dans un axe nord-sud de la Libye au Mozambique, la Russie se déploie en Afrique de l'Ouest. L'afflux massif d'éléments russe est un risque supplémentaire et Direct, comment mener des opérations sur zone avec la présence de ces fous de guerre dans le secteur, nous ne pouvons pas prendre le risque d'être assimilés à ces gens qui font commerce de la violence et des exactions nos forces armées porte haut les valeurs de la démocratie et de la lutte implacable contre le djihadisme avec le départ des forces européennes, ce sont les Maliennes et les Maliens qui se trouve sous la menace d'hors de, de Wagner, l'histoire est déjà écrite, quand la junte n'aura plus la trésorerie, les hommes de Wagner se payeront directement sur la bête, comme en République centrafricaine, le pillage deviendra la norme, malheureusement après la terreur jihadiste la population paiera le prix du sang et des larmes, tout cela, pourquoi des officiers de la junte sont des rentiers, sans considération pour le devenir, ni du Mali, ni du peuple malien, le pouvoir a été volé à la démocratie par la force, le nouveau pouvoir et maintenu par la force un pouvoir qui ne sert qu'un petit nombre dans le seul objectif est de s'enrichir un pouvoir qu'ils ne redistribuent rien aux citoyens dans cette affaire, ce qui restera, ce n'est pas tant la décision de partir, ni celle d'y être allé ce qui restera, c'est l'instabilité et le manque d'anticipation, quelle a été la stratégie de la France au Mali et au Sahel depuis ces 5 dernières années. Et vos fameuses Lignes Rouges posée par votre gouvernement depuis 2017, force est de constater que si elles ont existé ces lignes rouges n'auront eu de cesse de battre en retraite, ses lignes rouges apparaissent désormais comme autant de vaines tentatives de et de coup de poker à l'attention de Bamako et de Moscou. Des expérimentations diplomatique qui n'ont pas fonctionné, l'annonce du départ n'est pas un choix stratégique, mais une décision contrainte. Autant par la succession des événements au Mali que par l'impossibilité pour nos partenaires européens de poursuivre cette présence, le gouvernement s'est retrouvé dos au mur, le débat prévu en mai au Bundestag sur le mandat encadrant leur déploiement des troupes allemandes le le terme du mandat de la Minusma en juin prochain le nom le nouvellement d'ores et déjà décidé de l'engagement des troupes suédoises ou belge au sein de Takuba tous ces éléments ont formalisé la véritable ligne rouge, pas celle que l'on se fixe dans le cadre ou d'une stratégie claire mais celle que les aveux des événements nous impose. Or, gouverner, c'est prévoir la prise de décision du président de la République est imposé sous la pression, dès lors, nous pouvons relier toutes les sorties diplomatique que la France depuis 2017 sur la question du Sahel et même de l'Afrique à travers ce prisme, le sommet de Pau, des réunions et des autres chefs d'État, la publicité d'un président de la République, chef des armées, tout cela n'aura eu aucune prise sur le déroulé de l'histoire. En matière de politique étrangère, nous ne sommes pas loin d'observer que le président de la République n'aura procédé à des gesticulations après avoir tenu la main de pour 2018, il a enchaîné le dialogue des dialogues stériles avec ce président et avec Poutine au Liban l'initiative française n'a débouché sur rien une grande partie de l'opinion et les médias libanais, considère que le président de la République n'aura pas apporté de solution est, somme toute, accentué les difficultés. Et puis il y a eu toute la stratégie de la France dans la zone indo-Pacifique tomber en une annonce avec le retrait de l'Australie, de la vente des sous-marins français sur ce sujet, nous considérons que de nombreuses interrogations demeurent entières tous les accusations du président de la République et du gouvernement se sera heurtée à l'épreuve des faits, la crise en Ukraine, on sera hélas. Une de plus, même s'il faut chercher la paix jusqu'au bout, la politique étrangère n'est pas une simple affaire de communication politique consistant à créer un besoin par un nouveau coup d'éclat : la politique étrangère ne peut pas se résumer. à quelques envolées sans lendemain en matière de relations internationales, il n'y a pas de formule magique, il y a de la méthode de l'exactitude et de l'assiduité, ce qui fait le rayonnement de la France, ce sont la stabilité des valeurs qu'elle défend le sérieux de ses engagements, sa faculté à pouvoir plus loin comme on dira qu'en 2003. à la fin de ce quinquennat la France quitte le Mali par la petite porte, et le gouvernement tente d'esquisser le travail. Essentiel d'introspection et d'améliorations dont notre pays a besoin quant à sa politique internationale, on nous explique que tout va bien et que rien ne change vraiment puisque Barkhane continuera à partir des pays limitrophes, conséquence la France demeureraient clairvoyant, tout seul, mais des questions concrètes restent sans réponse, entre autres choses, cuite par exemple du survol de l'espace aérien malien pour protéger la Minusma et porter des coups aux bandes de terroristes Barkhane n'est qu'un exemple des nombreuses autres embarras du gouvernement actuel en matière de politique étrangère, alors que la compétition internationale s'est très fortement accrue que les superpuissances se réarme et pose inéluctablement le risque de la guerre. C'est toute notre politique étrangère que nous devons interroger de la formation aux métiers de notre diplomatie à notre réseau consulaire de l'aide au développement à la francophonie, des grandes orientations de notre stratégie dans le monde à notre place dans l'Europe, la France doit se redéfinir, pour être en capacité de faire face aux enjeux tels qu'ils se présentent, c'est le prix de notre amélioration collective, c'est le socle de notre nécessaire l'unité et continuité républicaine quant aux questions d'affaires étrangères et de défense, je vous remercie. Merci mon cher collègue, la parole est maintenant notre collègue Olivier Cigolotti pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le président, Monsieur le 1er ministre. Madame et messieurs les ministres, mes chers collègues. Je souhaite tout d'abord saluer l'initiative du gouvernement qui a demandé l'inscription de cette déclaration suivie d'un débat à l'ordre du jour de notre assemblée. Compte tenu des annonces faites par le président de la République la semaine dernière il s'avérait indispensable d'évoquer aujourd'hui l'avenir de l'intervention française au Sahel. Je tiens au nom de mon groupe à rendre hommage à nos soldats engagés dans cette zone à tous les régiments qui se sont succédé durant toutes ces années, mais aussi aux 59 militaires qui ont perdu la vie dans le cas des opérations Serval, puis Barkhane. Nos pensées vont à leur famille, à leurs proches à leur faire d'armes. La France est engagée au Mali depuis 2013. 9 ans après, force est de constater que ni l'opération militaire française, ni l'aide internationale n'ont permis d'engager le pays dans la voie de l'apaisement. Le pays et de façon récurrente, dévastée par les violences et une anomie politique. La décolonisation a créé le Mali sur les bases de l'ancien Soudan français regroupant des populations n'ayant historiquement que peu de relations et depuis 1960 l'instabilité politique aussi entre multipartisme et coup d'État militaire à favoriser une situation chaotique que même la constitution pourtant d'inspiration française en 1992 n'a pas pu apaiser. Les accords pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger de 2015 donc que très peu été mise en oeuvre, aucun des 5 piliers sur lesquels se fonde ces accords n'a été appliquée de façon satisfaisante. 3 phénomènes destructeurs de la cohésion sociale marquée aujourd'hui le Mali les violences armées, la corruption des autorités en place la progression des groupes jihadistes. Un fossé s'est accentué entre la position de la France qui souhaite éradiquer le djihadisme et les autorités locales qui souhaitent entrer en négociation avec certaines composantes. Ainsi la volonté de constituer une armée malienne nationale semble vouée à l'échec tant les divergences entre le Nord et le Sud sont prégnantes. Le Mali n'est prêt ni à un état très centralisé, il y a un éclatement comme aurait pu le laisser supposer les accords d'Alger. Dans ces conditions, comment vouloir imposer le retour de l'État et de façon sous-entendu de la démocratie. Il convient de rappeler que la crise malienne a une origine protéiforme. La rébellion touareg, précipitée par la chute du régime libyen, la multiplication des groupes armés terroristes et les nombreux conflits communautaires au centre et au nord. C'est dans un climat très lourd début 2020, que le président Emmanuel Macron a réuni ses homologues israélien pour un sommet à Pau. Même si certains ont critiqué la méthode : c'est à cette occasion que l'État islamique au Grand Sahara a été désigné comme ennemi prioritaire, c'est également à cette occasion que les États de la région réaffirmer collectivement leur souhait de voir la France les épauler dans la lutte contre le terrorisme. Les coups d'État de 2020 et 2021 ont généré des complications supplémentaires, le Conseil national de transition a remis en cause les avancées acquises précédemment allant jusqu'à repousser à une échéance lointaine, le processus de transition démocratique. Une ligne rouge a été franchie en fin d'année, avec l'arrivée des membres des groupes paramilitaires russes. Ainsi le désengagement des forces françaises initiée à l'Automne dernier a constitué un 1er niveau de réponse face à cette situation. Car la junte militaire au pouvoir, n'en est pas à une provocation près, remise en cause des accords de défense, remise en cause de la présence danoise au sein de la force Takuba interdiction de survol du territoire malien par les appareils opérant au profit de l'opération Barkhane. Toutes les nations contributrices à la force Barkhane ont de plus en plus de mal à faire entendre aux dirigeants sahéliens la nécessité pour ces derniers de mieux gouverner de mieux réformer les forces de sécurité. Avec le coup d'État au Burkina Faso, dans la zone, intervention de Barkhane seul le Niger conserve une gouvernance légitime, certes, nous ne pouvons plus demeurer dans son pays où nous ne sommes plus les bienvenus et ou de profonds désaccords entre la France et le Mali subsistent sur les modalités de règlement de la crise. Une succession d'événements dans cette région du Sahel, a contribué à la montée du sentiment anti-français et a fini par rendre impossible le maintien de la force Barkhane au Mali. Cependant, une question demeure sans réponse : à quel moment et pour quelle raison une force militaire de protection se transforme-t-elle soudain dans l'imaginaire local en force d'occupation. L'officialisation jeudi dernier du retrait militaire du Mali, par la France et ses partenaires européens me paraît être l'option la plus sûre pour nos soldats, d'une part, mais également la plus adaptée pour poursuivre notre engagement au Sahel et étendre notre soutien aux pays voisins du Golfe de Guinée et d'Afrique de l'Ouest. Alors que les groupes terroristes veulent métastasé, l'ensemble de la région et se rapprocher des poumons économiques que représentent Abidjan et Dakar. Notre mobilisation reste indispensable dans cette zone. En restant donner bien entendu avec les États voisins et tout particulièrement avec le Niger, dans le respect de leurs procédures constitutionnelles. En effet, le Niger allemande du G5 Sahel le plus susceptible de figurer au coeur du redéploiement du dispositif militaire de lutte contre le terrorisme. Certes, ce principe est acté. Cependant, le rapprochement avec la France et ses partenaires nécessite un travail de pédagogie auprès de l'opinion, mais aussi une validation démocratique de la part des citoyens nigériens. C'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères a annoncé que dès le mois prochain, le 1er ministre nigérien allait engager la responsabilité de son gouvernement sur cette question sensible par un vote devant l'Assemblée nationale du pays. Reste également en suspens un certain nombre de questions. Tout d'abord l'articulation et la restructuration de nos dispositifs militaires avec les autorités du Niger, mais aussi avec celle des autres pays de la sous-région, pouvez-vous, Madame, messieurs les Ministres nous éclairer sur ce point. Concernant notre départ du Mali, le président de la République a déclaré que la fermeture concrète des base française de Gao Ménaka et Gossi prendrait entre 4 et 6 mois, cette manoeuvre, il devrait être rapide et très sécurisé face au potentiel attaques des groupes armés terroristes. Mais elle sera également complexe en s'inscrivant dans le cadre d'un processus coordonné avec les partenaires africains, européens et dans un contexte de saison des pluies à partir de mai qui ne facilitera pas ces mouvements. Par ailleurs, quel avenir pour Takuba. La taskforce répondait à des besoins spécifiques des militaires maliens cet engagement unique valait pour ce pays, il faudra donc une phase de redéfinition afin de savoir si les pays contributeurs seront prêtes à poursuivent leur mission au profit de nouveaux partenaires. Enfin, je pense également aux enjeux liés à l'EUTM Mali et à EUCAP Sahel, ainsi qu'à la présence de la Minusma au Mali. Dans lesquels plusieurs pays européens sont engagés ces dispositifs devront nécessairement être revu et adapté un contexte nouveau. La situation actuelle impose un questionnement auquel il faut nous confronter avec réalisme, la France a-t-elle les moyens de rester le seul leader de la lutte contre le jihadisme. à l'heure de la présidence de la France de l'Union européenne, nous devons insuffler un débat majeur sur la possibilité d'un partenariat européen durable pour lutter contre le terrorisme, bien au delà de Takuba. Dans le même temps, il est désormais urgent d'agir diplomatiquement dans les pays de la sous-région pour favoriser le retour à une transition démocratique, redonnant de la légitimité aux représentants issus de ces éventuelles élections. Même si Barkhane est une addition de succès tactique qui abouti pour certains à un échec stratégique et diplomatique quitter le Mali ne veut pas dire pour autant abandonner la lutte contre le terrorisme, quitter le Mali ne signifie pas renoncer à la sécurité de la France et de l'Europe. Merci mon cher collègue. Donner la parole à notre collègue Alain Richard pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants, vous avez la parole. la parole. Président. Monsieur le 1er Ministre Mesdames et messieurs les Ministres, chers collègues mes premières son pamphlet dans ce débat, vont à nos soldats, des femmes et des hommes d'exception. Engagé dans la bande sahélo-saharienne leur combativité et leur abnégation mérite notre respect. Je veux leur témoigner au nom de mes collègues notre soutien résolu notre fierté et notre reconnaissance profonde à nos 59 soldats morts au Sahel pour la France défendra la liberté et notre sécurité ainsi qu'à leurs familles, je rends l'hommage déférent qu'il aurait dû leur mémoire restera intact, la nation n'oubliera jamais leur sacrifice nous pensons aussi avec affection avec le à leurs frères d'armes blessée. Leur action n'a pas été vaine, ils n'ont pas été vaincus. Sans le lancement de l'opération Serval en 2013, à la demande du président Traoré à l'époque sur la contre-offensive réussie de nos unités, la stratégie d'occupation territoriale l'implantation des jihadistes auraient réussi et l'État malien, ce serait très probablement effondrée sans Serval le Mali serait devenu un puzzle de territoire failli sans aucune cohésion étatique au contraire le processus démocratique avait alors pu reprendre tandis que les régions du nord ont été libérés, je sais que la progression des djihadistes vers le sud, a été stoppée, la France, par la suite, il n'a jamais mais ménagé ses efforts pour mobiliser ses partenaires européens et internationaux, aux côtés de nos militaires de Barkhane et avec succès, pour contrer la stratégie d'expansion et de déstabilisation régionale de groupes armés terroristes au Sahel, aux frontières de l'Europe, d'une certaine façon, et je ne fait qu'évoquer les multiples résultats tactique positif les résultats, les succès militaires obtenu au long de cet engagement. Au cours de ces 9 années notre action commune et la direction de nos autorités a permis d'aboutir à un cadre international solidaire et fiable pour répondre à ce défi, ce cadre à Pau n'est pas uniquement militaire, il porte aussi sur le soutien au déploiement de l'État, les administrations territoriales et des services de base et sur la reconquête par les États de la région du contrôle de leur propre territoire. Cela a abouti à l'Alliance Sahel qui reste un acquis solides mais dans le cas du Mali les multiples épisodes de formation ou de reformation de bandes armées prétendant combattre au nom de l'Islam et terrorisant la population ont été aussi l'effet de défaillances répétées des autorités en place devant les échecs de développement de la sous scolarisation facilitant de propagande primitive et du discrédit lié à la corruption. Plus largement, que les gouvernements, c'est un ensemble de milieu responsables, les dirigeants du Mali, où il faut mentionner les autorités religieuses qui n'ont pas mobilisé leurs énergies pour rétablir le dialogue et organisé, force du développement, la persistance des attaques terroristes et la récréation de ces mouvements ne pouvait pas être surmontée par les seules armées alliées devant de surcroît des forces maliennes souvent au-dessous de leur mission. Dans ce contexte, entendre aujourd'hui les autorités de fait malienne, dire que la France aurait failli à son engagement envers leur pays, mais tout simplement intolérables, irrespectueux envers nos soldats et relève de la manipulation la plus médiocre. Prenons le pouvoir à la suite de 2 putschs successifs, la junte militaire malienne est revenu sur son engagement, d'organiser des élections à brève échéance elle ne plus de non plus désormais aucune perspective crédible de transition civile avant 2025 et je ne parle même pas de la mise en oeuvre de l'accord de paix entre forces somaliennes signée à Alger qui ne progresse plus, qui, pire encore, et quasiment jeté aux oubliettes notre décision de quitter le Mali a été prise après la multiplication par cette junte de déclarations une action hostile à notre égard, après avoir tout fait pour entraver notre action militaire pourtant confié par un gouvernement malien lui légale. C'est ainsi que nous avons été empêché le survoler l'espace aérien et que notre ambassadeur a été contraint de quitter le territoire en urgence, nous ne pouvons donc approuver pleinement le président de la République quand il dit que nous ne pouvons pas rester engagé militairement aux côtés d'autorité le fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés, nous prenons acte avec responsabilité du choix malien de c'est de s'écarter de tous ces hommes ses partenaires constructifs, la junte s'est enfermé dans une logique d'isolement de provocation et le confrontation à l'encontre de la CEDEAO, ainsi que le ses autres partenaires africains et internationaux ce pouvoir de fait c'est aussi éloignés des intérêts et de la sécurité de sa propre population, d'autant plus qu'il a fait maintenant le choix de la société privée russe Wagner, en effet, comment ne pas condamner cette décision de préféré utiliser le peu de son public disponible pour rétribuer les mains des mercenaires russes plutôt que de financer le déploiement de services publics au bénéfice du peuple malien ou encore de lutter contre la dégradation de la situation humanitaire et là c'est de la sécurité alimentaire. Nous connaissons le mode opératoire déstabilisateur de Wagner, il passe par le recrutement et l'envoi d'agents militaires privées d'une zone de conflit, a une autre, par l'intimidation de la population civile. Des violations répétées du droit international humanitaire l'alimentation de la violence et l'instabilité ainsi que par l'apparition de société de concessions et l'exploitation des ressources naturelles du pays, tout simplement pour les payer, ce n'est pas une spéculation ce que je dis, c'est ce qu'endure aujourd'hui la population civile centrafricaine, c'est aussi ce qui s'est vérifié en Libye, en Syrie et dans donc dans le dans les Maliens sont donc les premières victimes de cette situation de plus l'expérience en Centrafrique, observant l'impact des exactions de ces militaires contre la Minusca. Ne peut que nous préoccuper, s'agissant de la Minusma au Mali, ce d'autant qu'une fois le redéploiement hors du Mali terminé, il n'y aura plus de soutien aérien français immédiat pour aider la Minusma en cas de difficulté. C'est dans ces conditions que l'Union européenne a décidé de sanction le 13 le 13 décembre dernier et nous devons les soutenir, je crois que c'est évident, personne n'est dupe, nous connaissons l'application de la Russie dans la fourniture d'armes et de soutien matériel à Wagner au Mali comme ailleurs le finiront pas de croire que la Russie n'a aucun agenda géopolitiques au Sahel, nous ne sommes pas non plus dupe des activités de propagande et une manipulation de l'information. Certaines sont conduites par des États tels la Russie, la Chine et la Turquie, à des fins politiques, d'autre part, les autorités maliennes elles-mêmes pour détourner les critiques et les frustrations des Maliens, ces activités ont certainement alimenter injustement le sentiment anti-français dans divers secteurs de la société malienne, nous ne savons la guerre de l'information fait rage, c'est au Sahel et il est à regretter que nous n'ayons que trop peu réussi à contrer ces attaques monsieur le 1er ministre c'est là une priorité importante, donnons-nous à l'avenir les moyens de mener efficacement cette contre-offensive de la l'information, notamment en mobilisant l'audiovisuel extérieur. réalité, la réarticulation notre engagement militaire au Sahel étaient nécessaires, il avait été actée dès le sommet de N'Djamena, puis précisé en juin dernier par le président attend le passage d'une logique d'opérations extérieures à un dispositif de coopération accrue mieux adaptée face à une modeste menace qui s'est diffusé le tout en suivant, comme vous l'avez expliqué expliquer monsieur le 1er ministre l'esprit de Takuba cette nouvelle logique partenariale de l'autre. Si on sera déterminante pour nous adapter aux évolutions des groupes armés terroristes en Afrique de l'Ouest et à la propagation vers les pays du Golfe de Guinée, le Niger et le Tchad seront des partenaires opérationnels essentiel, ils ont démontré leur solidité politique, de même, en plus du G5 l'initiative d'Accra autour du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, Togo et Bénin deviendra une base de mobilisation efficace, je veux en concluant saluer la volonté de mettre davantage les populations civiles au coeur de notre stratégie de lutte contre les groupes terroristes, de les sortir de leur classe de la victime pour en faire un 1er rempart contre ces groupes, c'est, c'est c'est ce qui a été votre expression, Monsieur le 1er ministre ce sursaut civil ne doit pas être vu rituel. Il est impératif pour nous de réussir son accompagnement en déployant des programmes civils et sociaux répondant aux besoins locaux, nous restons aux côtés du peuple malien et nous maintenons l'espoir que notre politique de développement renouvelé sera y contribuer utilement c'est dans cet esprit de résistance que nous approuvons les choix cohérent offensive et solidaire du président, que le gouvernement nous a présentés avec clarté, je vous remercie. Si parole au président, Pierre Laurent, pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Monsieur Monsieur le président, Monsieur le 1er Ministre Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. La dramatique situation au Mali et le bilan désastreux de l'intervention militaire française ont des causes profondes et non conjoncturel. C'est à mes yeux par là qu'il faut commencer pour en tirer des leçons. Les États de la zone sahélienne font partie des nombreux États du sud qui ont été depuis longtemps affaibli saigner et désarmé par l'ajustement structurel libéral. Les armées africaines sont faibles, certes, mais parce qu'elles ont subi les mêmes logiques de délitement que toute la société et leurs états et cela dans les domaines économiques, fiscales, sanitaires alimentaires éducatives judiciaires et sécuritaires, la violence endémique à prospérer dans les plaies de cette crise multidimensionnelle c'est la toile de fond de toute la crise sécuritaire depuis 10 ans. Il y a un an, j'ai, au nom de mon groupe pointé l'impasse de l'opération Barkhane 42ème expéditions militaires françaises en Afrique depuis les indépendances qu'avions-nous dit à l'époque. Je me permets une citation la situation humaine, politique et économique du Mali empire dans ce contexte de déstabilisation sociale et politique, les islamistes continuent de développer leur sinistre entreprise les leçons des guerres menées au nom de la guerre contre le terrorisme ne sont pas tirées à chaque fois, les pays sont laissés en proie au chaos pour des décennies, la désintégration de la Libye en est un exemple à l'est d'ailleurs directement à l'origine d'une partie des violences armées dans le nord du Mali, dans quel état laisserons-nous le Mali et les autres pays de la région si nous poursuivons dans cette voie, fin de citation. Nous avons poursuivi. Mais je rappelle que ce constat a été dressé plusieurs mois avant la venue au pouvoir du colonel Goïta et à la venue du de Wagner au Mali, c'est dire que les responsabilités politiques françaises dans le désastre actuel ne peuvent pas être car ce désastre était prévisible, les cartes de France Diplomatie mettent aujourd'hui en en rouge, près de 90 % du territoire malien contre 10 % il y a 10 ans, voilà le résultat de la militarisation à tout va les victoires tactiques contre les jihadistes que vous n'avez cessé d'invoquer pour justifier la poursuite de Barkhane non, en vérité jamais tari le terreau de recrutement des entrepreneurs de violence en 2021 près de 2000 événements violents ont été recensés au Sahel en augmentation constante depuis 2015, provoquant la mort de plus de 4800 personnes pour cette sol année la violence des groupes jihadistes contre civils représentent 60 % de ces violences, une part non négligeable et donc également imputables aux forces de sécurité et de défense, dont celle de l'armée française à titre d'exemple, je veux rappeler le bombardement français au Mali de Bounty. Qui avait fait 19 morts civils, et plus récemment les 20 et 27 novembre 2021, les morts et les blessés graves de manifestations au Niger et au Burkina Faso, contre le passage d'un convoi militaire français. Cette guerre a évidemment aussi coûté la vie à 59 de nos militaires dont nous saluons évidemment la mémoire mais la lumière sur l'ensemble de ces violences n'est pas encore fait, et elle devra l'être aujourd'hui notre armée va quitter le Mali mais allons-nous véritablement changer de paradigme, comme l'a déclaré Emmanuel Macron rien ne l'indique, au contraire, puisque nous voulons nous redéployer au Sahel, avec les mêmes objectifs en forçant la main, semble-t-il, cette fois au Niger pour nous y installer, pour quel résultat demain les mêmes très probablement dans ce contexte dans lequel l'image de la France s'est fortement dégradée, les tirs les tirer les ficelles de régime d'États africains fragilisés, avec des prises d'opposition à géométrie variable, selon qu'il s'agit du Tchad de la Côte d'Ivoire, de la Guinée du du Mali ou du Burkina Faso, nous appuyons dans ce cas d'les sanctions de la CEDEAO contrôle Mali sanction extrêmement dur et qui punissent plop un peuple malien en souffrance, mais aussi par ricochet les populations des pays limitrophes et les diasporas, notamment en France, alors que faire, nous demandions il y a un an, un plan de retrait programmé concerté, vous nous avez pas écouté aujourd'hui acculé, vous niez l'évidence de l'échec, nous le demandions pourtant pour y substituer un nouvel agenda politique, économique et de sécurité durable pour le Mali et la région enfin tourné vers un développement de l'Afrique par les Africains nous avons depuis 10 ans dépensé 30 fois plus pour intervenir militairement que pour financer l'aide au développement 28 millions d'APD en 2021 au Mali pour près de 900 millions pour Barkhane. L'APD absolument nécessaire, ne suffira d'ailleurs pas, même si elle est augmentée et mieux, c'est la refondation de notre relation à l'Afrique, qui doit être à l'ordre du jour et qu'on ne nous dise pas que la Françafrique, c'est fini, ou alors qu'on m'explique pourquoi nous avons l'an dernier, précipité le ravalement de façade du franc CFA en éco sont même que les parlements africains n'a été réellement concerter pour couper l'herbe sous le pied à tout projet de construction d'une souveraineté monétaire africaine qu'on m'explique aussi ce que faisait le 24 janvier dernier Nicolas Sarkozy et Yannick Bolloré dans le bureau de sa chère ami de la France, Alassane Ouattara, si ce n'est pour le convainc d'avaler la couleuvre de la vente des concessions portuaires d'Afrique de l'Ouest du groupe Bolloré au géant italien MSC alors même que la fin de ces concessions pourraient pourraient conduire à la reprise en main souveraine de ses infrastructures stratégiques oui il faut décidément changé d'époque, mais surtout arrêter de le dire et le faire vraiment dans le domaine sécuritaire notre appui militaire au terme d'un, au terme d'accord renégocié avec les pays concernés doit être recentrée sur le soutien exclusif aux armées locales ont retenons si ces pays le souhaite la formule d'un comité d'État-Major conjoint des forces africaines, formation et transfert de technologie aux armées nationales doivent être programmées pour rompre avec une une dépendance quasi exclusive avec l'ancienne puissance coloniale, le retrait des troupes françaises doit être concertée avec les pays de la zone Sahel, l'unité du Mali doit être garanti et les accords d'Alger renégocier, comme nous le proposons dans la campagne présidentielle démilitariser les relations internationales est une urgence, nous le voyons en Europe, en Afrique et ailleurs inspirons-nous pour l'Afrique de la feuille de route de Lusaka, faire taire les armes en Afrique, luttons contre les trafics d'armes, cessons de vente des armes à des États du Golfe qui entretiennent des relations troubles avec les mouvements jihadistes surtout refont dont nos relations économiques et je veux terminer en rappelons quelques-unes de nos propositions à ce sujet, il faut avancer urgemment vers la suppression des paradis fiscaux Offshore qui permet un accès rapide aux richesses illégalement acquises et Servent le pillage du continent africain, les flux financiers illégaux participent chaque année à la fuite de près de 1000 milliards de dollars du continent dans cette logique, nous réaffirmons que 10 % de l'aide publique au développement pourrait être dédiée au soutien au renforcement des systèmes fiscaux des pays en développement, deuxièmement, aider à la construction d'une souveraineté monétaire africaine sans laquelle tout financement du développement est structurellement handicapée la tutelle du franc CFA et doit être, et la France doit agir en vue de changer les critères d'allocations des droits de de tirages spéciaux du FMI et agir en faveur d'une réaffectation des DTS non utilisés, notre groupe a déposé une résolution en ce sens, enfin il faut réviser la logique actuelle des échanges économiques et des traités de libre-échange qui maintiennent ces pays dans une économie extravertie, contre toute logique de développement de l'en sources humaine et économique endogène et les empêche d'affronter les immenses défis du développement humain et de la lutte contre le réchauffement climatique pour le siècle à venir, l'intérêt commun de la France, du Mali, des pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest et la reconquête des moyens de développement propres par ces pays toute autre voix empreinte d'instrumentalisation au service d'influence exclusive dans la guerre d'influence des puissances est vouée à l'échec, ces 10 dernières années, nous le montre avec éclat, je vous remercie. Donner la parole à notre collègue André Guillaume pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. mes chers collègues, depuis quelques mois, la relation entre Paris et Bamako, tenez, de plus en plus à la chronique d'une mort annoncée, jeudi dernier, la décision du désengagement des troupes françaises au Mali est en effet l'aboutissement de l'engrenage en offrant plus d'autres alternatives comment sommes Mouloud arrivé là. Sur la trajectoire dite de rupture pour, comme l'a qualifié le président de la République, c'est certain, l'installation au pouvoir de la junte du colonel Goïta en mai dernier, puis celle de Maïga à la tête du gouvernement ont marqué un tournant dans les relations entre les 2 pays. Nous devons cependant nous interroger sur tous les ressorts qui ont poussé à mettre en cause la présence française au Mali, il nous appartient de tirer les enseignements de cette situation, tout d'abord par respect pour les 59 morts dont 53 soldats français morts pour la France et pour les nombreux blessés, ça a été dit, qui nous écoutent probablement cet après-midi et qui ont payé un lourd tribut à l'affaiblissement des troupes djihadistes, ils ont contribué, grâce à leur courage, à leur engagement éviter bon nombre d'attentats sur notre territoire en effet depuis 9 ans, plusieurs grands chefs islamistes et leurs petites mains ont été éliminés, dont l'émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et tué en juin 2020. Avant cela, en 2013, n'oublions pas la première réussite de nos soldats dans le cadre ou de l'intervention Serval, l'arrêt de la progression des terroristes, la préservation de l'État malien et le maintien de l'intégrité des terrils territoriale du Mali, conformément à la mission que leur avait confiés à l'époque, le président Hollande cependant gagné la guerre ne fait pas gagner la paix en l'espèce il a il a 5 doute manqué la capitalisation politique et par Bamako des gains militaires sur le terrain, la reconquête des territoires n'a pas été suivie d'une politique de service auprès des populations, par conséquent, dans certaines zones rurales, les Maliens sont plus enclins à laisser s'installer les organisations terroristes. Dans ces conditions, la première leçon consiste à savoir si nos opérations extérieures peuvent s'éterniser car nous sommes face à un État qui restent indéfiniment failli en outre notre présence militaire sur le terrain doit être accompagné par une action humanitaire menée conjointement avec ces États ne faudrait il pas systématiquement conditionner le maintien des forces françaises à un projet de reconquête institutionnel local établi par le pouvoir en place nos propres soldats ont aussi besoin de cet objectif-là pour comprendre le sens de leur mission, lorsque c'est le sud-est dure près d'une décennie, la seconde interrogation : doit-on rester coûte que coûte l'acceptabilité des populations locales n'est plus au rendez-vous, la France a une équation toujours compliqué lorsqu'elles interviennent dans des pays qui garde mauvais souvenir du temps colonial on allie on a vous savez, depuis quelques années, comme il y a la colère grandissait à l'encontre de la présence militaire française, pourtant en 2013 à la France, il y avait été appelé directement par Bamako, Paris était avait obtenu le soutien de l'Union européenne ainsi que par l'ONU, cependant, sur la durée, il est difficile pour notre pays de ne pas être assimilé à son ancienne image de puissance coloniale lorsqu'elle est instrumentalisée, à la fois par les autorités maliennes et par Wagner et ces que News une dans une partie de l'Afrique, il devient évident que la France a tout intérêt à se fondre au sein d'une force multilatérale s'agissant du Mali, on ne peut pas nier que cela était éteinte et entre Minusma le G5 Sahel et la force Takuba mais le conditionnement de Barkhane décidèrent à Pau, conjugués à la lenteur de la montée en charge, les forces spéciales européennes a laissé la France en première ligne ces réflexions invite à méditer sur l'idée d'une défense européenne qui ne soit pas, qui ne doit pas se limiter à des manoeuvres ou à des alliances industrielles en matière d'armement il faut franchi un cap plus conséquent sur le plan opérationnel, car c'est toute la sécurité et de l'Europe qui se joue au Mali, c'est un dossier par la présidence française de l'Union européenne, certes, un dossier de plus monsieur le 1er ministre sur le plan diplomatique. Quels autres le sommes pouvons-nous tirer de l'expérience malienne, il en est une, assez sensible qui consiste à savoir si dans certaines configurations, nous ne devrions pas lutter contre les tabous qui sont les nôtres, mais un forcé et forcément pas ceux des populations concernées lorsqu'un pouvoir incluse décide la mise en place d'un dialogue inclusif à l'espèce comme on à Al Qaïda quelle position adopter la France est prisonnière du terrorisme qui a fait trop de nombreuses victimes sur notre sol mais sommes-nous incapacité de poser les conditions dans les territoires aussi complexe à le président Keïta voulez également de négocier avec les 2 principaux chefs malien affilié à Al-Qaïda dans les indépendantistes touareg apparaissait comme leur 1er ennemi Léo pour Senghor disait ce que veulent les esprits distingué qui soit de l'Ouest ou de l'Est, c'est nous imposer une civilisation européenne nous en imprégnant sous la couleur de l'universel, à certains égards, cela peut faire au sens, enfin il me reste à évoquer le 3ème des de la politique de développement, une véritable urgence pour le Mali qui est au 100 84ème rang de l'échelle, défini par le PNUD comment l'Agence Française de Développement va-t-elle pouvoir assurer la continuité de ses projets dans un environnement sécuritaire plus qu'incertaine, certes, le retrait de Barkhane au Mali ne signifie pas l'abandon du Sahel, le gouvernement l'a rappelé,

avec l'Algérie, tapi dans l'ombre ou pour reprendre le dossier malien, mais avec qui, nos relations sont fluctuantes quant aux ensembles régionaux de la CEDEAO ou de l'Union africaine, les seules sanctions économiques ne saurait suffire, nous le constatons que dans un monde en permanence un mouvement un client des intérêts divergents, à des modèles sociétaux éloigné à des religions instrumentaliser peuplé d'hommes et de femmes baignant soit dans l'abondance, soit dans la pauvreté, les conflits sont potentiellement de partout et ce n'est pas la situation en Ukraine qui me démentira, quelles sont les leçons que nous devons en tirer d'abord que seule la recherche du bonheur de chaque individu sur cette planète semble universelle, nous aurons ainsi appris que la réponse militaire, aussi nécessaire soit-elle, doit être accompagné par un engagement sur le terrain pour éduquer les populations, développer les territoires concernés et lutter contre la pauvreté, si nous ne voulons pas être rejeté, rejeté par ceux-là mêmes qui nous avez réclamé le rêve. Je ne suis pas sûr que ceux qui sont censés nous remplacer plus animée de convoitise des richesses naturelles face au mieux que nous sur le pour le bonheur du peuple malien, ni pour l'éradication du terrorisme, le rendez-vous est pris pour terminer, la France est intervenue pour défendre légitimement ses intérêts sécuritaires et pour répondre à l'appel d'un pays menacé par le terrorisme, une campagne de dénigrement lâché contre elle avec les moyens modernes de communication vient vérifier si le vieil adage politique l'important n'est pas ce qui est vrai, mais ce qui est cru, c'est aussi une leçon que nous devons tirer je vous remercie. Je vais maintenant appeler le président Claude Malhuret pour le groupe, les indépendants républiques et territoires. Vous avez la parole monsieur le président. Monsieur le Président, Madame et messieurs les ministres, mes chers collègues, malgré la distance qui les sépare les événements du Mali et d'Ukraine ont un point commun. Ils sont une étape dans la dissipation d'une grandiose et merveilleuse illusion. Le temps dévoile les lignes de force de l'histoire, il nous enseigne que le 17ème siècles fut celui des monarchies absolues et de l'ordre westphalien. Le 18ème, celui des Lumières et de l'avènement des démocraties, le 19ème celui de la révolution industrielle et de la domination du monde par l'Occident. Le 20ème siècle fut celui du combat à mort des démocraties contre les totalitarismes, par 2 fois, les premières ont failli le perdre le 9 novembre 89, la chute du mur de Berlin signer leur victoire l'illusion fut de la croire définitive, 12 ans plus tard, en 2001 7 12 illusions s'est effondré en même temps que les tours jumelles de Manhattan. Et chaque année qui passe apporte un nouveau démenti à ceux qui croiraient encore. Lorsque Samuel une Huntington a publié en 96, le choc des civilisations dans l'euphorie de la victoire des démocraties, il fut loin de convaincre : en 30 ans plus tard, l'histoire nous montre qu'il était visionnaire, les conflits idéologiques de la guerre froide ont disparu, remplacées par les lignes de fracture entre civilisations, c'est le retour des religions, des nationalismes, des zones d'influence et de l'affaiblissement de l'universalisme au profit des particularismes, mauvaise nouvelle pour nous, car à la perte nette prépondérance s'ajoute le fait que nous sommes les seuls ou presque qui se revendiquent de la démocratie dans un océan de régimes illibéraux dictatoriaux religieux, militaire ou totalitaire. Le Mali en est un bon exemple où nous affrontons la conjonction du djihadisme islamiste de soudards anachronique prétendant lutter contre le colonialisme, 60 ans après l'indépendance de la Chine sur le plan économique et de la Russie sur le plan militaire et politique. Certains demandent de quand date nos difficultés au Mali, la réponse est simple du début. Ce que je dis là peut surprendre tant Serval fut un succès. Mais Serval n'était pas le début. Le début et nous y sommes un peu pour quelque chose, c'est que, en 2011 lors de notre guerre humanitaire en Libye étrange oxymore inventé par des éditorialistes enivré de la démocratie, victorieuse et des ONG, appelant à l'aide sur le terrain après avoir stoppé les colonnes de chars de Kadhafi chargeant sur Benghazi, nous nous sommes détournées, laissant s'aggraver la guerre civile, les affrontements des tribus, la disparition des frontières, l'explosion des groupes jihadistes dans tout le Sahel boosté par les trafics d'armes, d'argent, d'être s'humains et de drogue, voilà pourquoi succédant à Serval victorieux Barkhane n'a jamais eu que 2 issues possibles : ne jamais finir ou finir un jour par le départ sans victoire définitive. du des pays du Sahel, c'est que lorsque la démocratie est défaillante, la place est libre pour les 2 solutions les pires l'extrémisme religieux et les Centurions. Le djihadisme a menace désormais jusqu'au Golfe de Guinée et les coups d'État se multiplient. C'est ce qu'a très bien compris le dictateur paranoïaque de Moscou qui n'a aucun projet positif au Mali, ni ailleurs, et dont le seul but est d'en chasser les autres en installant à Bamako un quarteron de colonels formé à Moscou. Et en dépêchant après le Mozambique et la Centrafrique, les mercenaires de Wagner, de triste mémoire. Et c'est là que l'Ukraine fait écho au Mali. L'incarnation du ressentiment, l'homme qui s'est juré de revenir par la ruse ou par la force sur le rabougrissement de son empire son cauchemar, c'est que l'Ukraine marche vers la démocratie et qu'elle réussisse. Parce que l'exemple serait contagieux chez lui. 50 1000 soldats massés à la frontière et déjà entrés en Ukraine et il se présente comme l'agressé. Ce qui est effarant, c'est que certains ici même le crois. Dans leur combat contre les dictatures, les démocraties ont un énorme handicap, elles ont en leur sein une 5ème colonne les populistes d'extrême droite et d'extrême gauche qui ont un flair infaillible pour renifler les despotes de Le Pen à Mélenchon en passant par Zemmour c'est acquis gagnera le concours du Meilleur caniches. N'importe quelle personne saine d'esprit ne peut qu'être effaré par l'invraisemblable litanie des violations du droit international par la Russie, invasion de la Géorgie, soutien aux sécession de l'Ossétie de la brasier de la Transnistrie Crime contre l'humanité en Tchétchénie et en Syrie, annexion de la Crimée soulèvement du Donbass, pression sur la Moldavie et les pays baltes dénonciation maladive de l'OTAN cyberattaque massive chasse aux ONG d'instruction du Boeing de la Malaisie Airlines assassinat manqué de Navalny exil forcé pour Khodorkovski Kasparov assassinat réussi de Politkovskaïa de Lutvinenko de Markelov de Bourbon va de Magnus ski de Berezovski de même sauf et de bien d'autres, et aujourd'hui l'invasion. Mais les populistes continue de brailler, que les responsables sont les Américains. L'anti-américanisme rance de la vieille extrême droite anti-anglo-saxonne et de la vieille extrême gauche anticapitaliste la vieille rancune comment pardonner aux Américains de nous avoir sauvé 3 fois au XXe siècles pour ces tyranneaux file tout aussi responsables, ce sont les dirigeants européens, cette Europe qu'il déteste et qui veulent abattre cette Europe qui propose à ses partenaires, tout ce que Poutine comme eux-mêmes ne peut supporter la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et la solidarité entre les États membres. Il rabâche au auprès la propagande de l'ex-colonel du KGB la nation ukrainienne n'existe pas, l'Ukraine fait partie de la sphère de la Russie, la Russie a été humilié depuis la chute du mur, aucun mot bien sûr de l'humiliation pendant 5 décennies des Polonais, des Tchèques, de Hongrois et de toutes les autres victimes de l'occupation soviétique, à commencer par les Ukrainiens. Depuis 3 jours, c'est encore plus écoeurant il s'aplatir devant Poutine et pilonne Macron il ne parle que de souveraineté, mais ils réclament la soumission de l'Ukraine. Que les extrêmes tiennent ces discours de collabo et dans l'ordre des choses, ce qui est affligeant, c'est qu'ils détiennent sur une droite républicaine dont une partie est déjà Zemmour au Poutine et une autre si complaisante avec Poutine, qu'elle me donne, quand je l'écoute, l'impression d'entendre et le toc toc du parapluie de Daladier sur les pavés de Münich. Comme j'aimerais entendre enfin l'un de ses membres poser cette question. Qui imagine le général De Gaulle, entré au conseil d'administration d'oligarques russes complice de Poutine et corrompue jusqu'à la moelle. Si j'évoque Münich c'est qu'en 1938 les nazis expliqué que la nation autrichienne n'existait pas comme Poutine explique que la nation ukrainienne est une fiction, il disait vouloir défendent les minorités allemandes dans les Sudètes comme Poutine prétendent défendre les Russes ethniques du Donbass, il est plus que temps de se souvenir de cette phrase de Karl Marx, ceux qui oublient l'histoire sont condamnés à la revivre et nous sommes aujourd'hui en train de la revue. Pour en revenir au Mali, je pourrais donner à mon tour mon avis sur la façon de partir de nous redéployer au Sahel d'organiser en urgence la protection de nos alliés du Golfe de Guinée où les sont déjà l'. Le 1er ministre l'a fait avant moi et qu'il me suffise de dire que je partage son analyse. Mais je ne peux terminer sans un hommage particulier à nos soldats qui se battent depuis 10 ans dans des conditions dantesques et par une pensée pour les 59 d'entre eux qui sont morts au combat, certains prétendent qu'ils sont morts pour rien, ce qui est ignoble, ne serait-ce que parce que depuis 10 ans. Ils nous ont protégés en empêchant l'installation au Mali d'un califat islamiste d'où seraient irrémédiablement planifié des attentats en Europe et, enfin, ils sont le symbole et le guide de ce dont nous risquons tous d'avoir énormément besoin dans les temps qui s'annonce au Sahel, comme en Europe, le courage. La parole est maintenant. Président Guillaume Gontard pour le groupe écologiste solidarité et territoires. Je le président, vous avez la parole. Merci, le Monsieur, le président Monsieur le 1er ministre madame la ministre, messieurs les ministres, à quoi bon débattre quelles conséquences nos discussions aura sur la politique du gouvernement, un débat parlementaire, c'est bien, mais un débat avant l'annonce des décisions, c'est mieux et un débat avec vote avant l'annonce des décisions, c'est une démocratie qui fonctionne, ce n'est pas sur la politique étrangère et militaire de la France, pas plus qu'ailleurs, que le gouvernement se sera illustré par une considération marqué et une vraie prise en compte du Parlement lors de ce quinquennat comme d'habitude, toutes et tous, nous avons dû attendent patiemment la parole présidentielle. Ce n'est guère une surprise, un seul vote de la représentation nationale est intervenu pour autoriser l'intervention militaire au Mali de 2013, un seul vote pour plus de 9 années d'engagement, une période durant laquelle le périmètre d'intervention s'est agrandi et les orientations stratégiques ont évolué, mais jamais le Parlement ne s'est prononcée formellement toujours la prise de décision s'est trouvée confinée au palais de l'Élysée, l'image d'une telle pratique n'en est plus que saisissante en comparaison de ce qui se passe chez nos voisins européens oui donner sa place au Parlement prend du temps, mais ce n'est que bien peu de temps face à la durée, pour laquelle les décisions prises auront des conséquences le retrait des forces armées françaises du territoire malien nous y souscrivons la situation politique au Mali est devenue à soupe tables et tu ne permet plus un engagement militaire viable entre le refus par la junte au pouvoir, d'organiser des élections, des manifestations anti-françaises, empêchant des convois militaires, la présence de 800 hommes de la société privée militaire Wagner ça été rappelé les conditions opérationnelles pour nos soldats ne sont plus garantis je tiens à exprimer avec le groupe Écologie Solidarité et territoires mais pensées pour les 59 militaires morts au Sahel depuis 2013, leurs familles, leurs proches ainsi qu'aux nombreux blessés nous souscrivons à la décision de retrait, mais elle ne rend pas la suite de la politique française au Sahel plus aisée, un retrait même des questions et des défis pour les prochains mois, vous l'avez évoqué monsieur le 1er ministre d'abord sur la mise en 9 concrète et pratique comment opérer la fermeture des bases de Ménaka Gauci et Gao alors que plus de la présence française diminuera et plus nos soldats seront vulnérables à des attaques alors que des protestations anti-françaises pourraient bloquer les opérations et alors surtout que les relations avec la junte au pouvoir qui exige un retrait immédiat de nos troupes sont de plus en plus difficile sur Calais de nos partenaires, pouvons-nous compter dans cette logistique d'ampleur avec des délais aussi courts, il y a aussi des questions plus stratégiques posée par notre retrait du Mali des questions quant à l'avenir des missions multilatéral de la Minusma et ses 13000 casques bleus et l'EUTM comment assurer la protection de ses personnels qui est jusque là garantis par les forces armées françaises au Mali, au-delà de ces problèmes immédiats, des questions de fond se posent auxquelles il faudra répondent pour qu'il y a les leçons soient tirées de l'échec de notre intervention au Mali et qu'un vrai bilan soit fait de ces 9 dernières années, car il faut avoir l'honnêteté et l'Intelligence de le dire, des erreurs ont été commises, c'est bien ce qui manque cruellement dans les prises de parole gouvernementale des derniers jours. Présenté le retrait du Mali comme le résultat de l'arrivée de la junte au pouvoir et du facteur Wagner, c'est occulter d'abord les raisons qui ont rendu possible les de coups d'État et ne pas établir une analyse pertinente de la situation sahélienne, c'est ignorer les travers de nos relations à certains États sahéliens où il faut le dire, nous avons soutenu pendant des décennies, les dirigeants autoritaires dont les politiques pouvaient difficilement mener à une stabilité régionale à long terme, c'est ignorer la faiblesse des perspectives politiques de la sortie de crise et nier la verticalité des méthodes qui ont sous-entendu notre coopération dont l'exemple le plus frappant fut la convocation sommaire de nos partenaires à Pau il y a 2 ans. Si le gouvernement refuse de prendre en compte ces critiques alors c'est prendre le risque de l'impasse politique et militaire du Mali se répète, là où les forces armées françaises seront redéployés, la volonté d'élargissement de l'intervention militaire à des partenaires européens au sein de la tax force Takuba n'a pas connu non plus un enthousiasme débordant, quand bien même le gouvernement n'a eu cesse de la présenter comme un succès homme étant évidemment de préciser les chiffres des forces engagées. La situation sur le plan politique n'est pas meilleure en un an, 3 pays où intervient la France ont été l'objet de coup d'État militaire, ces événements rendent la coopération militaire multilatérale ardue, notamment pour le G5 Sahel dans lesquels la France placés de l'espoir, enfin on ne peut balayer d'un revers de main les protestations anti-françaises, bien qu'elle soit instrumentalisée par d'autres puissances cette instrumentalisation s'appuie sur une défiance prises existantes, alimentée par un manque de transparence sur les opérations militaires françaises, c'est particulièrement le cas concernant les frappes abouti en janvier 2021 et ont causé la mort de 19 civils selon la mission des Nations unies, là où il y a le soupçon s'installe la méfiance Tero du rejet si les dernières décennies d'intervention militaire à travers le monde nous ont bien appris une chose, c'est qu'on ne peut intervenir dans un être un dans un autre pays contre sa population. Les écologistes ont toujours dit : aucune solution militaire ne peut advenir sans solution politique, nous n'avons cessé de regretter le manque de prise en compte des contextes ultra-locaux et des problématiques communautaires dans la conduite stratégique des opérations de même, il aurait fallu dépasser enfin le tabou des discussions avec certains groupes armés qui porte des demandes profondément politique les refuser, comme interlocuteur revenait tout bonnement à enterrer une perspective de sortie de crise qu'aucune solution militaire ne peut advenir sans solution politique, ce sont les besoins des populations qui doivent être placés au centre de la stratégie française ce sursaut civil qui n'a pas eu lieu après son annonce au sommet de N Djamena doit arriver rapidement. Parce que qu'une solution militaire ne peut advenir sans solution politique, l'aide publique au développement, en direction des pays du Sahel doit être plus conséquent et mieux ciblée pour répondre aux besoins réels des populations locales, l'aide humanitaire doit aussi d'être augmenté 2 5 millions de personnes ont dû quitter leur foyer et 15 millions de sahéliens vivent de l'aide humanitaire aujourd'hui les besoins humanitaires ne sont assurés qu'à 48 % selon les ONG, quand en 2020 880 millions d'euros sont consacrés à l'intervention militaire, seulement 28 millions sont pourvus pour l'aide humanitaire, c'est cette balance qu'il faut rééquilibrer à l'avenir, parce qu'aucune solution militaire ne peut advenir sans solution politique la présidence française du Conseil de l'Union européenne doit être l'occasion d'élaborer un grand traité entre l'Union européenne et l'Union africaine, non à un texte de libre-échange qui ouvrent l'apport des pays africains à la prédation des multinationales européennes mais un texte de coopération sur un sujet essentiel, tels que l'eau, la sécurité alimentaire, le climat ou le numérique déployons une stratégie globale alliant militaire diplomatie et développement, sinon la réorientation de la présence de la France au Sahel ne sera qu'un nouvel enlisement pour la prochaine décennie. merci Monsieur le Président. La parole est à monsieur Christian Cambon, président de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées. Madame la présidente, monsieur le 1er ministre Madame Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce débat était bien utile et les interventions des orateurs des groupes ont été très riche, et je les en remercie, il démontre amplement l'utilité de débattre ici au sein du Parlement, il y a un an ici même nous débattions justement de la poursuite de l'opération Barkhane nous étions déjà préoccupé par l'extension du terrorisme au Burkina Faso et par le 1er coup d'État au Mali, pour autant, il nous restait quelques raisons d'espérer succès militaire contre les groupes terroristes, montée en puissance de Takuba renforcement du G5 Sahel ces tendances destinée alors un avenir possible pour Barkhane un an plus tard, la réalité et bien d'autres, les provocations constantes de la junte de Bamako nous on tous indignés d'autant plus en insupportable que 53 de nos militaires ont fait le sacrifice de leur vie et à mon tour, à cet instant, je m'incline devant leur mémoire et c'est une pensée douloureuse pour leurs familles et pour leurs compagnons et je tiens, du reste, à chaque fois que l'un des leur revient pour un dernier voyage aux invalides à y être présent au nom de notre commission. Ensuite, comment serait-il matériellement possible de poursuive Barkhane alors que la junte a remis en cause nos propres accords militaires comment mener des opérations au sein d'une OPE d'une population abreuvés par la propagande anti- française, dès lors, la décision du président de la République de quitter le Mali était nécessaire, elles étaient de bon sens. Mais ne revenions pas pour autant ce que nous avons fait au Mali, au contraire, au contraire, nous pouvons être fiers de l'action de nos militaires nous avons agi conformément à nos valeurs en nous souciant aussi du sort des populations sahéliennes elles-mêmes si férocement ciblée par les djihadistes. En vérité, cette situation confirme l'analyse que le Sénat ne cesse de développer. L'enjeu du développement revêtent une dimension essentielle dans la stabilisation du Sahel dans ce domaine, encore, la France a répondu présent, le Sénat s'est toujours engagé pour que les moyens soient à la hauteur des enjeux, peu à peu les montants ont suivi, rappelons que sur les 5 dernières années, le Sahel a reçu de notre part 2 milliards 200 millions Nous souhaitons encore plus de rapidité, plus d'efficacité dans nos axes dans nos actions visant à nourrir à former et à soigner les populations lorsqu'elles sont sécurisées, la pauvreté est en effet le terreau qui nourrit l'extrémisme. Sur le plan strictement militaire Barkhane nous aura permis de progresser sur le fond, sur le front de la défense européenne, nous avons pu convaincre et c'est un de vos succès, nous avons pu convaincre plusieurs de nos partenaires européens de nous rejoindre dans Takuba de partager notre engagement est d'accroître significativement notre capacité d'agir en commun, développant ainsi une culture stratégique commune à l'heure où tant de tensions se manifestent dans notre continent, voilà qui est une bonne chose, après Barkhane nous devons donc tenir compte de ses acquis alors à présent, quels sont les enjeux qui justifie une poursuite de notre engagement dans la région, tout d'abord, il faut bien sûr endiguer l'extension de la menace terroriste vers le Golfe de Guinée, des attaques ont lieu en Côte d'Ivoire au Bénin une autre zone des trois frontières et susceptible de devenir un foyer terroriste à la jonction du Bénin, du Niger et du Burkina Faso. Les États, ils sont quasiment est dramatiquement absent et les filières terroristes, ils sont déjà installés, pouvant se connecter avec d'autres organisations terroristes au nord du Nigeria. La stabilité des États du Golfe de Guinée est essentiel, c'est là que se trouvent les grands gisements de croissance et d'emploi, c'est là qu'une partie des sahéliens choisit chaque année d'émigrer, notre destin est donc lié à cette région, l'évolution inquiétante que nous constatons peut sans doute encore être inversée par une action civile et militaire vigoureuse éclairée par les succès mais aussi par les enseignements et les déconvenues de Barkhane. D'autre part, nous ne pouvons rester sans réaction face à certaines puissances qui étendent leurs zones d'influence déjà en République centrafricaine, l'installation du groupe Wagner, avec son cortège d'exactions, de mise en coupe réglée des ressources et de violentes campagnes anti-tout ceci nous avait déjà alertés aujourd'hui malheureusement le Mali prend le même chemin, pourtant ce que fait la Russie en Centrafrique, au Mali, n'a rien à voir avec ce qui a fait la France alors que nous mobilisons notre armée pour combattre les terroristes et que l'Agence Française de Développement investi des centaines de millions les mercenaires du groupe Wagner eux Servent de garde prétorienne un pouvoir déliquescent et se payent sur l'exploitation des richesses de ce malheureux pays sans aucune retombée pour les populations. Alors maintenant, monsieur le 1er ministre Madame Monsieur le Ministre qu'allons-nous faire. Tirer les leçons du passé, voilà qui est nécessaire et faisons de bons choix pour l'avenir, c'est sans doute plus important encore, il nous paraît en effet important de prendre du recul, la précipitation risque de nous replonger dans les mêmes difficultés dans les mêmes pièges fatals à Barkhane ce qui doit guider nos choix, c'est bien une nouvelle idée du rôle que la France peut jouer dans une, dans la région, voir en Afrique toute entière, ce n'est pas un simple repas le replâtrage dont nous avons besoin, mais une réflexion sur la nouvelle stratégie de la France en Afrique, si l'on cela ne marchera pas, ainsi ce redéploiement dont on parle ne doit pas ressembler à une simple translation de Barkhane au Niger : certes, le Tchad est loin à l'Est et le Burkina Faso, sort d'un coup d'État, donc nos options sont limitées, il n'y a-t-il pas un immense risque, tout se passe au Niger comme il vient de se passer au Mali, les campagnes d'opinion anti-françaises il y a déjà commencé, je rappelle que le président nigérien Bazoum a essuyé une tentative de coup d'État, 2 jours seulement avant son investiture et si vous ne vous assurez pas d'avoir le soutien sans faille de ce pays et des autres vous positionnerait notre armée vous leur ferait peut-être un cadeau empoisonné, il faudra aussi assurer la sécurité de notre de nos militaires pendant cette phase de transfert, c'est une opération, nous le savons très complexe à haut risque et qui doit être planifiée avec le plus grand soin, or la junte malienne nous met sous pression, il faut qu'elle sache que nous prendrons le temps d'assurer la sécurité de nos soldats, par ailleurs, vous envisagez pour la suite, un déploiement d'implantations plus petites, moins visibles, un soutien à géométrie variable à base de formation ou de conseillers militaires ou peut-être d'intervention à la demande, là encore, réfléchissons bien, car même si, bien entendu, ce n'est pas votre attention cela pourrait fortement ressembler à un interventionniste que nous avons souhaité abandonner il y a quelques années déjà dans nos relations avec le continent et il faudra bien l'expliquer, en outre, une telle stratégie permettrait-elle de concentrer des moyens suffisants pour être efficace, Farago face aux groupes terroristes, rien n'est moins certain à cause des distances et donc des opérations dans la nature va changer, qu'en sera-t-il du soutien de nos alliés dans cette nouvelle configuration après la fin de Takuba avez-vous déjà obtenu des assurances des uns ou des autres, vous nous le direz dans vos réponses, au-delà de l'action de la France et de ses partenaires, nous avons ainsi des interrogations sur les intentions et les capacités des acteurs de la région, ainsi, est ce que le le G5 Sahel peut se relever des récents coups d'État, les armées locales seront-elles toujours soutenu par la communauté internationale et qu'en sera-t-il notamment. De l'EUTM, organismes de formation financée par plusieurs, plusieurs pays, notamment européens, et qui est si importante pour que les armées africaines soient à la hauteur, par ailleurs, le président algérien a déclaré il y a quelques jours que la relation franco-algérienne, je cite, prenait une nouvelle tournure allez-vous Monsieur le Ministre, saisir cette occasion d'impliquer davantage l'Algérie dans une stabilisation de la région. Monsieur le 1er Ministre Madame Monsieur le Ministre, vous le voyez, nos interrogations, nos doutes, disons-le, sont encore nombreux, nous souhaitons en tous les cas que le Parlement soit régulièrement informée et de manière transparente sur l'évolution de notre dispositif, le travail entre l'autorisation du Sénat en 2013 et le débat sur Barkhane, que nous avons obtenu il y a un an 8 années s'étaient écoulées sans que le Parlement ne ne débattent spécifiquement de ce point et ça va, c'est à votre honneur Monsieur le 1er ministre d'avoir organisé de débats, souhaitons que nous restions sur cette tendance car c'est véritablement important de pouvoir sans échanger avec le Parlement, c'est une condition du contrôle démocratique et plus largement du soutien de l'ensemble de nos compatriotes à notre stratégie de lutte contre le terrorisme, alors Monsieur le 1er Ministre Madame Monsieur le Ministre, c'est donc un combat nouveau qui commence, mobilisant un engagement sans faille de nos armées, mais aussi une agilité plus forte de l'aide au développement, vous le savez, nous le savons tous, c'est à ce prix que la France se trouvera son influence et contribuera efficacement à son combat pour la paix, je vois. Merci La parole est à Madame Florence Parly ministre désarmer. Je laisse oui. Monsieur le président de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées, mesdames et messieurs les sénateurs, comme l'a clairement expliqué le 1er ministre de profonds bouleversements politiques et sécuritaires en Afrique de l'Ouest. Donc aucun. Au Sahel et tout particulièrement au Mali ont conduit le président de la République à prendre la décision d'entamer une nouvelle étape dans la transformation de l'opération Barkhane avant de répondre à vos questions, j'aimerais avant tout me joindre à vous pensez et rendre hommage aux 59 militaires qui sont morts au Sahel depuis le début de l'opération Serval en 2013. Je veux aussi rendre hommage à ceux qui ont été blessés dans leur Chair et dans leur esprit, en combattant farouchement le terrorisme. Leur sacrifice n'ont pas été vains. De même que l'engagement tout aussi exemplaire des 125000 soldats français qui se sont succédé, année après année au Mali n'a pas été vains nos militaires ont fait un travail extraordinaire, ils se sont relayés pendant 9 ans, depuis 2013 au Mali pour lutter contre le terrorisme et sans leur professionnalisme sans leur détermination et leur ardeur au combat le Mali aurait peut-être connu le destin qui fut celui de l'Irak et de la Syrie à partir de 2014 lorsqu'au fil de ses conquêtes territoriales Daech bâtissait un sanctuaire du terrorisme islamiste. Aujourd'hui le Mali n'est pas un sanctuaire terroriste. La situation depuis 2013 en effet beaucoup évolué. à commencer par la situation politique au Mali, car le pays est désormais dirigé par une junte militaire qui a rompu tous ses engagements. Et la conséquence directe des choix effectués par cette junte c'est que les conditions de notre engagement ne sont plus réunies, nous avons donc en pleine concertation vient insiste avec nos partenaires européens et sahéliens pris la décision de quitter le Mali. Cette décision, acte un état de fait, nous ne pouvons pas continuer un combat militaire aux côtés d'une junte qui a clairement signifié sa volonté de rupture avec les partenaires régionaux, la CEDEAO avec les partenaires européens et notamment la France. Nous quittons donc le Mali mais nous disons les choses franchement. Nous aurions pu y rester plus longtemps si les circonstances avaient été différentes. Car il faut bien réaliser que pendant ce temps, les seuls bénéficiaires de ces turpitudes politiques, ce sont les groupes terroristes eux-mêmes. Nous en avons conscience et c'est pourquoi nous allons continuer de lutter contre le terrorisme dans la région, mais avec des moyens plus légers, plus Agile. Nous allons continuer cette lutte avec nos partenaires européens et africains dans le cadre d'une stratégie collective adaptée aux évolutions de la menace et nous prendrons évidemment en compte le fait que le terrorisme s'étend de façon dangereuse vers l'Afrique de l'Ouest et nous allons donc en conséquence intensifier notre coopération de défense avec les pays du Golfe de Guinée, complétera sur quelques-unes des questions que vous avez posées au cours de ce débat, pourquoi partons-nous du Mali pour comprendre pourquoi nous partons il faut naturellement se souvenir des raisons pour lesquelles nous y sommes allés depuis 2013, c'est à la demande des États de la région que les armées françaises sont présentes au Sahel et pendant 9 ans l'État malien, au même titre que ses voisins, a réclamé soutenu et favoriser la présence militaire française sur son sol pour lutter contre le terrorisme, mais au cours de ces 9 années, la méthode a évolué. Pour autant, les résultats ont toujours été là parce que nos militaires ont été à la hauteur, mais aussi parce que le gouvernement malien rendait leur mission possible. Ces missions étaient doubles affaiblir les groupes terroristes et accompagner la montée en puissance des forces armées maliennes, or depuis quelques mois. Les autorités maliennes, il faudrait plutôt mieux dire la junte. A fait le choix de la rupture diplomatique et de la provocation politique. Dans ces conditions, nous ne sommes plus en mesure de conduire nos missions de façon satisfaisante en ne respectant pas le calendrier électoral et en faisant appel aux mercenaires de Wagner, la junte a fait le choix d'un modèle et de valeurs qui ne sont pas les nôtres. En expulsant du Mali, les représentants de la CEDEAO en renvoyant les forces spéciales danoises en expulsant l'ambassadeur de France et en installant pardon en insultant publiquement les membres du gouvernement français, elle a rejeté notre appui et choisit l'isolement. Aujourd'hui cette junte entrave l'action de nos forces sur le terrain, les conditions politiques et opérationnels ne sont donc plus réunies pour rester il y va d'une question de cohérence. Nous ne quittons pas le Mali à cause. Du développement d'un sentiment anti-français, certains d'entre vous ont mentionné cette question tout d'abord je voudrais vous dire que ce phénomène est tout de même difficilement mesurable. Il est d'autant plus difficilement mesurable, que c'est une vision qui est déformé par la loupe des réseaux sociaux dont les analyses elles-mêmes ne sont pas épargnés par les phénomènes de manipulation car nos compétiteurs ont en effet tout intérêt à donner l'impression que ce sentiment. Est désormais présent partout, ce que je peux vous dire, c'est que Barkhane partout où elle a été déployé, a toujours été bien accueillie par les populations locales avec lesquelles nos militaires entretiennent des Liens quotidiens. En conséquence, si nous partons cette uniquement. à cause de la rupture du cadre politique imposée par la junte malienne. Alors ce départ. Est-ce un constat d'échec. d'échec. Nous avons neutralisé les principaux chefs des groupes terroristes, nous avons désorganiser leur structure nous avons détruit leur ancrage territorial, nous ne les avons obligé à fuir et à se cacher. Où en serait le Mali, ainsi que les pays de la région, si nous n'avions pas fait ce travail. S'il y a échec c'est celui de la junte, qui n'a pas la volonté politique de mener avec détermination la lutte contre les groupes armés terroristes et qui n'a pas obtenu de résultats sur le plan politique, car souvenez-vous en, il n'y a eu aucune avancée sur l'accord de paix et de réconciliation alors je l'ai dit, nos objectifs, ils étaient militaire contre les groupes terroristes contrer notamment l'action de leur chef, le 1er ministre a détaillé les succès que nous avions remporté aussi bien vis-à-vis des chefs d'Al-Qaïda que des chefs de Daech notre autre objectif c'était la formation des armées sahéliennes, car oui, nous avons formé des milliers de militaires sahéliens, nous les avons entraîné, nous avons accompagné sur le terrain et nous avons combattu à leurs côtés. En 2013 c'est exact les les forces armées maliennes étaient très peu formés très mal entraînée sous- équipés et insuffisamment encadrées. L'armée de terre comporter 7000 hommes dotées d'équipements obsolètes, l'armée de l'air 1000 hommes avec des moyens aériens inadaptée. L'armée malienne et forte de 40000 hommes. Et nous avons grandement contribué à la former l'entraîner et l'équipe cette armée est bien plus forte, et elle a montré sur le terrain qu'elle était capable de faire face aux groupes armés terroristes, ce qui est une très grande réussite alors vous le savez, rien n'est définitivement acquis. Mais nous avons placé les groupes terroristes, apporter des armées maliennes et il appartiendra au Mali d'entretenir seul. Enfin, et je ne détaillerai pas, parce que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, le fera, nous avons permis le retour de l'État malien à certains endroits et nous avons fondamentalement revu. Notre aide au développement. Alors ce n'est pas parce que on se quitte en mauvais termes. Qu'il n'y a rien n'à en retenir et que ceux qui osent parler d'échec, regarde les résultats de l'opération Barkhane que ceux qui osent parler d'échec, regarde l'état du Mali en 2013 et que ceux qui osent parler d'échec m'explique comment, nous, nous aurions dû faire pour atteindre une victoire totale car on entend toujours beaucoup de commentateurs qui explique ce que nous aurions dû faire mais je veux simplement vous redire très simplement ce que nous avons fait. Nous avons redonné espoir à une population qui vit sous la terreur terroriste nous avons traité directement et avec courage une menace très dangereuse et nous assumons aujourd'hui nos actes et notre décision, nous ne pouvons pas rester au Mali, alors nous partons. La France et notamment les soldats français ont littéralement empêcher qu'un sanctuaire terroriste ne se forme au Mali. Alors bien sûr, il faut s'adapter, il faut s'adapter à l'évolution de la menace et une opération militaire, ce n'est pas une décision gravé dans le marbre Serval Barkhane ces 2 opérations se sont sans cesse adapter et elles se sont adaptées en fonction d'une menace terroriste qui se propage et qui descend vers le sud. Et nous répondons à cette évolution dans le domaine militaire, l'idée est de se réarticuler pour prendre en compte cette nouvelle géographie de la menace, nous réduisons par ailleurs notre empreinte pour aller vers une présence plus diffuse, plus intégrée avec les forces armées avec lesquels nous coopérons. Alors quant à Takuba takuba, va elle aussi évoluer, mais l'esprit de Takuba va perdurer et c'est d'ailleurs ce que nos partenaires européens souhaitent et si certains ici ont pu considérer que Takuba finalement était peu de chose, je voudrais rappeler que ce que nous avons réussi à faire en 2 ans. C'est ce que l'on attendait de l'Europe de la défense depuis 50 ans, nous avons monté une que la coalition européenne avec 10 États militairement capables et politiquement volontaires une coalition entre Européens, avec des soldats d'élite européens qui sont allés au combat face à des groupes terroristes et les résultats de Takuba sont significatifs, ils ont largement dépassé les attentes initiales alors peut-on parler de l'illusion que serait à Cuba. Je ne suggère pas d'utiliser cette expression vis-à-vis de ceux qui ont mené une opération qui a permis la neutralisation d'une trentaine de jihadistes entre le 1er et le 6 février dans le Liptako malien, cette opération a été menée par les forces spéciales de Takuba et les forces armées maliennes qu'elles accompagnent donc je crois que Takuba ah non seulement rempli son objectif opérationnel, mais que si Takuba quitte le Mali, hé bien, ce départ ne signe pas la fin de cette force d'ailleurs le 17 février le président Bazoum s'est dit prêt à accueillir un dispositif européen comparables sur le territoire nigérien car il estime que les capacités des forces spéciales européennes répondent à la menace des groupes armés terroristes et j'en suis, pour ma part, la première des échanges auront donc lieu ces prochains jours avec nos partenaires à ce sujet. Je voudrais maintenant. Répondre à une question qui, à vrai dire, ne suscitent pas un grand suspense. Est ce que la lutte contre le terrorisme s'arrête aujourd'hui. évidemment non, nous allons poursuivre avec nos partenaires africains et nos alliés européens notre engagement, je l'ai dit, c'est la près la forme de notre présence qui évolue parce qu'elle dépend de la volonté des États de la région parce qu'elles s'adaptent à la réalité de la menace donc nos opérations continues. Est ce que Wagner et la cause de notre départ, j'ai dit. La réponse est non. Wagner n'est pas la cause notre départ la cause, c'est la rupture provoquée par la junte malienne mais Wagner et le symptôme de la volonté de la junte de se maintenir à tout prix au pouvoir et de s'isoler de la communauté internationale et ce sont ces choix-là qui nous pose problème. Alors je ne sais pas s'il est utile de rappeler quel est le modèle avec des guillemets, au terme, modèle de Wagner puisque Wagner cette déjà déployés dans un certain nombre de pays, ce que l'on peut en dire, c'est que c'est un système qui est fondé sur la violence sur les exactions des populations civiles sur la prédation des ressources des États et que ce système loin de diversifier les partenariats du Mali, va conduire à isoler, celui-ci, pour terminer, je voudrais répondre à une question que beaucoup ont opposé cet après-midi, en ce qui concerne Barkhane et les éventuels contacts, d'une part avec Wagner et d'autre part, les conditions du désengagement de Barkhane au Mali, je voudrais vous dire que nous évite, nous prenons toutes les mesures pour assurer la sécurisation de ce désengagement. Nous nous préparons, évidemment, au pire, c'est d'ailleurs la mission des militaires de toujours se préparer au pire et nous continuons évidemment de suivre activement le déploiement de Wagner sur le terrain et nous sommes en train de travailler aux conditions de notre désengagement mais ce que je peux vous dire, c'est que nous nous tenons prêts à réagir avec la plus grande fermeté en cas de menace sur la force Barkhane et je veux être très clair devant vous : nous ne tolérerons aucune provocation et aucune entrave durant notre redéploiement. Madame la présidente, monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, avant de céder la parole au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et alors que les travaux du Parlement seront bientôt suspendu, je tenais à vous remercier pour la qualité des débats que nous avons vu ici au Sénat au cours de ces 5 dernières années. Qu'il s'agisse de l'examen plus de l'adoption de la loi de programmation militaire des débats de contrôle en séance publique, ou bien encore de nos échanges en commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées. La défense nationale, la protection des Français sont autant d'enjeux qui dépassent largement les clivages partisans, autant d'enjeux aussi qui nous rassemble tous. Monsieur le président, quand bon j'ai pleinement conscience que l'information transparente et régulière des parlementaires participent à la compréhension de l'action du gouvernement par l'ensemble des Français et je me tiendrai nous nous tiendrons naturellement à votre disposition, comme nous l'avons toujours fait pour continuer de vous rendre compte, merci. Merci, Madame la Ministre. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

Madame la présidente. Monsieur le président Combo mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs. Quelques mots pour. Terminer ce débat d'abord en en me réjouissant de la qualité des interventions qui ont été faites. de leur rigueur et de leur côté non polémique par rapport à un enjeu qui est considérable pour nous-mêmes et pour les pays d'Afrique. Je voudrais aussi vous faire part d'une certaine émotion personnelle. j'étais ministre de la Défense compte. Le président Hollande a pris la décision courageuse, je crois, d'engager les forces françaises au Mali. J'ai même présidé. Aux obsèques du chef de bataillon Damien Boiteux premier dès le 1er jour de l'intervention. Je me souviens avoir initié dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur de France, une stèle où se sont égrenées s'graines toujours les noms des 59 morts. Pour la France et pour le Mali et pour notre sécurité. Et j'avoue avoir à la fois la tristesse. Parfois de la colère. Kant, je vois la non reconnaissance. De ces actions de ce soutien. Par des autorités qui se sont imposés par la force au Mali. Quand je vois nos propres forces traité des de force d'occupation, voire de mercenaires. Par ceux-là mêmes qui dont les prédécesseurs ont appelé au secours la France à un moment particulier dramatique et qui a cette présence française a permis d'éviter que le Mali ne devienne un État djihadistes. Donc, je voulais vous dire ça à à ce moment précis, au moment où nous nous avons pris une décision de réarticulation de dispositifs qui passe par l'abandon de nos positions initiales au Mali. Dans dans le débat qui vient d'avoir lieu. Il y a 3 points majeurs que je voudrais souligner, sans revenir sur surtout des interventions. Mais qui n'apparaissent utiles pour contribuer à éclairer la la situation. S'il y a un échec, je reviens sur l'intervention du président Retailleau. D'abord, on lui en lui rappelant peut-être un point mais dans le détail de de l'agenda, c'est toujours un peu difficile de s'y retrouver mais le le le Search Et le sursaut civils ces Djamena. Ces 2 étapes différentes, même si elles sont à articuler pour bien garder le calendrier c'est janvier 2020 et N'Djamena 6 février 2021 et la décision de réduction c'est juin 2021 et là maintenant, la décision de reconfiguration pour garder le calendrier. Mais si on revient en arrière. Au-delà de ces aspects militaires et des aspects d'adaptation sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Il y a, à mon avis, un sujet dont on ne parle plus jamais. Et qui est pourtant l'essentiel et s'il y a un échec. C'est celui-là : l'échec, ce sont les accords d'Alger. Parce que Monsieur Gontard, il y a une solution politique. Elle a été initiée en 2015. Avec l'ensemble des acteurs qui ont signé des papiers. Qui, qui prévoyait d'abord la réintégration des groupes que l'on appelle les groupes armés signataires dans les forces maliennes. Qui prévoyait une décentralisation, une mise en valeur de des capacités du nord du pays, tout cela sous l'initiative de la diplomatie algérienne, les accords d'Alger avec la validation des Nations unies adoptée acceptée par le Conseil de sécurité, avec le soutien de l'Union africaine, il y a une solution politique est sur la table et une des questions que nous devons nous poser, c'est comment se fait-il que ces accords d'Alger solution politique qui suivait le début de l'opération Serval ne soient restées lettre morte et contrairement au procès que j'ai entendu tout à l'heure par certains, c'est peut-être là qu'il faut chercher les responsabilités de ceux qui n'ont pas voulu mettre en oeuvre, accord d'Alger et aujourd'hui, le sujet reste vacant si on aboutit à cette évolution, c'est bien parce que il n'y a pas eu la volonté de mettre en dehors des accords et ce n'est pas, je le dis au président Combo, je ne crois pas que ce soit un refus de la diplomatie algérienne de vouloir à vous faire avancer les affaires il y a une telle inertie qu'à mon avis, tout le monde a abandonné. j'ai participé à des réunions régulières ou on vous disait on va maintenant plus accord d'Alger, mais rien n'a bougé, je pense que s'il a des gens qu'on n'en parle pas assez, il est bien là, à identifier et sans doute à identifier les responsables et je dis que les responsables politiques maliens ont ou pas importante, de responsabilité sur ce sujet, enfin faut dire il faut appeler les choses par leur nom, les anciens,

ce qu'a dit monsieur Todeschini, je crois qu'il y a une réalité africaine aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'on en soit tous conscients. Qui est la diffusion du terrorisme sur tout le continent africain. On est plus dans la situation de 2013 où il y avait une opération qui a dit ce qui fondait sur qu'on a et et sur Mopti et sur Bamako, ça aurait été grave mais aujourd'hui il y a une dissémination une diffusion du terrorisme soit par Al Al-Qaïda mais directement sous les ordres, Al Qaïda du Moyen-Orient, soit par Daech. Mais pas uniquement au Mali, je reviendrai sur l'évolution, pas uniquement dans le ce qu'on appelle la zone des 3 frontières mais aussi dans le Golfe de Guinée, ça l'a été évoqué par plusieurs d'entre vous, mais au-delà, Boko Haram, Nigeria, Tchad, mais au-delà, la Somalie, les shebab, mais au-delà, le Mozambique, c'est tout récent, et l'inquiétude sur la sécurité devient une âcre études continentale africaine. Et c'est sans doute ça l'enjeu le plus important, donc ce n'est pas entendu monsieur Todeschini dire vous êtes, nous sommes allés nous n'avons pas vaincu le terrorisme, alors le problème, c'est que ça devient un enjeu africain

c'est sans doute. La préoccupation majeure des responsables africains aujourd'hui c'est, c'est le sujet sur lequel elle a été centrée le la dernière assemblée générale de l'Union africaine, il y a 15 jours y a, comme vous le savez, permis l'élection de du président Macky Sall, mais c'est une question majeure pour notre avenir à nous, Européens, qui deviendra aussi majeur dans les semaines qui viennent, que notre sécurité par rapport aux risques venus du Moyen-Orient. Je voudrais faire une 3ème remarque concernant l'intervention d'Alain Richard. C'est vrai que nous avons face à cela, un enjeu considérable de contre-offensive dans le domaine de la formation. Parce que s'il y a une pénétration du terrorisme partout, il y a aussi des offensives de manipulation qui sont menées par certains États. Pas uniquement par les Russes. Par d'autres États ailleurs qui aboutissent à la nécessité d'un partenariat nouveau je reviendrai avec les Africains et qu'il était important de relever la. dernier dernier point, ça revient à vos propos initiaux du président Retailleau sur la difficulté d'agir dans un état quasi faillite, ben oui, c'est un constat et si il y a développement du terrorisme, c'est bien parce que il se développe surtout dans les interstices dans les failles des, des États affaibli non structurées c'est une raison supplémentaire d'accompagner les pays africains dans l'affirmation de leur démocratie et l'affirmation des partenariats avec l'Union européenne, je vais revenir dans un instant. Remarque suivante. Il y a eu sans arrêt, madame la ministre des armées, il y a fait référence, mais je voudrais le rappeler une évolution dans notre posture au au Sahel. à la fois dans notre posture militaire et de notre posture civils. Parce que nous sommes passés d'un engagement à dire à la limite de la substitution à l'armée malienne, c'est le le le début de l'opération Barkhane un engagement de partenariat avec l'armée malienne, puis un engagement plus élargie sur l'ensemble du Sahel avec une logique de soutien au la force conjointe du G5 Sahel logique d'appui renforcement de leurs capacités partenariat réel puis un élargissement de la d'intervention de l'espace d'intervention, puis un élargissement d'européanisation puis une présence internationale de la Minusma et des forces et de forces européennes dans le cas de gluten et de Takuba, progressivement, nous étions toujours dans le mouvement. Toujours soutenu d'ailleurs, je le dis parce que j'entends des des Échos qui semble ne pas relever tout cela se régulièrement soutenu par des résolutions des Nations unies. enfin la mobilisation pour la Minusma faisait l'objet d'un débat annuel, il va encore faire l'objet de la débat à la fin du mois de mai prochain au Conseil de sécurité. Cette mutation et cette agilité d'adaptation se traduit aussi dans le domaine civil, je voudrais rappeler parce qu'il a été fait l'état d'insuffisance de développement, je voudrais rappeler que parallèlement à la mise en oeuvre de l'opération Barkhane après Serval, nous avons lancé avec les Allemands, l'Alliance pour le Sahel. L'Alliance pour le Sahel 25 États, les 5 africains du Sahel, plus 20 partenaires extérieurs, dont l'Allemagne, dont la France, dans des pays européens, c'est présidée par l'Espagne, cette alliance pour le Sahel a permis depuis le de son lancement, c'était en 2014, 2015 de mobiliser 22 milliards d'euros sur l'ensemble de la zone, c'est la mobilisation, c'est pas encore la mise en oeuvre, mais grâce à l'alliance pour le Sahel il y a eu, par exemple, près de 6 millions de sahéliens qui désormais disposent de l'eau potable,

à l'action militaire, mobiliser nos partenaires euro-. En particulier pour que l'Alliance pour le Sahel devienne une réalité, et l'Agence française pour le développement, il y a contribué de manière significative, mais avec d'autres, ce n'est pas uniquement une affaire française il appartient surtout de faire en sorte que lorsque des territoires sont libérés, entre guillemets, de la présence terroriste. Immédiatement, on puisse accompagner le retour de l'État sur les territoires ainsi libéré sans tant qu'on ne le fait pas, on laisse la porte ouverte au retour d'autres terroristes parce que vous avez bien noté que entre Daech et Al-Qaïda, ça ne veut pas, donc la conflictualité entre ces 2 filières terroristes contribue à la diffusion du terrorisme lui-même le le retour de l'État, on revient à l'interrogation du président Retailleau le la présence de l'État, le retour de l'État dans les libérations de territoire est essentiel : le retour de l'État, ça veut dire le retour de l'école. ça veut dire le retour du dispensaire, ça veut dire le retour de du de la sous-préfecture, si on peut utiliser ce terme dans les différents pays pour que l'État reprenne conscience et quand on regarde l'évolution du terrorisme dans les 5 pays concernés. C'est bien là où l'État est revenu. le la sérénité et la paix, a progressé, je pense à la Mauritanie. Il y a quelques années encore, était un pays soumis au terrorisme, de violents, je pense aussi au Niger. Puisque la préoccupation principale du président Bazoum c'est précisément lorsque les forces terroristes se retire immédiatement les l'État puisse reprendre sa place, donc nous sommes dans une logique de transformation permanente de notre action et voilà pourquoi nous, le président de la République a souhaité avec un partenariat avec avec les Européens, avec une discussion avec nos partenaires africains, une réarticulation de dispositif à la fois, civils et militaires et nous sommes en train de travailler à ce que sera ce dispositif à madame la ministre des armées, a évoqué une partie de cette adaptation, sur le modèle militaire pour arriver à une présence sur le terrain plus légère, mieux intégrés aux forces des États qui le demanderont et de ce côté-là, c'est vrai que Takuba a joué un rôle de laboratoire, l'esprit de Takuba. Monsieur le président, comment souffrent toujours. Il se trouve que j'ai eu l'honneur de participer tout à l'heure au conseil des ministres du sous la présidence du chancelier, où j'ai été amené à évoquer les questions liées à ce qu'on l'on évoque maintenant. Et j'ai senti la tension allemande sur la nécessité de poursuive cette ses objectifs de sécurité la la tension allemande du conseil des ministres, donc tout ça est une logique sur laquelle nous devons poursuivre notre sensibilisation pour considérer que le parc. Tenariat avec l'Afrique au niveau militaire était aussi une forme de notre propre sécurité, je rajoute que il faut aussi que nous avons sa gestion modèle civil en développant une approche préventive partout où ce sera possible pour empêcher les régions les plus vulnérables de basculer, ça vaut pour tous les secteurs, que j'ai indiqué tout à l'heure et ça vaut honnêtement plus particulièrement maintenant sur les territoires du Golfe enfin le la partie nord des pays du Golfe, c'est-à-dire l'autre, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin, ils sont demandeurs que nous puissions nous les Européens, je ne dis pas nous uniquement la France que nous soyons, nous les Européens partenaires. De cette stabilisation indispensable en raison de la montée des périls et des menaces sur l'ensemble de de cette de ces régions voilà dans quelle orientation nous sommes. Et nous le faisons dans le cas de la coalition internationale pour le Sahel, parce que il y a une coalition internationale pour le Sahel comme il y a une il y a une coalition internationale contre Daech et cette coalition, elle est composée de 60 partenaires. Essentiellement européens mais aussi des partenaires internationaux des organisations internationales et cette coalition va poursuivre son travail pour en raison de l'ampleur de l'enjeu que que nous constatons dans cette montée en puissance du terrorisme dans cette voudrais terminer mon propos en en rebondissant sur une des observations en particulier du président : comment, mais d'autres aussi sur la nécessité de refonder notre relation avec le continent africain et et ça me paraît indispensable. ce que souhaitent, ce qu'a souhaité initier le président de la République. En faisant en sorte que le 6ème sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine puisse se tenir sous présidence française, ça s'est passé à la fin de la semaine dernière à Bruxelles et je crois qu'a été acté une alliance nouvelle avec le continent africain, en tout cas c'est ce comme cela que cela est apparu qui permet à la fois dans l'Union européenne de de s'affirmer comme 1er partenaire du continent, mais qui permet aussi aux Africains de se mobiliser pour une nouvelle donne de la relation entre l'Afrique et l'Europe nouvelle donne qui puisse permette à à l'Afrique de de rebondir après la pandémie qui intègre les enjeux de souveraineté sanitaire et vaccinale de l'Afrique qui intègre aussi le président Laurent est parti mais je, je pense qu'on lui fera français ce que je vais lui dire maintenant, c'est que la mobilisation des DTS pour l'Afrique, c'est fait. C'est fait depuis le sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine le l'autre jour, la mobilisation des DTS à hauteur de 100 milliards de dollars, c'est acté et c'est une initiative française et l'initiative du président de la République dans cette logique-là, il faut que nous puissions poursuivre les investissements sur les infrastructures, les investissements sur la transition énergétique de juste et les investissements liés à au développement de de d'ensemble agro-écologique agro-écologique reconnue et respectée je ai dit à monsieur Gontard en particulier que un des grands enjeux, va être de faire en sorte que pour le Sahel, ce qu'on a ce qu'on appelle la Muraille verte soit effectivement mises en oeuvre par l'ensemble des acteurs et je suis heureux que le président Issoufou, l'ancien président Issoufou soit considéré comme le leader de cette opération et le manifestera dans un que nous allons organiser dans 10 jours à Montpellier, donc nous sommes sous une nouvelle donne avec l'Afrique se sont une nouvelle donne dans notre relation avec le sel et avec le Mali et dans cette nouvelle donne, je termine sur un notre observation personnelle, je pense que nous ne devons pas abandonner la la population malienne, ni les forces, ville de la société civile malienne à la junte et je veux profiter de cette tribune pour. Leur lancer pendant 10 ans, je me suis mobilisée sur ces populations un un message de soutien et d'amitié, il y avait un très fort qui nous unissent, avec la population malienne, il y a, il y a un très fort qui ont été tissés par l'histoire et par les diasporas maliennes en France et ces Liens, on ne les oubliera pas, en tout cas moi je ne les oublierai pas. Merci monsieur le ministre. Je vais suspendre la séance pour quelques instants afin de permettre à chacun de s'installer pour le prochain point à l'ordre du jour, la séance est suspendue.

La séance est reprise, mes chers collègues, pour la bonne information de chacun, je vous indique que nous suspendrons la séance à 20 heures et qu'elle sera reprise à 21 heures 30 pour la suite de l'examen des 2 propositions de loi à l'ordre du jour l'ordre du jour, appelle à la discussion de la proposition de loi visant à créer une garantie à l'emploi pour les chômeurs de longue durée dans des activités utiles à la reconstruction écologique et au développement du lien social, présenté par Monsieur Patrick Kanner, et plusieurs de ses collègues, c'est une demande du groupe socialiste, écologiste et républicain et dans la discussion générale, la parole est à monsieur Patrick Kanner, auteur de la proposition de loi, Monsieur le Président.

Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, monsieur le Ministre, mes chers collègues, le texte que nous aimons, examinons aujourd'hui, part d'un constat que nous pouvons tous faire, quelles que soient les banques que nous occupons dans cet hémicycle depuis plusieurs décennies, nous avons pris l'habitude de vivre dans une société où le chômage de masse n'est plus une exception et malheureusement la règle. Pourtant, nous le savons, le chômage est un poison lent qui mine nos sociétés qui fait peser un risque toujours plus grand sur notre modèle social tout en favorisant et on le voit encore aujourd'hui le populisme, sur le plan politique autre menace pour notre démocratie. La reprise économique qui fait suite à 2 ans de crise pandémique permet au gouvernement de se réjouir des bons chiffres du chômage au sens du BIT du terme s'il convient de nous féliciter qu'actuellement une partie des Français trouvent du travail plus facilement d'ailleurs souvent en CDD ou en intérim, l'heure n'est pas aux réjouissances comme pourrait laisser penser les déclarations de plusieurs ministres, 659000 demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, toutes catégories confondues a baissé pour les spécialistes en moyenne au 4ème trimestre 2021, le chômage, l'Est, d'un poids trop important, notre société et comment nous réjouir quand nous connaissons déjà les terribles effets de la réforme de l'assurance chômage, votre réforme, Monsieur le Ministre, en tout cas celle de votre gouvernement, en particulier sur les plus précaires, et sur ce que cette réforme a fait basculer dans la précarité, certes pour accompagner la part de la population sans emploi ou en contrat précaire, les mesures d'accompagnement existent et sont nécessaires, nous avions d'ailleurs proposé de lait de les étendre avec le Revenu minimum jeunesse à plusieurs reprises ici au Sénat ou à l'Assemblée nationale et nous sommes, nous sommes malheureusement heurté au mur de la majorité sénatoriale, mais aussi du gouvernement. Pour rejeter notre proposition, vous n'aviez qu'une chose à nous opposer l'insertion par l'emploi. Pour être très clair, changer de trottoir. Comme si l'un exclu et l'autre, ce n'est pas le cas et nous le prouvons aujourd'hui avec cette proposition de loi audacieuse qui posera débat je n'en doute pas, mais qui méritent aujourd'hui d'être étudié avec attention, nous nous attaquons ici au chômage de longue durée qui est synonyme d'exclusion sociale pour les personnes qui sont confrontés et pertes de richesse pour la société sont considérés comme chômeurs de longue durée, toute personne n'ayant pas exercé d'activité durant un an. En 2020 les chômeurs de longue durée représentaient près de 40 % des demandeurs d'emploi en France serait donc pas marginal et ce n'est plus acceptable, redonner la possibilité aux chômeurs de longue durée, d'avoir accès à un emploi et donc une priorité pour éviter qu'il n'atteigne un point de non-retour, point de longs retours qui les condamnent souvent un déclassement social irrémédiable avec cette proposition de loi, nous voulons rendre effectif le droit d'obtenir un emploi, je répète, le droit d'obtenir un emploi qui est présent dans notre Constitution nous proposons donc que l'État puisse garantir ce droit pour les chômeurs de longue durée qui le souhaitent, avec les 2 laboratoires d'idées qui sont hémisphère gauche et l'institut Rousseau, que je salue, que peut-être dans les travées, hé bien, nous sommes partis du constat suivant la pénurie d'emplois ne résulte pas d'un manque de travail, mais d'une organisation du marché du travail qui engendre cette pénurie. Parmi les victimes de cette pénurie, certains se retrouve durablement éloignés de l'emploi, avec son lot de précarité précarité sociale, précarité psychologique précarité sanitaire et cela se reproduit de génération en génération, nous pensons que le rôle de l'État, en concertation avec les territoires avec les élus locaux et de corriger cette injustice et de tout mettre en oeuvre pour que la relégation d'une partie de la population ne soit jamais une fatalité jamais un invariant jamais insolvables, nous proposons ainsi avec mon groupe à chaque personne au chômage depuis plus d'un an et qui en fait la demande, une offre d'emploi à temps choisis, payés au SMIC horaire, ces employes donne les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'un CDI classique l'objectif ici est de fournir un emploi toutes les personnes durablement exclus du marché du travail, si ce dispositif croit en l'émancipation par le travail il n'impose rien. Cela permettra d'éviter à une partie de la population de s'enliser dans la trappe à pauvreté qu'est le chômage de longue durée et augmentera les possibilités pour les personnes concernées par ce dispositif de pouvoir ensuite rebondir, rebondir vers un emploi mieux rémunéré, voilà un dispositif d'insertion par l'emploi que vous devriez soutenir monsieur le ministre, si vous étiez finalement cohérent avec vos propositions, oui, pour répondre à la potentielle demande il nous faudrait créer mes chers collègues, un 1000000 d'emplois, j'entends déjà ici le procès en utopie. Ils n'ont pas lieu d'être par car notre proposition permettra de créer un 1000000 d'emplois pour un coût inférieur inférieur aux politiques de lutte contre le chômage, existence, j'y reviendrai. Je profite de mon intervention pour saluer le travail du rapporteur Jean-Luc Fichet ici présent et signaler que mon groupe reprendra reprendra les amendements qu'il avait déposée mais malheureusement rejeté en commission et qui améliore sensiblement le texte sur plusieurs points, pour arriver à notre objectif, nous rendons possible une montée en charge des dispositifs de contrats aidés existants dans les secteurs marchands et non marchands et nous développons l'insertion par l'activité économique, chers collègues, nous avons également souhaité nous appuyer sur la fameuse et juste expérimentation territoire zéro, chômeur de longue durée portée par notamment l'ancien député grand Guillaume, qui a fait ses preuves et qui est reconnu par tous tous les acteurs sur le territoire après avoir échangé avec l'association plutôt que de généraliser l'expérimentation de manière anticipée à travers un dispositif pérenne, nous souhaitons supprimer le plafond d'extension à 60 territoires afin de permettre à tous les projets partenariaux territoriaux existants, il y a venir d'intégrer de l'expérimentation qui est ainsi portée s'il respecte bien sûr le cahier des charges de l'association, nous proposons également de simplifier l'habilitation de nouveaux territoires par la prise d'un simple arrêté préfectoral, un amendement sera présenté en ce sens, la question de la formation sera aussi à leur prise en compte, grâce à cette alimentation, ensuite parce que nous pensons que l'État et les collectivités doivent s'engager dans une démarche innovante permettant d'adapter réellement l'emploi, la transition écologique nous avons orienté notre texte vers un déploiement d'emplois dits pour embarquer tous les citoyens dans la dynamique de transition écologique et faciliter de son acceptation sociale, l'État doit pouvoir offrir aux Français des perspectives et opportunités nouvelles, notamment en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi aujourd'hui, nous considérons que cette approche inclusive et solidaire est le préalable à toute transition écologique d'envergure parmi ces emplois vers les Échos activités qui produisent des biens ou services ayant pour finalité la protection de l'environnement ou la gestion des ressources mobilisées aujourd'hui virgule 8 % de l'emploi en France, c'est bien trop peu, elle concerne l'agriculture biologique, la protection de la nature des paysages de la biodiversité. Le recyclage, la récupération des eaux de la recherche, le développement ou encore l'ingénierie des énergies renouvelables, de nouvelles compétences, mes chers collègues vont et tant mieux se déployer dans les prochaines années à nous de les encourager, mais déjà un certain nombre d'emplois peuvent être rapidement créée localement en fonction des besoins identifiés dans chaque bassin de vie, enfin je parlais tout à l'heure du des procès en utopie qui ne manqueront pas de fleurir comme toujours quand on propose un dispositif novateur peut se parfois souvent se heurter au mur du conservatisme, mais je l'affirme ici le financement de cette garantie à l'emploi ne poserait aucun problème, à terme, cela permettra même d'économiser de l'argent public, moi je suis ministre, l'ONG ATD-Quart Monde, a estimé en 2015, les coûts du chômage, d'exclusion, le chômage de longue durée à 36 milliards d'euros par an pour la puissance publique amorcer le financement de c'est un 1000000 d'emplois verts coûterait moins de la moitié de cette somme, permettez-moi de le dire, à comparer aux 137 milliards d'euros de profits enregistrés par les groupes du CAC 40 en 2021 dernière information en date, en supprimant la flat tax que vous avez créée en créant un impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, en annulant la baisse de 10 milliards des impôts de production du plan de relance, qui représente 10 du plan de relance souhaitée par le gouvernement et en augmentant le taux de la taxe sur les transactions transaction financière, hé bien nous de donnons les moyens d'enclencher cette dynamique vertueuse, à terme, cette garantie l'emploi sera financé par la puissance publique, notamment à travers de l'activation des dépenses liées au chômage, c'est à dire par la transformation des allocations et des aides sociales que perçoivent les chômeurs en salaire, c'est le meilleur moyen, mes chers collègues, de lutter contre le soi-disant assistanat si utilisé dans la bouche de certains de nos collègues ici présents pour conclure depuis 40 ans, les politiques de lutte contre le chômage, présente un bilan décevant et n'ont pas permis d'éradiquer le chômage de longue durée avec cette proposition audacieuse sociétal vertueuse offrons la possibilité de sortir de cette ornière, mes chers collègues, je vous invite à ne pas laisser passer cette opportunité et je vous en remercie. Si Monsieur le Président. Parole établissent Jean-Luc Fichet. Rapporteur de la commission des affaires sociales. Madame. La présidente. Monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, la création d'une garantie à l'emploi pour les chômeurs de longue durée, vise à donner une portée concrète au droit d'obtenir un emploi programmées proclamé par le préambule de la Constitution de 1946 rendre effectif ce droit nécessite non seulement de créer des emplois, mais aussi d'aller à la rencontre des personnes qui en sont privés, de les accompagner vers et dans l'emploi et d'assurer leur formation professionnelle, la privation d'emploi ne se réduit pas à la catégorie administrative de demandeurs d'emploi de longue durée, qui rassemble 2 6 millions de personnes, selon l'Insee, elle concerne de nombreuses personnes découragées ou invisible qui n'apparaissent pas dans les chiffres du chômage, l'ampleur de ce phénomène sa persistance et ses conséquences sur notre cohésion sociale justifie que tout soit mis en oeuvre pour l'éradiquer. à cette fin, la proposition de loi déposée par le président Patrick Kanner, et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain mobilise plusieurs outils existants, relevant de l'économie sociale et solidaire qui ont vocation à jouer un rôle complémentaire. Premièrement, les contrats aidés concernent des personnes connaissant des difficultés d'accès à l'emploi mais pouvant être orientés directement vers un milieu ordinaire de travail l'employeur recevant alors une aide à l'insertion professionnelle pendant une durée limitée. unique d'insertion le contrat unique d'insertion, ils prennent la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi dans le secteur non marchand et du contrat initiative emploi dans le secteur marchand. Ces contrats ont plus souvent été utilisé comme outil conjoncturel de réduction du chômage que comme véritable solution à la pluie, des politiques d'insertion afin de donner à ces contrats toute leur place dans la mise en oeuvre et de la garantir l'emploi et d'éviter l'alternance de mesures de freinage de relances qui compromet leur mobilisation rapide en période de crise, l'article 3 fixe à compter de 2023 un nombre minimum de 200000 contrats aidés dans le secteur non marchand et l'article 4 prévoit un minimum de 50000 contrats aidés dans le secteur marchand, deuxièmement l'insertion par l'activité économique, vise à faciliter l'insertion professionnelle de personnes éloignées de l'emploi pendant une durée limitée, en principe à 24 mois au moyen de modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement au sein de structures spécialisées, le S. I. A. E. Il y a, est devenue un instrument central des politiques de l'emploi mais les ambitions quantitatives affichée par le gouvernement : atteindre 240000 postes dans l'ensemble de et s'il y a eu à la fin du quinquennat reste encore très largement théorique. Afin de soutenir le développement du secteur, l'article 2 impose à compter de 2023 un minimum de 100000 contrats au sein des entreprises d'insertion. l'expérimentation territoire zéro, chômeur de longue durée constitue dans les territoires concernés, la solution du dernier ressort la voiture balai de la garantir l'emploi. Initié en 2016 cette expérimentation permet à des personnes privées durablement d'emploi d'être embauchés en contrat à durée indéterminée à temps choisi au sein de l'entreprise à but d'emploi les EBE en postulant que personne n'est inemployable et en visant l'exhaustivité, elle apparaît aujourd'hui comme la nouvelle frontière du développement des politiques de lutte contre le chômage d'exclusion. L'article 1er, prenant acte du succès de cette expérimentation vise à la pérenniser sans attendent 2000 26 et à accélérer son extension. Le nom de territoires participants seraient quintuplés tous les 2 ans, dans la limite des collectivités volontaires et du nombre de territoire encore non couverts, sa cible seraient également élargi aux personnes âgées de moins de 25 ans priver durablement d'emploi depuis 6 mois et de et domicilié depuis au moins 3 mois dans l'un des territoires participants. Nous avons cependant entendu les réserves des acteurs de l'expérimentation avec lesquels nous avons eu des échanges approfondis. Pour respecter le caractère de projet expérimental et la démarche du territoire au coeur de territoires zéro, chômeur de longue durée, il souhaite opportun de remplacer ces dispositions par une suppression du plafond actuel de son territoire auquel il ne peut être dérogé que par un décret en Conseil d'État ainsi. Tous les projets émergents remplissant les conditions du cahier des charges pourraient être admis sans plus attendre dans l'expérimentation par arrêté du ministre chargé de l'emploi. La proposition de loi vise également à orienter cet investissement en faveur de l'inclusion de chômeurs de longue durée vers des activités contribuant à la lutte, la crise environnementale. Cette orientation n'apparaît pas contradictoire. Ali à eux il y a depuis longtemps investi des activités liées au développement durable, tels que la gestion des déchets. De même, dans les territoires zéro, chômeur de longue durée, la transition écologique représente 38 % des activités des EBE. Afin de systématiser cette approche. L'article 3 prévoit que les aides au titre d'un contrat unique d'insertion ou d'un contrat d'action par l'économique ne peuvent être accordées que si le contrat porte sur des activités ayant pour finalité la protection de l'environnement ou la gestion des ressources. Concernant les contrats aidés dans le secteur marchand, l'article 4 conditionne l'aide au poste à la Halle atteinte par l'employeur de la neutralité carbone ou à son engagement dans la décarbonation de ses activités. Je considère que cette orientation est souhaitable si elle reste souple et ne conduit pas à limiter le développement de ces contrats. Je veux rappeler que l'expérimentation territoire zéro chômeur et plus généralement la garantie à l'emploi pour en elle-même la chance de son propre financement, en effet, le chômage de longue durée représentent pour la collectivité, un coût de plus de 30 milliards par an au titre ou des sols, des allocations chômage. Sans compter ses conséquences en matière de consommation de dépenses sociales et de recettes fiscales et sociales lutter contre ce fléau qu'est la privation d'emploi, c'est donc à terme générer des économies substantielles, pour autant, en parallèle du dispositif ambitieux qu'elle propose et dans le souci d'en assurer le financement, la proposition de loi contient un projet de réforme fiscale de grande ampleur à même d'entraîner un surcoût un surcroît de recettes fiscales de 10 à 11 milliards d'euros. J'ajoute que les 4 piliers sur lesquels repose cette réforme contribuerait en outre à la résorption des inégalités économiques et sociales dont la croissance constitue en période de sortie de crise, plus encore que jamais un obstacle fondamental à la convergence de toutes les énergies et de la cohésion nationale. La première de ces réformes consistent en l'annulation d'une partie des mesures de baisse des impôts de production intervenue en 2021 ces dispositions se sont avérés utiles pendant la crise sanitaire, il n'est pas juste que toutes les entreprises en ait bénéficié, même celles qui génèrent des profits importants toute en contribuant au réchauffement climatique. Nous 5 qui prévoit leur annulation permettrait donc d'associer les entreprises au financement de la solidarité nationale autour de 7 milliards d'euros, ce qui se justifie tout particulièrement à l'heure où la croissance atteint des niveaux sans précédent 2ème réforme la position des grandes fortunes en la matière, l'article 6 prévoit le rétablissement de l'ISF, sous la forme d'un impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, pour mémoire, ce gouvernement a supprimé l'ISF en 2018, il lui a substitué les filles qui ne repose que sur des biens immobiliers dans le but d'inciter à l'acquisition de titres de capital d'entreprise française plutôt qu'à la rente immobilière au terme de mes auditions, il est apparu qu'aucune étude ne permettait pour l'heure, d'affirmer que cet objectif a été atteint, bien au contraire, à ce jour, une seule chose est certaine : la suppression de l'ISF a largement profité aux plus riches, l'article 7 prévoit en outre de supprimer le prélèvement forfaitaire unique créé en 2018 est devenue l'option par défaut pour la position des revenus du capital, enfin dernière réforme fiscale et non des moindres, l'instauration d'une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévues à l'article 8 pourrait permettent de générer des recettes supplémentaires à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros, il s'agirait là d'une juste contribution des marchés financiers au financement de la lutte contre le chômage de longue durée, d'autant plus légitime que leur bonne santé ne s'est jamais démenti depuis le début de la crise sanitaire face à l'urgence sociale et la crise environnementale, nous devons parvenir à articuler les enjeux du droit à l'emploi de la transition écologique et de la justice fiscale sans les opposer la commission des affaires sociales n'a pas adopté ce texte, ce que je regrette, je vous invite à titre personnel a voté cette proposition de loi, je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail.

madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, monsieur le président, Kanner mesdames et messieurs les sénateurs, le groupe socialiste, écologiste et républicain présente aujourd'hui sa proposition de loi visant à créer une garantie à l'emploi pour les chômeurs de longue durée avec une précision dans les activités utiles à la reconstruction écologique et au développement du lien social, alors évidemment je voudrais d'abord vous dire que. Je partage le gouvernement partage votre diagnostic sur la nécessité de donner à chacun, sans exception, opportunité d'accéder à un emploi pour trouver sa place dans la société, d'ailleurs je pense que ça fait partie de ce qui doit nous réunir assez largement tous dans cet hémicycle. J'en veux pour preuve, même si j'ai compris, Monsieur le Président Carter que vous n'aviez pas trouvé que ce bilan était suffisamment positif mais malgré tout, permettez-moi en matière d'emploi de de souligner quelques éléments d'émancipation pour le travail a été du 1er au dernier jour du quinquennat au coeur de nos préoccupations et des réformes qui ont été mises en Oeuvres. Je voudrais être clair dès le début de mon intervention et vous dire que même si je partage votre diagnostic, je suis en désaccord et le gouvernement est en désaccord avec votre proposition qui pourrait, moi je le crois plutôt fragilisé la situation de l'emploi en déstabilisant les acteurs et en détricotant des réformes majeures. Nous partageons donc l'objectif d'autres textes, mais pas les moyens. Pour y parvenir, tout d'abord sur la pérennisation et l'extension progressive à tout le territoire, l'expérimentation territoire zéro, chômeur de longue durée, cela nous sommes prématuré, vous l'avez défendu monsieur le rapporteur avec vigueur et sur le fond, encore une fois, nous partageons l'intérêt de cette expérimentation, puisque nous-mêmes nous l'avons portée je crois que cela a été assez largement emporté, y compris dans cet hémicycle, moi je crois qu'il faut simplement respecter ce qui est prévu dans ce texte sur l'expérimentation en 0 chômeur et ne pas aller plus vite que la musique, nous avons une loi du 14 décembre 2020 quand même relativement récente et je crois que nous avons là déjà des éléments d'extension l'expérimentation à 50 nouveaux territoires dans cette loi, je crois que il faut traiter cela avec la progression, mais aussi il y avait besoin pour ce sujet du territoire zéro chômeur de pouvoir à chaque fois construire et sur le territoire, l'impact les conséquences, la performance de ce dispositif, nous avons déjà 9 territoires, de plus, dans l'esprit et dans les faits, sur ce que vous souhaitez, ce rythme de montée en charge, moi je crois qu'il ne doit pas se faire au pas de course, j'allais dire au pas de charge, ne doit pas faire au détriment de la qualité des parcours des personnes et des projets de territoire, moi, d'ailleurs je, je sais qu'ici, devant cette assemblée on on sait ce que ça que les territoires, on fait aussi le temps qu'il est parfois nécessaire de prendre pour faire réussir sur son territoire de telles expérimentations. Ensuite, sur la création de 100000 contrats supplémentaires relevant de l'insertion par l'activité économique d'ici à 2023, j'ai envie de vous dire mais nous partageons aussi cet objectif, il est mais j'ai presque aussi envie de vous dire mais j'ai l'impression que vous partagez l'objectif mais vous ignorez les efforts qui ont déjà été engagées votre article 2 propose de développer le nombre de parcours d'insertion, alors que cette démarche sur le fond, on est déjà au coeur de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, cette stratégie prévoit d'accueillir plus de 100000 un nouveau bénéficiaire dans l'insertion par l'activité économique entre 2018 et 2022, et de les orienter vers les métiers en tension. Pour atteindre à cet objectif, malgré la crise, nous avons fortement soutenu ce secteur, si bien que la moitié du chemin a déjà été parcouru avec 55000 personnes accompagnées supplémentaires sur l'année 2021 par rapport à 2017. Si je regarde mon département du Nord, mais nous le partageons avec Monsieur le Président Kanner qui connaît bien Vitamine T, un des leaders français de l'insertion par l'activité économique, où je suis moi-même, comme vous, je suis allé plusieurs fois, ils ont eux déjà fait évoluer cette réalité avec je, regardez les chez eux 3349 salariés en parcours d'insertion. Donc je je donne cet exemple là parce que je crois qu'il est d'abord très vivant dans dans mon département et la région, et en plus qui il est connu aussi d'un certain nombre de de sénateurs qui peut-être aussi dans leur territoire, ont ce même type de référence et si je veux juste agrandir un petit peu le spectre quand je regarde ce que fait ce que porte Brigitte Klinkert ma collègue de l'insertion 400 millions d'euros ont été alloués aux structures d'insertion par l'activité économique pour les aider, d'une part à surmonter la crise sanitaire et d'autre part à se moderniser, à se positionner sur des secteurs porteurs, comme par exemple le BTP, les métiers du numérique, les hôtels, cafés, restaurants, mais évidemment pas que les métiers de transition écologique que vous avez évoquée. je, je vous dis clairement d'initiatives sont d'ores et déjà lancée pour continuer de sécuriser cet objectif de 100000 bénéficiaires supplémentaires en 2000 22 et les dispositifs que nous mettons en place, je crois que permettent de dire que l'objectif est déjà rempli donc pas nécessaire d'inscrire dans la loi, puisque à une unique exception près pendant la crise sanitaire, le nombre de personnes en parcours on y E sur un mois, n'est jamais tombé sous la barre des 100000 depuis 2017 votre objectif, j'allais dire, est déjà atteint. Enfin, le recours aux contrats aidés ne nous semble pas le levier le plus approprié pour développer les emplois verts dans les secteurs public et privé, j'ai bien noté d'ailleurs sur le rapporteur, ce en quoi projet de loi que vous présentiez pouvait chercher à louer des objectifs qui sur le fond sont intéressantes poursuivent et que nous poursuivons, alors vous voulez, ce qui est de faire une sorte de synthèse pour le coup, suis vous voulait sourire avez vous, je veux dire, vous essayez de faire du et en même temps sur ce sujet, mais sur le fond, moi je crois que là-dessus, nous avons déjà des objectifs très clairs, si on regarde les le revendique le 3 et 4 que vous proposez. Vous vouliez adapter l'emploi, la transition écologique, créant 200000 contrats aidés, c'est c'est lui CAE au sein de l'économie sociale et solidaire dans les collectivités, les associations, c'est vrai, et 50000 contrats aidés dans le secteur marchand. Bon, je crois que ces aides comme de simples subventions encourageant la mise en oeuvre et la transition écologique serait à mon à mon avis un très clairement une forme de dévoiement des contrats aidés et d'ailleurs je crois en tous les cas avec certains, certains d'entre vous, ici, moi j'ai eu, on a eu à à échanger, à discuter, lorsque nous avons nous-mêmes transformer un certain nombre de dispositifs de contrats aidés, notamment vis-à-vis des collectivités locales et territoriales qui se sont inquiétés, à un moment donné, de trouver des ressources et nous avons à plusieurs reprises aussi discuter sur l'importance de l'accompagnement et la nécessité d'être dans un métier de demain, c'est pour ça que nous nous avons choisi l'ensemble des métiers en tension. Moi je crois qu'il ne faut pas courir plusieurs lièvres à la fois pour je ça cela serait au détriment de l'activité des acteurs engagés dans l'insertion des plus éloignés de l'emploi, c'est pourtant cela que vous vivez en réalité, nous pensons qu'il est possible de mener de front les 2 combats mais sans confondre les outils, monsieur le rapporteur, c'est peut-être en cela que nous divergeons l'insertion du public et l'emploi et la réussite de la transition écologique, certains employeurs ont déjà d'ailleurs recours aux contrats aidés quand il le souhaite développer, c'est vrai, leur engagement en matière écologique, c'est déjà le cas aujourd'hui, c'est possible. D'autres utilisent des outils différents, moi, je pense notamment au service civique, qu'est ce que je je devrais répondre aux maires de mots territoire qui aujourd'hui a recours à un service civique pour ce type d'activité, il serait plus il devrait prendre un un autre type de contrat, moi je pense qu'il faut garder de la lisibilité à ce dispositif pour assurer l'adaptation des emplois aux nouvelles compétences sont c'est vraiment nécessaire, notamment par la transition écologique ont par ailleurs mis en place, je crois, moi, des outils qui sont plus adaptées, je vous donne juste quelques chiffres mais vous les avez en tête ce que nous avons mis sur la table au niveau du gouvernement pour accompagner dans les compétences, les demandeurs d'emploi que près de 15 milliards engagés au titre des plans d'investissement sur les compétences, je pourrais aussi vous dire et je sais que vous le percevez aussi le plan de réduction des tensions de recrutement qui est doté d'une enveloppe très significative 1,4 milliards d'euros pour soutenir en particulier, le développement des formations associées à une promesse d'embauche dans les secteurs en tension que j'évoquais tout à l'heure, ce plan d'ailleurs porte une attention particulière et là aussi je reviens sur votre objectif, monsieur le rapporteur. Vous avez cette volonté, je la sens de votre expression de proposer quelque chose aux demandeurs d'emploi de longue durée, mais c'est ce que nous portons avec ce plan de réduction des tensions de recrutement puisqu'on peut nous les accompagnons, à la fois par une aide vis à vis des entreprises mais aussi 2000 euros pour les demandeurs d'emploi de longue durée qui se forment aux métiers en tension, on a bien son regard là pour le coup du en même temps et vis-à-vis de l'entreprise avec une aide de 8000 euros et vis-à-vis du demandeur d'emploi qui est accompagné, récompenser aussi de son engagement pour le travail, enfin la commande publique et privée, me semble être un levier de transformation plus efficace pour les ados, mais j'ai eu l'occasion d'en débattre avec certains d'entre vous, notamment dans des campagnes électorales précédentes, notamment dans le cadre des nouvelles obligations des clauses sociales et environnementales imposées par la loi du 22 août 2021 dite qui m'a et résilience, moi je pense que là-dessus, en la matière, les collectivités locales territoriales régionales ont un rôle à jouer et je pense aussi que ce sujet est partagé assez largement sur ces bancs, voilà je voudrais terminer sur votre titre de très rapidement parce que, évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vois que c'est plus ça détricotage de ce peut-être ce qui ne vous convient pas dans ce que nous avons porté jusqu'à maintenant, évidemment, vous comprendrez, monsieur le rapporteur, que je ne serais pas favorable à à tout cela et je évidemment vous demanderai en tous les cas, ce sera la position du gouvernement de ne pas adopter cette proposition de loi, je vous remercie. Merci monsieur le ministre. Mes chers collègues, avant de suspendre la séance, j'ai une communication à vous présenter, conformément aux dispositions du 5ème alinéa de l'article 13 et à celle de l'article 56 de la Constitution, la commission des lois a fait connaître qu'elle a émis lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable à la nomination de Monsieur François ces 20 voix pour, une voix contre et un avis défavorable à celle de Madame Jacqueline Gourault, 12 voix pour, 16 voix contre aux fonctions de membre du Conseil constitutionnel, par ailleurs, en application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique et de la loi ordinaire du 23 juillet 2010 prises pour son application, elle a émis un avis favorable 28 voix pour, une voix contre à la reconduction de Monsieur Julien Boucher aux fonctions de directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 21 heures 30 pour la suite de l'examen de ce texte, la séance est suspendue.